La séance est reprise avec l'dit. Ils on de la proposition de loi relative à la maîtrise de l'organisation algorithmique du travail. Proposition présentée par Monsieur Pascal Savoldelli et Madame. Si pour se. Laurence Cohen et plusieurs de leurs collègues hein dans la discussion générale. Nous sommes parvenus à l'intervention de madame Jocelyne Guinness pour le groupe Union centriste. Guider, vous avez la parole.

Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure mais c'est cher collègue. Tout d'abord je tiens à remercier monsieur Pascal ça vaut. Pour son engagement et notre collègue rapporteur Madame Katia pour se polie pour la qualité de son travail. Cette proposition de loi visant à encadrer le recours aux algorithmes et la numérisation des relations de travail. Il s'agit de renforcer la responsabilité des employeurs et la protection des salariés. Cette initiative parlementaire s'inscrit dans le prolongement du rapport d'information de Pascal ça vous du 29 septembre 2021. Sur l'ubérisation de la société et l'impact des plateformes numériques sur les métiers et le marché de l'emploi. Selon cette mission d'information, elle tend à remettre en cause notre modèle social et économique en l'imposant en effet à leurs travailleurs, les pratiques du management, alors qu'il serait nécessaire de mieux les encadrer. Des recommandations sont ainsi formulé autour de 4 grands axes, l'amélioration des conditions de travail, le développement du dialogue social, l'encadrement du management, ainsi que la transparence et la régulation des algorithmes, des plateformes. Antérieurement. Ce rapport, la proposition de loi relative au statut des travailleurs a été rejeté par notre assemblée en juin 2020. Notre collègue Madame Catherine Fournier souligné alors que la transformation de la relation commerciale du travailleur indépendant de plateforme et on en comptera relevant du droit du travail centré sur les plateformes de service était trop restrictive et vous et fi de la diversité de celle-ci. J'appelle aussi votre attention sur le travail réalisé par notre collègue Bruno Retailleau. Une proposition de loi déposée en août 2022 relatives aux travailleurs en station de dépendance économique vis-à-vis des plateformes numériques. Ce texte met l'accent sur le développement du numérique a donné naissance ça de nouvelles formes d'organisation du travail. L'émergence de ces dernières a permis l'accès à l'emploi des personnes qui ont été parfois éloignées. Les profits de ces travailleurs sont variés anciens chômeurs, étudiants, actifs, souhaitant compléter les revenus d'un emploi salarié. La question de leur protection est aussi abordée par une réflexion sur leur statut. Cette proposition de loi s'appuie notamment sur les conclusions d'un rapport de la commission des affaires sociales. En mai 2020 travailleurs de plateformes au-delà de la question du statut. Quelle protection. De Madame, Frédérique Puissat, monsieur Michel Forissier Madame Catherine Fournier, il a estimé nécessaire de dépasser ce débat sur le statut de développer des droits et une couverture sociale indépendante de ce dernier. Le texte de Bruno Retailleau vise en effet à mettre en oeuvre cette recommandation. Ne touche pas au régime des travailleurs indépendants mais créer un nouveau type de contrat sur mesure qui permettra aux travailleurs de bénéficier d'une protection sociale améliorée de mesures de prévention en matière de santé, ainsi que de garanties sur la transparence du fonctionnement des algorithmes. Ces différents travaux menés au Sénat témoigne de l'intérêt de ce sujet. Ces initiatives parlementaires mettent en lumière la nécessité de mieux connaître ce phénomène qui présente tout un spectre d'activités et de citations sociale. Né dans divers secteurs des mobilités la plateforme hésitation s'étend désormais à l'ensemble de l'économie. Elle se traduit par une explosion du nombre de travailleurs de plateforme 28 millions de personnes dans l'Union Européenne aujourd'hui 43 millions en 2025, selon les estimations. Cette nouvelle façon de travailler, nécessite un nouveau regard sur les conséquences de son amplification et nous impose de réorganiser le dialogue social dans un contexte où les discriminations se développe, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate. Force est de constater que ces personnes souvent précaires isolé et contraint de recourir à ces formes d'emploi cumul des fragilités faiblesse des rémunérations protection sociale incomplète Exposition aux risques professionnels soumise à un degré élevé de contrôle. Elles peuvent ressentir un sentiment de dépendance à l'égard des plateformes. Nous défendons l'idée d'un travail décent dans le monde en ligne pour lutter contre les effets discriminatoires. Il nous semble important que la chaîne de responsabilités soient. Comme humaine, même si le fonctionnement repose sur ce sur les algorithmes. Allemands les algorithmes doivent être contrôlés, encadrés puisqu'ils sont utilisés à des fins de gestion des ressources humaines d'organisation du travail et de recrutement. Notre groupe approuve la démarche parlementaire consistant à proposer des améliorations aux conditions de vie et de travail des travailleurs de plateformes et diminuer ainsi leur Exposition au risque. Certes, nous ne pouvons pas voter contre cette proposition de loi qui vise à améliorer la transparence de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi qu'à responsabiliser les employeurs. Toutefois, chers collègues, nous savons qu'au niveau de l'Union européenne une proposition de directive sur la reconnaissance d'une présomption irréfragable de salariat pour certains de ces travailleurs est en cours de négociation, il est nécessaire que ces travaux aboutissent. Par conséquent, il nous semble prématuré de légiférer sur ce sujet avant que se concrétise. Les résultats de ces travaux. Prendre cette précaution nous paraît logique puisque notre travail législatif risque d'être détricoté à l'avenir. La prise en considération de la dimension européenne constitue une étape importante dans la construction de solutions concernant l'amélioration des conditions de travail. Ce combat au niveau européen tracera à de nouvelles perspectives pour aborder cette thématique qui occupera certainement une place importante dans les débats sur les droits sociaux des travailleurs dans les prochaines années. Pour l'ensemble de ses arguments. Le groupe Union centriste, ça se tiendra je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Corbisez pour cinq minutes pour le groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre. Madame la rapporteur monsieur le vice-président de la commission. Mes chers collègues. Le développement technologique a longtemps été associée à la notion de progrès. Et force est de constater qu'il a pu être porteur d'avancées réelles dans de nombreux domaines socio-économiques y compris dans le monde du travail. Néanmoins, il l'emporte aussi son lot d'inquiétudes et de questionnement. Dès lors qu'il percute les droits des salariés ou interfèrent avec les conditions de travail ou les process de recrutement à l'image de la récente polémique autour du groupe Amazon dont l'algorithme d'analyse des candidatures favoriser au final, celle des hommes. Quel humour ça plan Amazonie. Les débats sont d'ailleurs danse actuellement sur les risques que porte en soi la progression exponentielle de l'Intelligence artificielle qu'il s'agisse de son fonctionnement désincarnée ou des abus potentiels de son usage. Est évidemment est absolument pas recevable l'argument qui consiste à dire que l'outil est par nature innocent et que ce sont les usages qui peuvent être détournées. Il est au contraire de la responsabilité des concepteurs de garantir toutes les sécurités du d'utilisation et de celle du législateur de fixer le cadre d'exercice de cette responsabilité. C'est précisément ce que les ai proposé de faire dans cette proposition de loi déposée par nos collègues du groupe CRCE. Certes, la commission n'a pas adopté le texte au motif qu'il n'apporterait pas de garanties supérieures aux salariés et que des travaux du même ordre sont en cours au niveau européen. Et alors pourquoi attendre l'Europe. Je crois pour ma part que lorsqu'il s'agit de la relation au travail, les garanties et protections des salariés mérite toujours d'être interrogé renforcer d'autant plus dans un contexte où les discussions européennes semble pour le moment assez mal engagé. gardant en mémoire que l'économie des plateformes concernera d'ici 2025, 43 millions de salariés. Au de des plateformes nombres d'entreprises ont aujourd'hui peut le virage numérique avec les objectifs affichés d'améliorer leurs processus d'organisation de simplifier et d'accélérer leurs moyens d'action ou encore d'optimiser la gestion du travail. L'informatique peut certes aider mais n'oublions pas que derrière ces logiciels et ces algorithmes. Il a des programmateurs qui paramètres sur leurs outils en fonction de consignes ou commande qu'on leur donne. La décision automatisée, d'autant plus dangereuse qu'elle prise par nature de façon opaque et qu'elle peut reproduire à l'envie des comportements discriminants avec le risque d'une standardisation des décisions. Cela est d'autant plus inquiétant que pour les. Il a dit prenantes capable d'acquérir une autonomie croissante et dont le fonctionnement devient complexe à expliquer, voire difficile à maîtriser. Partant de là, il me semble pertinent, comme le formule l'article 1 de la proposition de loi de clarifier la nature juridique du recours à l'algorithme comme une expression du pouvoir de direction et compte de contrôle de l'employeur, traduisant ainsi l'une des conclusions de la mission d'information sénatoriale consacrée à l'uberisation de la société. Même si automatique ah visible une décision issue d'un traitement automatisé n'emporte pas moins des conséquences pour le salarié et celui-ci doit être en mesure d'une part de se défendre face à une décision qui lui est défavorable et d'autre part de la contester, si elle est l'expression d'une discrimination. De ce point de vue contraint de l'employeur a apporté la preuve que son algorithme n'est pas discriminatoire va dans le bon sens. Enfin la proposition de loi s'attaque au sujet épineux des plateformes et du lieu de subordination qu'elle impose à ses collaborateurs présenté souvent à tort comme indépendant. Or le plus souvent ils n'ont que peu ou pas de maîtrise sur la gestion de leur mission ni sur la fixation de leurs tarifs. Comme ils ne peuvent pas véritablement négocier leur contrat ni contester les sanctions qui leur sont appliqués. Il s'agit ici sans attendre l'issue des négociations européennes et avec la préoccupation de protéger les salariés de ces plateformes d'intégrer dans notre droit du travail. Les juristes prudences Hubert Deliveroo et Élite taxi. Au-delà, cette définition permettra de niveler les responsabilités entre les employeurs lambda. Elle est conforme. Lesquels ont trop souvent exploité les failles du vide juridique les concernant. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues. Notre groupe est favorable à cette proposition de loi, je vous remercie. Merci la parole est maintenant monsieur Serge Babary pour le groupe Les Républicains pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales. Madame la rapporteure. Mes chers collègues. Un certain humanisme à la française assez largement partagé. Qu'il soit d'origine religieuse ou laïque. Il nous a toujours fait considérer avec inquiétude et circonspection l'intrusion d'automatismes dans les relations interpersonnelles dans le monde du travail. Souvenons-nous de l'essai de Georges Bernanos. La France contre les robots. Qui dès 1947 formulé une violente critique de la société industrielle. Estimant que le machinisme limiter la liberté des hommes et perturbé jusqu'à leur mode de pensée. L'actualité concernant les nouvelles formes d'emploi freelance micro-entrepreneurs salariés porté et les modes d'engagement particuliers sur les plateformes numériques, nous interpelle. Il s'agit d'accompagner et sécuriser le grand mouvement de fonds en faveur de ces nouvelles formes d'emploi et il apparaît urgent d'examiner l'ensemble des composantes du travail indépendant pour révolutionner notre pacte social et adapter notre système à ces transformations. Il convient de réinterroger le dispositif actuel de protection sociale dans leur contenu. Leurs équilibres et dans leur application. Il est vrai que la tentation d'une uberisation sociale à partir de l'organisation algorithmique du travail à dévoyé ces perspectives. Cependant aujourd'hui plus de 28 millions de personnes dans l'Union européenne travaille pas intermédiaire de plateforme de travail numérique en 2025. Ce nombre devrait atteindre 43 millions de personnes. C'est un secteur particulièrement dynamique et innovant. Entre 2016 et 2020 les revenus de l'économie des plateformes ont ainsi été multiplié presque par 5. Passant d'un montant estimé à 3 milliards d'euros à environ 14 milliards d'euros. Les conditions d'emploi, les travailleurs des plateformes suscite de nombreuses inquiétudes partout dans le monde. Elles sont liées à leur statut juridique sont-ils salariés en contractant indépendants donc responsables de leur propre assurance sociale et exerçant un contrôle sur leurs revenus. L'issue de cette controverse leur protection sociale n'est pas anodine. Le débat juridique, économique et social et donc vif en Europe, les États ont apporté des réponses différentes, soit par la loi, soit par la jurisprudence. Par ailleurs, le développement de management par algorithme soumet les travailleurs à une pression constante et un contrôle intrusifs. La première objection à cette proposition de loi et son caractère prématuré puisqu'une proposition de directive européenne est discuté depuis le 10 décembre 2021. Elle vise à garantir que les personnes ne travaillant par l'intermédiaire de plateforme de travail numérique se voit accorder le statut professionnel légale, correspondant à leurs modalités de travail réel. Elle fournit une liste de contrôles pour déterminer si la plateforme est un employeur. Si au moins 2 de ces critères sont remplis, les personnes travaillant par l'intermédiaire de la plateforme devrait jouir des droits du travail et des droits sociaux qui découle du statut de salarié. Après des mois d'intenses négociations. La directive a finalement été approuvé en plénière du Parlement européen, le 2 février dernier. Lequel a supprimé les critères de présomption de salariat ce qui risque d'entraîner une incertitude juridique de conduire à des requalifications massives et au total de causer des pertes d'emplois. L'Europe doit cependant avancer au même rythme sous peine sinon de créer des inégalités de concurrence. Qui affaibliront la compétitivité de nos entreprises. La 2ème objection et qu'elle est réductrice. Les mutations du travail ne concerne pas seulement les plateformes numériques, mais de nombreuses autres branches professionnelles comme l'ont montré les travaux de la délégation aux entreprises sur l'évolution des modes de travail et de management. Rapportée par nos collègues Martine Berthet Michel qui a et Fabien Gay. De juillet 2021, le rapport on appelait donc il y a une réflexion globale sur la définition juridique du travail indépendant qui ne peut se réduire à la seule dimension des plateformes de mise en relation. Il apparaît également que le secteur public s'emparent de cette possibilité en utilisant des algorithmes pour l'orientation des jeunes. C'est le cas de la démarche de Parcoursup et de France emploie. La 3ème objection et que la traduction par la proposition de loi des pistes identifiées dans un rapport d'information le collègue Martine Berthet Pascal je Savoldelli. Sur l'impact des plateformes numériques sur les métiers de l'emploi de septembre 21 les inadapté. Il faut par ailleurs prend regarde ne pas repousser les micro-entrepreneurs. Vers le travail non déclaré avec une réglementation, que l'on souhaite toujours vertueuse mais qui souvent provoque des effets contre-productifs. Pour autant ce taylorisme numérique est un vrai sujet que la proposition de loi soulève a raison. Il crée une surveillance constante des travailleurs par une Intelligence artificielle qui les surveille tout le temps chaque heure chaque minute, chaque seconde. Ce management déshumanisant crée un profond sentiment d'anxiété chez les employés, voire de perte de confiance envers l'employeur pouvant conduire à un désengagement dans le travail. Cependant, ce reflex législatif est-il le bon. Nous avons trop tendance en appeler à la norme pour accompagner l'évolution économique c'est une réflexion conduite en ce moment d'ailleurs par nos collègues. Jean-Pierre Moga Gilbert Luc devina. Il faut simplifier les normes applicables aux entreprises. La solution est sans doute moins normative que managérial. Les employés accepte un peu mieux d'être gérée par une Intelligence artificielle. Si l'employeur prend le temps de leur expliquer le pourquoi et le comment de cette approche managériale. Car cela contribue à diminuer l'insécurité professionnelle ou encore l'asymétrie d'information et le pouvoir. L'employeur doit adapter son Style de gestion afin que l'ajout d'une Intelligence artificielle ne soit pas perçue comme une déshumanisation des ressources humaines mais comme un plus qui vient améliorer la gestion des ressources humaines au bénéfice des travailleurs eux-mêmes. Ah ce vrai sujet une réponse pertinente adaptée et proportionnée s'impose. Ce qui n'est pas le cas de la proposition de loi, laquelle, si elle a le mérite d'attirer notre attention et je me réjouis du débat qui s'ouvre à cette occasion ne peut être adopté je nous donne en revanche rendez-vous lors de la transposition de la prochaine directive européenne en nous gardant bien de contribuer à la surtransposer. Ainsi, vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci Madame, Colette Mélot, vous avez la parole pour le groupe les indépendants. Madame la présidente, madame la ministre. Madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Depuis sa sortie fin 2022 et plus encore depuis celle de sa dernière version. J'ai pété ne cesse de faire parler et nourrit autant d'inquiétude qui ne fait d'adeptes. Parmi les craintes, on évoque les risques liés à la confidentialité des données. Ce relatif à l'exactitude des informations transmises par le Tchad bottes et des risques de plagiats. Il est aussi régulièrement question des risques de suppressions d'emplois que cette Intelligence artificielle générative pourrait causer à ce titre, dans un rapport publié le 26 mars dernier des m'autonomistes que ce type d'Intelligence artificielle pourrait exposer plus de 300 millions d'emplois à l'automatisation. Mais cette inquiétude de l'articulation entre le travail et l'évolution technique et numérique est-elle une nouveauté. Pas vraiment. La crainte des évolutions techniques et de leur impact sur le travail de l'homme existe depuis longtemps et n'a pas en attendu les pontes de la Silicon Valley en 1589. La reine Elizabeth première d'Angleterre interdisez la machine à tricoter les bas de crainte qu'elles ne prive ces sujets d'emploi. Plus récemment, dès l'apparition du verre en France en 2011. Des alertes été lancée sur le risque d'uberisation de la société et la nécessité d'adapter notre droit du travail aux évolutions numériques. C'est donc en permanence que nous devons nous interroger sur le rapport entre les évolutions techniques et le travail c'est ce sur quoi porte la présente, proposition de loi plus exactement celles-ci nous proposent de légiférer sur l'impact des algorithmes dans la relation. cette PPL s'inscrit au-delà du seul cadre des plateformes numériques, l'usage d'algorithmes dans la relation de travail est aujourd'hui présent bien plus largement y compris dans des secteurs qui ne sont pas directement liées au numérique. Processus de recrutement, gestion des carrières ou évaluation des salariés. Les algorithmes interviennent de plus en plus dans la gestion des ressources humaines. Ce texte a le mérite d'ouvrir le débat sur cette nouvelle forme de management qui est le management. Algorithmique et sur les enjeux qu'il soulève. Si ce type d'inquiétude n'est pas nouveau, ce qui inquiète davantage, c'est le nombre important et le type d'emplois qui pourraient être concernées. C'est aussi la rapidité avec laquelle il pourrait l'être. Il nous revient d'encadrer leur usage de sorte qu'il ne se fasse pas au détriment des salariés. Reconnaissons-le pour les travailleurs comme d'ailleurs pour les employeurs, les algorithmes ont souvent quelque chose d'abstrait, voire d'opaques cette PPL pose ainsi des questions tout à fait légitime sur l'articulation entre algorithmes et pouvoir de l'employeur sur les critères et les paramètres retenus par un algorithme ou encore sur les le statut des travailleurs des plateformes numériques. Toutes ces questions sont pertinentes. nous ne pensons pas que les réponses soient dans ce texte, un effet les dispositions législatives, déjà en vigueur n'exclut pas du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. Les décisions prises avec un algorithme. Elle ne les exclut pas non plus du principe de non-discrimination est-il donc nécessaire de légiférer de façon à préciser que tous ceux qui ne serait pas exclu d'une règle qui est inclus. Nous ne le pensons pas. Sur la question du statut des travailleurs des 2 plateformes nous estimons plus pertinent d'attendre la directive européenne qui devrait arriver sous peu. Plus d'un millier de personnalités du monde de la tech signé une lettre ouverte appelant à suspendre le développement de l'Intelligence artificielle et s'interroger. Devrions-nous automatiser tous les emplois devrions-nous développer des esprits non humains qui risquerait de nous dépasser en nombre et en Intelligence. Nous rendent obsolètes et nous remplacer, devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation. Autant de questions auxquelles les 6 mois de suspension demandée par les signataires ne suffiront sans doute pas à apporter des réponses. Les signataires n'a, n'apporte pas non plus mais ils alerte au moins sur ce sujet. À l'image de cette PPL est cependant intéressant d'en débattre et je remercie l'auteur de de la PPL de nous avoir permis d'y réfléchir notre groupe votera contre ce texte. Merci la parole est maintenant Madame Raymonde Poncet Monge pour le groupe écologiste solidarité territoire.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Mark Mac GAN, ancien dirigeant d'Hubert devenus lanceurs d'alerte. Soulignait lors de l'audition du 23 mars dernier dans le cadre de la commission d'enquête relative aux révélations des Hubert face à l'Assemblée nationale. Combien de fois et j'ai eu à faire à des gouvernements qui nous accusait chez Hubert à raison d'être des hors la loi mais en privé, ce même gouvernement nous promettait de trouver des solutions rapides et favorable à la croissance effrénée pardon exigé par nos dirigeants et nos investisseurs en quoi ça sert la démocratie de cacher des rencontres avec des dirigeants d'entreprise. Il poursuit, comment se fait-il que le fer de lance de ceux qui cherchent à vider de leur sens. La directive européenne ne soit autre que la France la même France qui a créé la Sécurité sociale en 45, le SMIC qui ont 50, les congés payés, le minimum vieillesse, le RSA et la retraite à 60 ans. Nous saluons la proposition de loi de nos collègues du groupe CRCE. Qui au-delà des plateformes numériques dite de mise en relation adapte une partie de notre droit à l'avancée de l'organisation algorithmique du travail dans les entreprises. Il nous apparaît effectivement fondamental et urgent. De définir juridiquement l'algorithme comme intégration automatisée du pouvoir de direction d'organisation et de contrôle de l'employeur employeurs seul responsable in fine et des critères et finalité retenu dans le cahier de charges. Auprès des programmateurs informaticien. Le traitement automatisé qui s'en suit ne peut masquer et. Le concepteur derrière le management algorithmique oui selon une formule pertinente de de la proposition de loi. L'algorithme est devenu le contremaître des temps modernes. l'employeur doit pouvoir répondre d'un possible bien de discrimination de l'algorithme et à l'obligation de s'en expliquer et de le corriger et dans le cas dans ce cadre, le comité social et économique devrait avoir connaissance des logiques de fonctionnement des algorithmes pour exercer pleinement ses propres Enfin, concernant le cas spécifique des plateformes numériques lorsqu'elle définit et contrôle les caractéristiques essentielles de la prestation et de la relation de travail là. L'article 3, nous invite à intégrer dans le droit du travail. La jurisprudence de la Cour de cassation en contestant leur qualité de simple mise en relation. Nous appelons dès lors la France. À soutenir enfin au Conseil de l'Union européenne, la directive visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes. Adopté au Parlement européen. Effectivement ce 3 février. Elle établit une présomption légale de salariat. D'autres pays européens ont déjà des vies Car le récit d'indépendance de prétendue indépendance des opérateurs de ces plateformes. Se révèle souvent une fiction déconstruite par la force de rappel d'une exploitation sans régulation. Faites-vous livrer là où la vie vous mène. Propose Hubert via une campagne commerciale des livraisons réalisées au détriment des conditions de travail des coursiers contrôle en temps réel opacité de la fixation des tarifs dépendance à l'algorithme dans les fêtes, le modèle économique des plateformes numériques participent massivement à la précarisation et à la paupérisation des travailleurs. Plus de la moitié des travailleurs de plateforme de l'Union européenne gagnent moins que le salaire horaire Net du pays dans lequel il travaille. Le journal Le Progrès et d'autres. Journaux régionaux publié mardi. Un dossier sur Le Berre réalisation titré les forçats de la livraison. Selon la Commission européenne cette directive permettrait à la France. Outre l'amélioration essentiel des revenus du travailleur de rentrer entre 328 à 780 millions de recettes annuelles supplémentaires. Nous l'avons déjà signé souligné durant l'examen de la réforme des retraites. Voici de vrais alternatives au financement de la protection sociale renoue enfin avec le progrès social, aussi le groupe écologiste solidarité et territoires votera cette proposition de loi qui reprend d'ailleurs plusieurs recommandations de la mission d'information sénatoriale. Je vous remercie. Monsieur Ludovic et vous avez la parole pour le groupe du Rassemblement démocratique progressiste et indépendant. Merci. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi entend encadrer davantage la numérisation des relations de travail en définissant juridiquement l'algorithme en renforçant notamment également les prérogatives d'information et de contrôle des comités sociaux économiques et en légiférant sur le cas particulier des plateformes de mise en relation. En effet, en 2021, nous avons mené une mission d'information dont j'avais été le vice-président. Je salue le travail du président Pascal Savoldelli qui était avec nous sur ce sujet portant notamment sur l'impact des plateformes numériques et sur les métiers Nous avons formulé diverses recommandations autour de 4 grands axes, avec notamment l'amélioration des conditions de travail, le développement du dialogue social, l'encadrement du management algorithmique ainsi que la transparence et la régulation des algorithmes, des plateformes. Ainsi madame la rapporteure si nous soutenons l'objectif de votre texte qui est bien l'amélioration de la protection des salariés. Dans le cadre d'une relation algorithmique du travail nous sommes cependant, nous ne sommes cependant pas totalement en adéquation avec les moyens invoqués en effet concernant l'article 1er, nous ne pensons pas que le dispositif proposé apporte des garanties supplémentaires aux travailleurs car l'employeur est déjà responsable de ses décisions, même lorsqu'il a recours à divers moyens technologiques. Nous serions plutôt favorable à un dispositif qui permettrait d'améliorer l'information des travailleurs sur ces plateformes qui faciliterait leur accès aux données générées par leur activité et qui contribuerait à les supprimer automatiquement à intervalles réguliers de l'historique de leur donner. La garantie de l'intelligibilité des algorithmes pour les travailleurs hé bien la première étape indispensable pour faire du contenu de la gauche un véritable objet de négociations et pour permettre que ces problématiques intègre le dialogue social. Concernant l'article de si nous sommes favorables à une lutte plus accrue contre les discriminations au travail qui peuvent être aggravé par l'utilisation des algorithmes. Nous pensons cependant que le dispositif proposé est déjà satisfait par le droit en vigueur. Il nous faut également rappeler que la procédure relative au contentieux des discriminations au travail peut déjà s'appliquer au recours, comme l'a dit Madame la Ministre ce matin contre les décisions des employeurs prises à l'aide d'outils technologiques au fil des auditions que nous avons menées durant cette mission d'information, nous avons acquis la conviction qu'un algorithme n'était pas seulement une suite d'opération permettant de traiter des volumes importants des chaînes de données mais bel et bien une chaîne de responsabilités humaines le long de laquelle il demeure possible d'intervenir à chaque moment de son utilisation. Cela peut être effectué en rappelant la possibilité pour les salariés par exemple d'utiliser le statut de lanceur d'alerte. Si votre article numéro 3. Soulève le sujet très attendue de la définition et de la qualification des travailleurs des plateformes nous pensons cependant que nos travaux gagnerait à être orientée sur l'amélioration concrète des protections dont bénéficient ces travailleurs. Je ne vous apprends rien. Des négociations sont en cours en ce moment, au moment où je vous parle au Conseil de l'Union européenne au sujet de la directive lié à la présomption légale de salariat. Cela été présenté en décembre 2021 par la Commission européenne cette requalification que nous soutenons permettra un réel, renforcement des droits des travailleurs des plateformes. Le développement des plateformes numériques. Il a considérablement transformé notre rapport au travail, ainsi que notre modèle social et économique. Le travail est bien le secteur qui a subi l'une des évolutions les plus considérables. Notre société ces dernières années, nécessitant une adaptation très forte de la part des travailleurs. La généralisation du télétravail induite par la crise sanitaire et plus récemment les débats animés sur le sujet des retraites ont démontré toute l'importance et les inquiétudes des Français à ce sujet. Ainsi, si nous soutenons certains des constats effectués par cette proposition de loi. Et je tiens ici à saluer tout le travail effectué. Notre groupe RDPI ne votera pas en faveur de ce texte. Toutefois, nous nous positionnons pour engager une réflexion d'ensemble sur le sujet du travail et des valeurs qui l'accompagnent pour aboutir in fine et à l'élaboration des textes législatifs. Je vous remercie. Madame Corinne Féret, vous avez la parole pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame Madame la présidente. Madame la ministre madame la rapporteure. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre de la proposition de loi relative à la maîtrise de l'organisation algorithmique du travail. Le groupe socialiste, écologiste et républicain accueille très positivement ce texte tant qu'il est en phase avec l'actualité chaque jour démontrent que la plateforme. Mise à Sion, pardon du travail n'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie contre notre modèle social avec au coeur de sa matrice l'opacité de la boîte noire que l'algorithme. Nous avons toujours affirmé n'être en rien opposé au développement de l'économie numérique et aux plateformes collaboratives qui rendent de nombreux services à nos concitoyens. Mais nous avons souhaité faire continuellement la distinction entre ces interfaces et les plateformes numériques de travail qui dérégule le marché du travail et de nombreux secteurs d'activité. Formulées aussi des propositions afin de réguler cette plateforme plateforme isolation de l'économie, c'est ainsi que notre collègue Monique Lubin porter dès 2019 une proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numérique. En France, plusieurs milliers de femmes et d'hommes ont été séduits par les promesses de plateformes qui proposent une organisation du temps du travail sans contrainte hiérarchique. En pratique à cette illusion de liberté se substituent fréquemment une réalité bien plus brutal. Les travailleurs se retrouvant très rapidement, pieds et poings liés face aux exigences des plateformes du jour au lendemain. Certains d'entre eux voire voir le voient leur compte suspendu souvent sans aucune justification. Ce d'autant plus dur, qui sont privés de nombreux droits sociaux du fait du statut fictif de travailleurs indépendant. Nul ne peut plus nier que la dématérialisation des entreprises à laquelle nous assistons avec l'Intelligence artificielle et plus largement le numérique bouleverse toutes les relations de travail de plus en plus de travailleurs seront géré par un algorithme qui attribuera des tâches les rémunérera organisera leur travail les évaluera et même les sanctionnera, l'enjeu se trouve désormais dans la maîtrise de ses algorithmes. Il est de notre responsabilité de garder la main mise sur les innovations technologiques avant de nous faire dépasser par celle-ci encadrée et contrôlée telle devraient être nos maîtres mots si le rôle de simple intermédiaire de mise en relation est souvent avancé par les plateformes elles-mêmes pour décrire le fonctionnement des algorithmes. Personne ne peut plus le que le management algorithmique contribue au contraire à déterminer des conditions de travail et de rémunération des travailleurs bien au-delà d'une simple mise en relation entre offre et demande. Les algorithmes de tarification les mécanismes d'incitation et les systèmes de notation ont des effets Directs sur le comportement des travailleurs des plateformes modifiant leur organisation à leur temps de travail ne leur permettant pas d'avoir de la visibilité sur le revenu, ni sur leur projet professionnel. Un algorithme n'est pas seulement une suite d'opération permettant de traiter des volumes importants de données mais bien une chaîne de responsabilités humaines le long de laquelle il demeure possible d'intervenir à chaque étape de sa conception et de son utilisation. faisons, nous sommes bien évidemment favorables à la proposition de loi du groupe CRCE qui reprend d'ailleurs plusieurs propositions du rapport de la mission d'information du Sénat sur l'uberisation de la société que nous avions approuvé en plus de participer activement à cette mission. Notre groupe avait rédigé une contribution notamment pour insister sur la légitime question du statut des travailleurs des plateformes. Oui nous devons inscrire dans la loi que les décisions des des employeurs prises à l'aide de moyens technologiques sont des décisions relevant de leur pouvoir de direction. Oui, il importe en cas de litige portant sur une discrimination au travail, que ce soit à l'employeur d'apporter la preuve que les outils qu'il utilise ne sont pas source de discrimination. Notre collègue Olivier Jacquin dans sa PPL visant à contrôler la place de l'algorithme dans les relations contractuelles avait d'ailleurs déjà émis ce souhait hé oui enfin, il convient de conforter le mouvement jurisprudentielle actuelle en faveur de la requalification de certains travailleurs des plateformes. Ceci en soulignant bien la distinction réelle entre d'une part le véritable opérateur de mise en relation, et d'autre part les plateformes d'emploi qui exercent un contrôle juridique et économique sur les éléments essentiels de la relation qu'il nie qui les lie avec les travailleurs. Il est grand temps d'avancer sur ces sujets, l'Intelligence artificielle est utilisée dans des outils qui vise à éclaircir la prise de décision ou pour surveiller les employés. Cela crée une asymétrie de pouvoir et d'information. L'algorithme déformant l'ensemble des conditions de travail. Nous avons le devoir aujourd'hui d'agir pour y remédier. Je vous remercie.

Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Pascal Savoldelli pour la présentation de la proposition de loi visant à mettre en oeuvre une maîtrise de l'organisation algorithmique du travail. Celle-ci s'inscrit. Dans la continuité de son Tour de France et de son travail pour la création d'un véritable statut des travailleuses et très travailleurs des plateformes numériques. Je remercie également ma collègue Katia pour polie pour la présentation de son rapport et pour les auditions que la conduite et qui ont permis d'enrichir le travail de Pascal. Cette réflexion sur le travail dans notre société est essentiel. Plutôt que de voter pour la retraite à 64 ans et de voler les 2 plus belles années de vie à la retraite des travailleurs et des travailleuses. Le gouvernement et la droite sénatoriale aurait été plus inspiré d'avoir un débat sur le partage des richesses et le sens du travail. Nous ne pouvons plus en faire l'économie. Le travail connaît des mutations avec la généralisation de l'information et la robotisation amorcé dans les années 1980 et maintenant avec une étape supplémentaire. L'Intelligence artificielle et les algorithmes. Ces algorithmes qui dicte les contenus dans nos téléphones nos articles de presse. Nos pensées et nos vies en nous orientant seulement vers ce que nous aimons. Ils nous privent de découverte et donc de l'inconnu mais il modifie aussi notre rapport au travail et notre vie en société. Nous leur sommes donc subordonnée en tant qu'être humain citoyennes et citoyens et travailleurs et travailleuses. Il est urgent d'encadrer l'Intelligence artificielle et les algorithmes même et l'autre qui est fondamentalement opposé aux droits sociaux et syndicaux à réclamer avec une certaine, une centaine d'experts mondiaux. Une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles, c'est bien un comble car elle pose un problème de protection des données de dérégulation du marché de l'emploi et de circulation de fausses informations. Sous couvert de neutralité d'équité ses algorithmes sont en réalité des aides à la décision de l'employeur. Demeure le seul donneur d'ordres et donc ils sont subjectifs. Il s'agit d'un nouvel outil de contrôle des travailleurs et travailleuses de management mais aussi de discrimination et même parfois de répression syndicale, ce n'est plus le patron qui vous licencie, c'est l'algorithme qui vous suspens. C'est pourquoi nous proposons de modifier le code du travail pour que les décisions prises à l'aide de moyens technologiques relève du pouvoir de direction de l'employeur qui lui programme la machine à son Avantage. Car la relation de travail est certes moins directe avec l'employé mais elle reste. Contractuel et accroît la domination, l'employeur en faisant peser de nouvelles contraintes sur les salariés en étant maître de sa programmation et en organisant l'opacité. Il reste le décideur unique et le donc il y a bien un lien de subordination ces algorithmes incite à davantage de rendement en autant les travailleurs et travailleuses et les pousse à toujours plus de productivité. Il est d'ailleurs urgent de leur garantir un droit à la déconnexion car le contremaître numérique lui ne prend jamais de pause et surtout l'algorithme est froid avec lui plus de débats plus d'associations du salarié aux prises de décision ou même de discussion sur le sens du travail. L'Intelligence artificielle et l'algorithme c'est travaille et tais-toi. Ne pas légiférer, c'est refuser d'équilibrer la relation entre les employeurs et les travailleurs. C'est donc laisser ses salariés en dehors du Champ du code du travail et refusé de les protéger face à un système qui s'étendra peut-être demain à tous les champs du salariat. Car qui dit algorithmes dit souvent salariés déguisés reconverti en auto entrepreneur sans droit ni salaire mais avec une rémunération à la tâche et la contrainte de faire 60 heures par semaine pour s'en sortir. La commission des affaires sociales du Sénat a estimé qu'il était prématuré de légiférer avant l'aboutissement des travaux européens. Pourtant le sénat français devrait faire avancer la législation nos propositions de loi porte cette ambition. Elle prend acte de la résolution adoptée par la Confédération européenne des syndicats, du 6 décembre dernier, celle-ci a établi la nécessité pour les syndicats, les représentants des travailleurs de bénéficier d'une expertise externe pour évaluer l'impact des algorithmes, sur les conditions de travail. Oui, il faut de la transparence et de l'expertise pour rééquilibrer la relation au travail des plateformes numériques et nous proposons de lever la zone d'ombres concernant le véritable statut des travailleurs et travailleuses dès lors que les plateformes encadre juridiquement et économiquement l'activité des travailleurs, ils ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs indépendants, ils doivent être reconnus comme ce qu'ils sont à savoir des salariés dans un rapport de subordination avec les plateformes face aux entreprises qui ne respectent ni leurs obligations fiscales. Ni leur obligation administrative, la loi doit imposer le respect de leur obligations sociales et donc nous voterons cette proposition de loi.

Monsieur le président. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure, chers collègues, je veux à mon tour remercier notre collègue Pascal Savoldelli, et le groupe communiste de nous permettre une nouvelle fois de débattre de l'impact du numérique sur le travail des nouvelles formes de travail de la plateforme nisation. Et de ce qu'on appelle plus communément l'uberisation. Chers collègues, c'est le 4ème texte sur lequel sur le sujet que nous étudions depuis 4 ans, après déjà 2 missions d'information et je ne compte pas le nombre de textes déposés. Pour continuer d'alimenter nos réflexions. À croire que l'on parle davantage du travail, grâce aux initiatives parlementaires que dans les projets de loi du gouvernement. La question au fond central qui est devant nous et simple. Comment s'assurer que le progrès technologiques permettent l'émancipation des travailleurs et non leur assouvissement via un contremaître 2.0. Corinne Féret a eu l'extrême gentillesse de citer ma proposition de loi de 2021. Refuser ici dans laquelle nous étions déjà en avant la nécessité de contrôle et de transparence des algorithmes. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui continue d'avancer dans la bonne direction et je m'étonne que la majorité sénatoriale continuent de se cacher sur ce sujet majeur après le revirement opéré l'année dernière lors des débats sur les ordonnances dites Mettling. En 2019, la commission des affaires sociales a affirmé dans un rapport être opposé au tiers statut mais en 2021, vous avez donné un blanc-seing au gouvernement dont l'intention tout comme celle de la rapporteur de l'Assemblée nationale était limpide, je cite, réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination de telle sorte que le risque de vol qualification soit aussi réduit que possible. Je ne fais que vous citez Madame la Ministre puisque vous étiez la rapporteur sur ce texte vous oubliez pourtant que nombre de ces travailleurs sont des indépendants fictif, comme les a qualifiés. La Cour de cassation. Grâce à l'excellent rapport de Katy ah pour politi j'apprends que notre collègue Frédérique Puissat évoqué en commission une position plus nuancée, porté par la majorité sénatoriale, sans pour autant nous en dire dans davantage et sans poser d'amendements à ce texte j'ai peine à comprendre. Et si je peux rejoindre notre collègue Pascale Gruny sur le fait qu'il faille s'assurer que les textes que nous votons soit en conformité avec la directive de Nicolas Schmit en cours de discussion au niveau aurait pas et que vous n'avez même pas citer Madame la Ministre je ne peux dès lors que vous appelez toutes et tous à voter la proposition de résolution européenne que j'ai déposé hier avec mes collègues Monique Lubin et Laurence Harribey nous y'appelons le gouvernement à soutenir ces directives qui garantit de véritables droits aux travailleurs des plateformes. Je rappelle que cette directive reprend beaucoup des propositions que le groupe socialiste défend ici depuis des années et dont notamment dans ma PPL de 2021 la présomption de salariat l'inversion de la charge de la preuve en matière de requalification et la transparence des algorithmes Ces directives reprend par ailleurs une idée que je mets au débat depuis plusieurs années une adaptation du devoir de vigilance des multinationales à l'uberisation pour garantir aux travailleurs un ultime filet de sécurité. En effet, l'article 8 de la directive institut qu'ils pourront exiger des explications sur les décisions. Algorithmiques les impactant avec obligation pour la plateforme de répondre par écrit, sous une semaine, un article qui est donc en parfaite concordance avec la présente, proposition de loi. Mais surtout, chers collègues, en votant ce texte nous disons au gouvernement qu'il fait fausse route, qu'il doit arrêter de bloquer une directive proposant un cadre de régulation des algorithmes pour la protection des travailleurs des plateformes et espérer son adoption sous la présidence espagnole de l'Union européenne dès lors avec mon groupe nous vous appelons malgré les réserves qui ont pu être émises par les uns ou les autres à voter ce texte. Je vous remercie. Merci je l'addition générale est Close, la commission n'ayant pas élaboré texte nous passons à l'addition des articles de la proposition initiale. Je mets donc aux voix l'article 1er qui est pour.

Donc je vais essayer de vous convaincre de tous voté l'article hein et, et notamment en reprenant ce qu'a dit Madame la Ministre parce que Madame Lamy, J'en profite mais franchement tout à l'heure je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, vous avez dit que tous les dispositifs étaient bon. En termes de dialogue social et de lutte contre le salariat déguisé et cet article défini là l'algorithme au plan juridique comme pouvoir direction et de contrôle. Mais je vais vous dire, madame la Ministre, franchement. Allez voir les livreurs. Allez voir les femmes qui font le ménage à les voir, je vais vous en citer moi des professions qui sont détournés plaide pas forme numérique de travail vous savez ce qu'ils disent.

Mais franchement, aller voir les prud'hommes, aller voir les juges aux prud'hommes ce qui disent la difficulté qu'ils ont parce que maintenant il y a de plus en plus de contentieux. Et vous verrez, madame la Ministre, que les leviers de négociation. Soyez à la place de ces hommes et ces femmes. Comment vous défendez vos intérêts particuliers et la négociation collective, quand en face vous avez un outil totalement dématérialisée et des musées déshumanisé. Donc voilà si on veut être levier béquille je pense ça serait bien de voter déjà au moins l'article 1 maire merci à mes collègues de l'air de faire un petit geste. Puisque vous m'y invitez, je vais donc le mettre aux voix cet article 1. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté.

La parabole historique de la relation entre la technologie et le travail qui me, qui me semble tout à fait intéressante chers collègue, vous auriez pu aussi es beaucoup plus loin, Pline l'Ancien. Qui rapporte que l'empereur Tiber avait mis à mort un ouvrier verrier qui lui proposer le verre incassable parce que ça mettait en danger toute la profession des des verriers. Il y a aussi la révolte des canuts en 1819 contres les machines à à ton de l'aidera mais en l'occurrence il ne s'agit pas du tout de cela. Jusqu'à présent il y avait une relation sociale du travail entre des employeurs et des salariés, là il y a une nouvelle chose qui arrive qu'est la plateforme considéré comme un monstre noir neutre complètement technique qui fonctionne avec des algorithmes et qui donne l'illusion que son travail ne serait que de mettre en relation des clients et des auto-entrepreneurs, ce qu'il faut bien comprendre, chers collègues, c'est que dans cette. Technique algorithmique ce qui a c'est. La Noga sur la négation totale de la relation sociale du travail et in fine et la négation de ce qu'est l'entreprise avec des plateformes. Vous en avez plus d'entreprise et vous n'avez plus aussi d'entrepreneurs. Donc je pense que ce qui est ce qui est en jeu et tout à fait fondamental parce que ça touche à beaucoup de points qui concernent notre société. Je pense aussi à la difficulté que nous avons pour légiférer contre les Gafam et contre leur incapacité à pouvoir réglementer les propos haineux en ligne. Il s'agit du même problème on nous laisse à croire que les plateformes seraient des outils techniques complètement neutre. Ce que nous voulons nous, c'est remettre du social. Derrière ça, nous sommes tout à fait contre l'irresponsabilité sociale organisée par les algorithmes. Merci madame la présidente. Merci je vais donc mettre aux voix, l'article 2 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est également adopté. Je vais maintenant mettre aux voix, l'article 3. Qui est pour. Qui est compteront qui s'abstient. Il est également adopté. Et mes chers collègues, sur l'ensemble du texte. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Il y a une demande de scrutin public par le groupe les républicains. Mais monsieur ça Denis. Je vous donne la parole avant le Merci madame la présidente Madame la Ministre mes, mes chers collègues. Pourrait réagir mes propos parce que. Je vais. Essayer d'interpréter la demande de scrutin public. Parce Parce que pourquoi il y a scrutin public. Parce qu'que aura à travers la question de l'algorithme. Il y a des questions. Qui ont été évoqués d'ailleurs par plusieurs de mes collègues. De tous les bancs. C'est que derrière. Il y a la question du temps de travail. Hé oui il y a la question de comment définir un salaire comment défini la valeur ajoutée. Il y a ces questions-là qui sont derrière. Et et ces questions là sont. Je m'excuse, mais je vous le dis et d'ailleurs elles sont pas que de gauche. Il y a plein de gens en ce moment qui se mobilisent par rapport aux retraites parce qu'ils sont préoccupés aussi par leur niveau de retraite mais aussi leur niveau salarial leurs conditions de travail, le sens de leur travail et Donc là je je je dis ça parce que. Des fois on nous dit, notamment au gouvernement qui aurait, il y aura. Une confusion un brouillard sur le clivage gauche droite. On voit bien qu'à la fin sur cette question là, il y a réellement un clivage gauche droite, mais la droite n'est pas quelque chose d'uniforme et monolithique. Il y a des droites en France et comme il y a des gauches, sauf que là, les gauches sont rassemblées unis et là les droites non pas tout à fait la même approche du sujet merci. Y a-t-il d'autres explications de vote. Donc nous allons procéder au scrutin. Et le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin est donc clos. Alors votants 319 exprimés, 262 pour 104. Contre 158. De ce que le Sénat n'a pas adopté.

on se pose un certain nombre de questions que vous avez l'air très bien évoqué au moment de vos données intervention sur les enjeux de la condition de travail sur les enjeux du temps de travail. Également sur la responsabilité des des employeurs dans cette situation-là et notamment ça t'appelle. Beaucoup d'élus locaux. Il y a les parlementaires, mais aussi les locaux, des élus locaux qui vivent au quotidien cette situation-là donc, merci d'avoir apporté ces débats dans les différents groupes. Merci d'avoir porté le débat la Commission sociale cet après-midi c'était plus une litanie de d'intervention, mais à la commission sociale, nous avons vraiment évoqué le sujet et je voudrais remercier le le travail et la rapporteur qui a su au-delà de reprendre un certain nombre d'arguments qui avait su en tout cas levé le débat en commission Affaires sociales en pose un certain nombre de questions pour faire réagir, notamment ceux qui travaillent sur les conditions du de du et des conditions au-delà de tout ça, je pense que c'est un sujet qui sera de nouveau d'actualité dans cet hémicycle parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, on va-t-en beaucoup de la directive européenne mais je crois que ça ne fait pas tout et donc en tous les cas je voulais en tous les vous donne donné rendez-vous parce que nous aurons certainement avec le gouvernement l'occasion de revenir sur le sujet. Très bien je vous remercie. Je vais donc suspendre la séance. Je. Madame pardon. je voudrais effectivement à mon tour vous remercier pour la qualité des débats. Je sais qu'effectivement, beaucoup d'entre vous sont pleinement impliquée depuis. De longues années maintenant avec cette, cette volonté de travailler autour des conditions de travail plus largement pour l'ensemble des travailleurs. En France, mais, mais évidemment de s'adapter aux évolutions sociétales et de ce que vient de ce que viennent. Percuter finalement ces nouvelles formes de travail ces nouvelles modalités également. De pilotage des activités si je puis dire. C'était évident que cette question elle a toute sa place dans le débat public. Elle a d'ailleurs je tiens à le redire eu toute sa place dans le cadre des Assises du travail. Je vous propose que nous puissions travailler sur le compte rendu aussi des Assises du travail et puis avancer au au regard. Des évolutions. Des textes européens mais également des concertations nationales autour de ces enjeux pour que nous puissions évidemment nous assurer que notre socle

Texte législatif qui arrive aux différents niveaux et des différentes évolutions qu'on pourra porter ensemble. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autre demande d'intervention dans ce cas je vais lever la séance pour 10 minutes. Elle sera reprise à 16h, la séance et. Suspendu.

La séance est reprise et l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement. Dans la discussion générale. La parole est d'abord à monsieur Roland Lescure Ministre délégué chargé de l'industrie.

madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices. Notre vision est claire pour EDF. L'énergéticien national est au coeur de la transition énergétique du pays. C'est aussi la vision qui régnait il y a près de 77 ans, quand Marcel Paul, un ministre communiste. A présidé à la création d'EDF. Avec comme objectif un monopole de l'énergéticien qui a conduit 77 ans plus tard. Ah d'électrification du pays. La construction du 2ème parc nucléaire au monde. Nous envoyons nous en bénéficions encore des fruits aujourd'hui avec un mix électrique parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre au monde et parmi les plus compétitifs. Depuis 20 ans évidemment notre énergéticiens nationale a été affecté pour du bon et du moins bon par l'ouverture sur l'Union européenne avec la loi de février 2000 sur la modernisation du service public de l'électricité. Et le sommet de Barcelone en mars 2002 qui a conduit à la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Certes ce marché intégré à des défauts et nous y travaillons. Reconnaissons quand même tous ensemble que ce marché est aujourd'hui le plus gros systèmes intégrés en électricité du monde qui fait. Quasiment tous les jours que compte la France a besoin d'électricité, elle peut en apporter de ses voisins et inversement, quand elle en a trop, elle peut elle-même en exporter ailleurs ayant vécu une dizaine d'années au Québec qui depuis 2 jours à un million de Québécois privés d'électricité. Je sais de quoi je parle et je vois combien cette capacité de l'Europe à avoir au marché de l'électricité intégré nous a été favorable. Notre vision pour EDF et clair. Le groupe Électricité de France est et restera un instrument essentiel pour mettre en oeuvre la politique énergétique de l'État français et au Un champion à l'exportation. Aujourd'hui et ça a été extrêmement bien spécifié dans la lettre de mission du nouveau PDG Luc Rémont dont vous avez collectivement voté la nomination à ce à ce titre le sujet d'EDF. C'est essentiellement la production les capacités opérationnelles et la conduite des grands projets industriels. de millions de de des dizaines de milliards d'euros pardon, tous les ans pour lesquels il faut des moyens et la crédibilité financière. EDF a besoin de retrouver sa maîtrise industrielle dans le nucléaire, EDF a besoin de monter sur les énergies renouvelables, avec des objectifs ambitieux pour les 30 prochaines années. Pour cela, le gouvernement a pris ses responsabilités, l'État a toujours accompagné EDF dans ces opérations de recapitalisation ce soit en 2017 en 2022. On n'a jamais autant investi dans le nucléaire que depuis 2017 on va évidemment accéléré tout ça mais il faut quand même le reconnaître. Nous avons sécurisé le calendrier de l'EPR de avec le projet de loi nucléaire que vous avez voté en première lecture. EDF aujourd'hui est néanmoins une société endettée, une société avec de gros besoins d'investissement. C'est donc conformément aux engagements pris par le président de la République durant sa campagne que nous avons lancé dès cet été, une offre publique d'achat pour prendre le contrôle à 100% du capital d'EDF. Vous avez libéré 9,7 milliards de crédits budgétaires avec cette nationalisation nous renforçons les moyens d'EDF pour investir dans les prochaines années et nous crédibilisent son sérieux financier. Vous le savez, l'offre publique d'achat est en cours de finalisation d'ici début juin après épuisement des derniers recours. Ce gouvernement répond donc aux vraies problématiques du groupe EDF et nous avons été il faut le reconnaître, un peu surpris quand cette proposition de loi visant à nationaliser EDF est tombé dans un calendrier un peu surprenant et il faut le reconnaître dans de l'examen à l'Assemblée nationale flirtant parfois avec des théories du complot. Cette PPL vise à répondre à des angoisses qui n'ont aucun lieu d'être. Bruno Lemaire a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je l'ai dit moi-même devant la tribune de l'Assemblée nationale et je vous le répète le projet Hercule est mort et enterré, il n'y a aucun projet ni visible ni caché de démantèlement de notre opérateur national. Je salue le travail sénatorial qui durant l'examen en commission a fait preuve de sagesse en réécrivant une bonne part du texte issu de l'Assemblée nationale. Je salue particulièrement le travail et l'esprit de responsabilité du rapporteur pour cette remise à plat. En particulier le texte de la commission supprime les articles 1 et 3 de nationalisation du groupe EDF qui pouvait fragiliser l'OPA en cours de finalisation, tout en arrivant, reconnaissons-le, à contretemps. Retire de l'article de les références aux activités d'un groupe unifié dans le capital aurait été totalement accessibles qui rendait du coup absolument impossible. Les opérations courantes de gestion d'actifs par EDF, dont les 3 milliards de cession d'actifs dans lequel l'électricité, l'électricien pardon national est d'ores et déjà engagés. Ce texte issu de la commission, modifier également l'article 3 bis pour restreindre le périmètre d'extension des tarifs réglementés de vente au chant des TPE qui ne sont pas encore éligibles. Sur cette base, nous avons donc matière à avoir une discussion je dirais apaisée et constructive. Il nous reste malgré tout de points. De désaccord sur lesquels je souhaite attirer votre attention, on y reviendra évidemment dans le cadre de la discussion des amendements. D'une part sur l'article de. Cet article inscrit dans la loi que les tiens détient 100% du capital d'EDF. Pas de problème avec ça, nous partageons cette proposition qui redonne une place importante au Parlement, qui aurait ainsi à se prononcer sur n'importe quel réouverture du capital. Il n'y a aucune ambiguïté sur nos intentions, je le répète, le projet Hercule a été abandonnée, mais cela va sans dire, ça va peut-être mieux en l'écrivant. En revanche, telle qu'il était formulé aujourd'hui cet article prescrit l'ouverture d'au moins 1,5% du capital d'EDF aux salariés et anciens salariés du groupe et ce d'ici le 1er janvier 2024. Je l'ai dit l'OPA n'est pas encore terminé, il nous reste notamment à convaincre suite au recours encore déposé à peu près 5% des actionnaires à apporter leurs titres dont un samedi, un certain nombre d'actionnaires salariés. Il nous semblerait pour le moins prématuré d'envisager de l'intéressement les participations via de l'actionnariat salarié pour quelques mois alors que nous reviendrions d'acheter les 10 actions de la part des salariés en question. La situation financière d'EDF. Il faut être clair, ne le permet pas aujourd'hui. Nous proposons dans le cadre de la discussion. Un amendement de compromis qui vise à laisser ouverte la possibilité d'actionnariat salarié pour l'avenir, tout en évitant de la forcer en la rendant automatique et ce dès le 1er janvier prochain. 2ème point de discussion et j'en terminerai là vous avez proposé l'extension du tarif 10 réglementés du TRV à toutes les TPE alors qu'aujourd'hui il est réservée aux TPE petite consommatrice. C'est peut-être bien mais ça coûte cher Monsieur le. Président gay. D'abord. Il faut reconnaître que ça remet en profondeur. En question, la logique même du TRV qui dans le cadre des discussions avec la Commission européenne qui ont permis de l'adopter, visait avant tout à protéger les consommateurs. J'allais dire comme vous et moi et les petites entreprises qui avaient elles-mêmes une consommation similaire aux ménages à être protégées par ce tarif réglementé. Le discussion avec la Commission vise à ce que toutes les entreprises qui ont une consommation je dirais plus proche d'une consommation industrielle soit-elle au au tarif de marché la rédaction vous avez proposé est mieux rédigé limite le Champ aux TPE pour autant à le mettre en place une discussion complexe il prendrait beaucoup de temps avec la Commission de régulation de l'électricité avec la Commission européenne qui prendra sans doute bien bien plus longtemps que nécessaire. Alors qu'aujourd'hui notre objectif 1er il est de protéger les TPE, les PME les ETI et les grandes entreprises contre la crise énergétique. Ça ne fais pas plus long puisqu'on aura l'occasion discuter tout ça dans le cas de la discussion. Pour conclure vous rappeler juste que nous sommes évidemment en phase avec les objectifs réaffirmés par cette PPL réécrite par nos soins. Avoir un opérateur national de qualité inscrit dans la durée qui pourra investir tout ce qu'il faudra pour que les 77 ans qui s'ouvrent soit aussi rempli de succès que les 77 ans qui viennent de s'écouler. Merci à tous et à toutes. Merci Nat parole est maintenant rapporteur Gérard longuet, rapporteur de la commission des finances. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous examinons dans l'enthousiasme général une PPE qui a été voté à l'unanimité ou presque à l'Assemblée nationale 7 TPE présentée par l'excellent député de l'Eure, Philippe Brun, ancien député. Ancienne circonscription de Pierre Mendès France. A été voté à la quasi-unanimité ce qui cache un profond malentendu dans les intentions des différents. Députés qui se sont exprimées à cette occasion. Trois points dans ce texte de loi qui nous vient de l'Assemblée et pour lequel la commission des finances au nom de laquelle je rapporte a tenu à apporter des modifications substantielles le 1er concerne Mayotte qui apparaît mystérieusement on demande un rapport sur l'électricité de Mayotte qui appartient pour partie au département pour partie à EDF Swat, ce n'est pas l'habitude de notre assemblée, d'accepter des rapports mais il aurait été impossible de trancher sur le fond dans les délais d'étude qui était donné à notre commission des finances, le 2ème point beaucoup plus important et qui explique en grande partie du groupe politique auquel j'appartiens, ici au Sénat et qui a été le vote des l'air de l'Assemblée. C'est en effet le soutien apporté aux entreprises. La commission des finances a estimé que nous pouvions faire sauter le verrou. Du transformateur de 36 VA kilovoltampères pourquoi, parce qu'il divisait inutilement. La condition des artisans qui pour les uns, bénéficierait du bouclier fiscal pour la raison qu'ils seraient en dessous et pour les autres, exerçant à peu près même métier étant dans les normes de le de la définition des TPE par l'Union européenne ne pourraient pas en bénéficier. Donc dès lors qu'on a moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires et quelle que soit la la De transformateurs nous pourrons ils pourront bénéficier du. Bouclier tarifaire TRV. Aller plus loin. On reviendra dans le débat des amendements aurait été impossible et dangereux juridiquement. tant vis-à-vis des sociétés qui délivrent de l'électricité. Vis-à-vis de l'Union européenne. Alors le 3ème point est beaucoup plus important, il est passionnant même c'est la crainte exprimée avec force par l'auteur de la PPL sur le risque de démembrement. D'EDF. Et là je crois il faut remercier monsieur Brun parce que avec sa PPL il nous oblige à réfléchir, Monsieur le Ministre, chers collègues. Sur le marché de l'électricité telles qu'il vient d'être secouée depuis un peu plus d'un an est telle qu'il peut évoluer dans l'avenir et c'est ce marché de l'électricité européen. Qui doit donner aux dirigeants d'EDF. Je dirais des indications sur les libertés dont ils doivent jouir pour diriger leur entreprise. plus grand respect pour Marcel Paul et pour des raisons personnelles. En plus, mais nous ne sommes plus en 1946 le marché de l'énergie électrique est libre pour la production, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2002 et il est libre pour la vente. Au consommateur. Qu'il soit d'ailleurs, petits ou grands que l'on produise ou non de l'électricité et personne en Europe ne songe à remettre en cause cette liberté. Cette liberté et ce marché ont-ils été catastrophique. La réponse est non. En réalité, entre 2015 et 2020, le prix moyen du spot c'est situé entre 35 euros le mégawatt et 40 euros le mégawatt. Au point d'ailleurs, c'est une anecdote que la reine à 43 a été moins sollicités ou pas sollicité du tout pendant cette période. Je reviendrai sur la reine. Nous avons donc un marché qui est libre. Mais il y a de vraies questions qui ne sont pas tranchées et qui relève Monsieur le Ministre. Des négociations intergouvernementales et ensuite du Parlement européen. D'une part confirmé la liberté à laquelle sont attachés. L'immense majorité des Européens sur la production et la distribution et la vente d'électricité, je dis bien la vente d'électricité. Et puis se poser la question, quelles sont les priorités de ce marché électrique. Faut-il décarboner la société ou faut-il la verdir pas Il s'agit simplement de la verdir le malheureux nucléaire se retrouvent confrontés aux mêmes difficultés de financement qui l'handicape aujourd'hui. Nous avons un 2ème sujet majeur. À l'aune de l'expérience ah du conflit. Pas du conflit l'invasion. De la l'Ukraine par la Russie. Quel est le le souci d'indépendance acceptons-nous de placer l'indépendance énergétique au rang qui doit être le sien, c'est-à-dire une principale préoccupation, celle qui avait d'ailleurs inspiré. Georges Pompidou et Pierre Messmer lorsqu'ils ont présenté en mars. 1974. Un mois avant la disparition. Du président Pompidou le programme énergique. Elle le programme nucléaire français sur lequel nous vivons encore dans la lancée. Donc question verdir ou décarboné question indépendance ou prix. Occasionnel le meilleur marché, ce qui a été longtemps le gaz russe. Il faut le reconnaître, mais c'est aujourd'hui frappée d'incertitude. J'ajoute. Peut-on imaginer un une organisation du marché qui dépendent moins du spot. Et donc du coût marginal de la dernière entreprise de production électrique thermique. En général allemande marchand la limite, est-ce qu'on ne peut pas avoir des systèmes différents, car le marché de l'électricité bute sur un problème que connaissent bien nos amis électricien. C'est que l'électricité ne se stocke pas. Et donc la régulation est à peu près impossible et les écarts de prix sont spectaculaires. Ce qui aboutit, quand on a un signe, un, un marché qui fonctionne essentiellement sur le coût marginal à des écarts de prix qui sont à peu près insupportable pour le consommateur. J'ajoute que nous sommes français, fier de notre réalisation nucléaire on aimerait en profiter un petit peu et de ne pas être entraîné à la hausse par des cette opération du coût marginal ces questions sur le marché sont absolument préalables. Elle pèse déjà sur le statut et c'est là où je m'adresse non pas je m'adresse à vous mais au delà du Sénat à l'auteur de la PPL le démembrement. D'EDF. Il existe en partie. Le transport et la distribution. Pourquoi parce que nous avons l'obligation au nom de cette liberté d'accepter l'accès des tiers au réseau et comme il y a des monopoles techniques, je ne parle pas de monopole économique je parle vrai de de monopole technique. Il est impensable de multiplier les réseaux tant de transport que de distribution. Il faut donc bien accepter que RTE et Enedis quoi que propriété. De la puissance publique ou de. D'EDF pour RTE. Puisse. d'un défaut d'un des des utilisateurs des réseaux, mais qui n'est que aujourd'hui, l'un des utilisateurs du réseau ce cette première différence vaut aussi pour la question que j'évoquais à l'instant qui est la question de la reine.

Orteils c'est-à-dire ou bien vous prenez ou bien vous payer une certaine somme. Ce qui est le cas des assurances après tout l'assurance paraît cher qu'avant l'accident, on la paye tout le temps même quand on n'a pas d'accident et quand un accident on est content d'être assurée. La reine a joué ce rôle d'assurance sauf que c'est une assurance qu'on paye après l'accident, ce qui est évidemment beaucoup plus facile, c'est comme gagner sur les courses de chevaux. Après l'arrivée hé bien ce système là de la reine est au coeur de des préoccupations. De même, nous avons des fournisseurs extrêmement sérieux, y compris français d'électricité qui accepterait volontiers de participer au financement du nucléaire français non pas pour l'exploiter Dieu les en garde enfin Dieu ou la l'ASN où l'IRSN. Je ne sais pas mais en tous les cas il. Il ne souhaite pas exploité, il souhaite simplement. Pour avoir des droits de tirage avec une certaine stabilité. On pourrait même imaginer nous législateurs après tout ça relève de de notre rôle de conduire les. Les entreprises qui revendique de fournir de l'électricité de de garantir 70% de l'approvisionnement par des contrats à long terme que la commission jusqu'à présent on refuse et donc je lui ai dit vous avez un formidable combat mais c'est quand on verra les éléments de ce combat les points à gagner les points au contrôler et puis les les malheureusement les embuscades dans telle ou telle règlements que nous pourrons nous retourner vers les dirigeants d'EDF en leur disant attention, là vous avez une opportunité qu'il faut saisir ou au contraire vous avez un risque qu'il faut assumer et c'est la raison pour laquelle je me retourne vers vous d'abord mais vers Philippe Brun également en l'exigeant votre PPL on connaîtra. Quand on ne connaîtra les règles du jeu définitif. Aujourd'hui elle est prématurée et donc je propose une mesure conservatoire, 100% du capital l'État à la main. Le Parlement est en pleine responsabilité et laissant à chacun à faire son métier. Ayons confiance en nos électriciens et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté et s'est terminé de faire d'EDF une une fierté nationale. C'est dans le texte. le texte. Vous savez que nous sommes dans des niches que le temps est contraint donc je demanderai à chacun des orateurs. Par respect pour. Les porteurs de ces propositions. Loi de respecter leur temps de parole de façon à ce que l'on puisse finir les 2 PPL merci. Monsieur bien que vous avez la parole.

Alors que le doute plane sur l'avenir du groupe EDF et malgré l'abandon du projet Hercule. Les députés ont voté la proposition de loi visant à la nationalisation du groupe EDF. Mais au Sénat. Il a été rebaptisé protéger le groupe L actrice France donne démembrement. Spectre d'exclus le ne fait pas totalement. Et nourrit des inquiétudes. Il visait à réorganiser. Ça pour subvenir aux investissements nécessaires, d'une part. Pour prolonger la de rénover du parc nucléaire d'autre part développer le jeu énergies renouvelables sans oublier le père il visait à créer 3 entités, la première au regroupant Nucléaire et réseaux de transport d'un 2ème associant commercial et réseaux valable. La 3ème incluant les barrages hydroélectriques. Avec un risque, c'est de vendre par appartements les branches les plus rentables. Du 1er opérateur européenne d'électricité. Selon la formule consacrée. Sofia les joueurs les pertes et privatisant les profits. On comprend mieux les craintes des auteurs du texte. Nul doute qu'on devrait en connaître. Quoi qu'on en dise. Une croissance exponentielle. Du prix et de la une formation de l'électricité. Au rythme du développement d'activités très énergivores comme celle du numérique. Avec sa cohorte de serveurs informatiques. Ou encore du choix d'un Business model à Lyon du industriel du tout électrique. Pour les véhicules automobiles. Dans ce contexte aggravé par une géopolitique European internationale. En crise. Nous devons. D'orientation avec la plus grande prudence. L'État doit garder la maîtrise de l'infrastructure stratégique l'. Qui sont la production et la distribution de l'activité. D'indépendants est-ce énergétique du pays. Sa dynamique économique et l'approvisionnement des foyers français. D'autres facteurs doivent être pris en compte. Comme par exemple l'interaction entre les métiers de la filière. Qui doit être garantie par la puce public. La coordination entre la gestion des barrages hydroélectriques. Et le refroidissement des centrales nucléaires doit être assurée. Comment faire en cas de privatisation par branche. Il en va de notre sécurité nationale. Avant de conclure, j'évoquerai le texte transmis au Sénat. Il comportait articles, il n'en compte plus que 3. La majorité je entends via le la vider de sa substance. Car il touche qu'on pourrait le rachat par l'État des par des petits actionnaires minoritaires toujours en cours. À la création d'un amendement auquel je suis favorable à tous mes collègues du groupe RDSE. juste un à l'article 3 BIJ tarif réglementé. Pour les TPE et commerces de proximité. Rien ne justifie la suppression de l'article 1er visant Rodin sur des élèves pour garantir la propriété publique et l'unité du service public de l'énergie. Quant à l'article 2 modifiant. Le code de l'énergie là aussi vidé de sa substance. Et l'obliger à passer par la loi en cas de tentative de privatisation des activités d'EDF. Depuis leur production, le transport, l'exportation jusqu'aux prestations de maintenant je de sécurité. À titre personnel. Sans rétablissement de l'article 1er, à l'issue de nos débats. Je ne voterais pas ce texte car je n'oublie pas l'inquiétude des Français et du gouvernement. Face au spectre des coupures d'électricité durant l'hiver qui vient de s'achever. Je vous remercie Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Alors la PPL dont nous allons discuter de cet après-midi traite de 3 sujets, le dernier sans lien Direct avec les deux premiers que j'aborderai successivement à savoir la nationalisation d'EDF sont possible démembrement et enfin l'extension des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Alors sur la nationalisation, sans grande surprise, le groupe Les Républicains soutient le travail du rapporteur et dont je remercie ici et ça a déjà été fait la qualité. Qui a supprimé l'article 1er qui prévoyait la nationalisation. Alors nous ne disons pas pour autant que la garantie d'une non privatisation d'une activité hautement stratégique au même titre qu'ADP ne se pose pas et je vous renvoie tous ici à ceux qui ont participé au débat de la loi pacte en effet la souveraineté énergétique de la France repose sur EDF dont l'État posséder. Déjà 84% des parts du capital une montée au capital pour passer à 100% est actuellement prévu. 9. 9 milliards, 7 ont d'ailleurs été votées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative au mois de juillet dernier dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée. À un prix de 12 euros par action qui a été validée par le conseil d'administration d'EDF. cette OPA s'elle présente un inconvénient, à savoir que la procédure échappe. Presque totalement au contrôle du Parlement et c'est d'ailleurs une des critiques qu'ont exprimé les députés les républicains, tout en reconnaissant que la nationalisation n'était certainement pas la meilleure réponse à apporter et donc nous partageons également cette position l'Pass étant en cours, la nationalisation n'a pas de justification. par cette offre publique d'achat, en fait, l'État cherche à se donner les moyens de mettre en oeuvre une politique de relance du nucléaire. Nous avons envie de vous croire, même si c'est quand même votre majorité, je suis obligé de le rappeler, qui a mis fin au programme Astrid en 2019 et je parle là sous le contrôle du vice- président de l'Opecst notre collègue Stéphane Piednoir a commis un rapport publié en juin en juillet 2021 qui justement mais en avant toutes les les méfaits de cet abandon pour la stratégie énergétique française. Alors Monsieur le Ministre effectivement relancer le nucléaire est un défi technique. Quel type de réacteurs. Allons-nous construire mais c'est aussi et surtout un défi financier. Aujourd'hui le groupe EDF est très endetté. J'ai regardé 64,5 milliards de dette à fin 2022, alors qu'il pour le nouveau nucléaire alors qu'il faut en même temps financer le programme de grand carénage, près de 60 milliards d'euros en tenant compte des impératifs d'adaptation au changement climatique, la commission des finances a travailler très récemment sur le sujet alors en mars 2021, Bercy estimé que le programme de six EPR2 hors EPR2 hors frais financiers pourrait coûter entre 52 et 57 milliards d'euros, je cite, dans un scénario de bonne maîtrise industrielle mais pourrait aller jusqu'à 64 milliards d'euros dans un scénario plus dégradée. Alors Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de financement. J'ai cru lire ou comprendre qu'un appel aux investisseurs étrangers pourraient être envisagées. Cela ressort d'une visio-qu'a eu en janvier 2021, l'ancien patron d'EDF, à savoir Jean-Bernard Lévy ou encore qu'il pourrait être fait appel au fonds du Livret A qui jusqu'à présent me semble être contraire consacré au financement du logement social. Donc vous l'avez bien compris, Monsieur le Ministre, si nous n'avons pas d'opposition à cette offre publique d'achat. Nous avons de véritables interrogations sur le financement de la stratégie qui est poursuivi. et à court terme. Cette OPA elle pose une seule question qui est celle du devenir des actionnaires salariés. Alors depuis le 8 février 2023, date de clôture provisoire de l'offre les tiens d'État, l'État détient près de 96% du capital, 1,17% restent encore détenus par les salariés. Donc aujourd'hui rien n'oppose. N'empêche, éteint en fait de se retirer de la cote. Ça, c'est techniquement possible avec plus de 90% du capital mais on remarque quand même que l'OPA la clôture définitive de l'opération a été retardé notamment aujourd'hui parce que l'État fait face à un procès de de petits actionnaires qui porte notamment sur le prix de rachat des actions qui est jugée trop faible. Alors dans les faits. Le prix de rachat fixé à 12 euros constitue en fait une prime par rapport à la valorisation du marché de court terme de l'entreprise. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, l'action est descendu à près de 7 euros mais pour les salariés qui regarde en fait le prix auquel ils ont acheté à savoir. 20 32 euros pour les non-salariés et 25. Euros en 2005 pour les salariés, c'est une véritable perte. Puisqu'il y a une division par plus de du cours. Si on ajoute à ça l'inflation. Autant vous dire que la perte est encore beaucoup plus importante. Alors ces petits actionnaires, au nombre de 82.000 salariés ou anciens salariés. Il souhaite l'être maintenu au capital et la justice. Se penchera enfin rendra sa décision dans le procès en cours, le 2 mai pour cranter dans la loi le passage. D'EDF à 100% dans le giron de l'État. La commission des finances à l'initiative de Gérard Longuet a inscrit dans la PPL l'objectif d'une détention du capital à hauteur de 100% au plus tard le 1er, 2024 et dans le texte initial de la commune. Enfin dans % de ce capital pouvait toutefois être accordée aux salariés ou aux anciens salariés d'EDF alors je je vous avoue et nous en avons eu des discussions en commission des finances que je m'interroge en fait sur la mise, on la mise en oeuvre concrète de cette disposition notamment puisque dans la mesure où l'offre publique d'achat prévoit une montée à 100% du capital, par l'État, on se demande ensuite comment il serait possible d'en rétrocéder de pour 100 aux salariés. Je m'interroge aussi sur l'intérêt en fait pour les petits actionnaires parce qu'ils vont se trouver avec une action qui n'est pas liquide à partir du moment où l'entreprise n'est plus coté. Par ailleurs, en fait, aujourd'hui il faut quand même se le dire, je vous ai pas raté la date mais l'entreprise n'est pas du tout profitable en 2022, elle a fait près de 18 milliards d'euros de perte alors pour différentes raisons hein. L'existence du mécanisme Darren ce mécanisme doit disparaître en on ne connaît pas des suites qui seront données mais ces suite ont des conséquences très forte sur la rentabilité du groupe. On ne. Voilà et ça c'est des vrais sujets sur lequel il va falloir avoir des explications. Et donc aujourd'hui je me demande si en fait un versement de dividende sera possible pour ces salariés pour ses actionnaires tant les besoins d'investissement sont très importants aujourd'hui déjà en fait en terme de trésorerie EDF emprunte entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an pour venir verser des dividendes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis 2016 en fait, l'État ne demande plus de versement de dividende en cash, mais récupère en fait avec des des des des actions une montée de capital pour justement soulager la trésorerie de l'entreprise. Alors j'ai bien vu que le gouvernement a déposé un amendement à la proposition de la Commission dont j'avoue ne pas avoir beaucoup mieux compris en quoi il serait il répondrait mieux entre guillemets à à ces interrogations. Donc nous aurons je pense très certainement l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Sur le démembrement je vais pas rappeler ici le projet Hercule qui avait été envisagé en 2019 qui a été en en abandonné depuis juste pour vous dire que le groupe LR du Sénat, lui, n'a pas d'opposition de principe à ce qui a pu être écrit dans une note adressée à l'Autorité des marchés financiers à savoir poursuivre le plan de sections d'actifs à hauteur d'environ 3 milliards d'euros entre 2022 et 2024 nous n'avons pas d'opposition dès lors bien sûr que cette décision participeront d'une stratégie d'entre d'indépendance énergétique et de décarbonation, c'est la raison pour laquelle nous soutenons pleinement la réécriture de l'article de l'État possédera désormais une entreprise qui agit dans le cadre fixé par le code de l'énergie et cette nouvelle rédaction elle permet notamment de lever un certain nombre de risques qui pesaient sur les filiales d'EDF et notamment RT enfin et pour finir sur l'extension des tarifs réglementés de vente. Alors les députés socialistes eux ont prévu une mesure qui est d'une part, d'un coût financier très important. Alors le gouvernement nous annonce de 18 milliards pour tous ceux qui étaient dans cette mi-cycle au mois de décembre j'avoue que nous avons toujours maintenant de une suspicion en fait quand tu le gouvernement nous annonce des chiffrages. En matière de dispositifs d'énergie. Nous nous souvenons d'un sous-amendement à 6 milliards et enfin comme nous attendons toujours les chiffres à l'appui des assertions qui ont été faites au mois de décembre, nous vous accordons un crédit limité sur le coût de la mesure mais j'entends que ça doit quand même être très onéreux. Puisque l'application de l'article 13 du règlement européen d'octobre 2022 prévoit que l'État doit d'indemniser les fournisseurs dès lors qu'ils vendent à perte. Enfin cette extension aux entreprises de taille intermédiaire. Les étés il lui et qu'elle est contraire au droit européen, puisque les aides d'État sont temporaires sont possibles uniquement pour les TPE PME. par contre, nous vous rejoignons sur l'objectif de la mesure qui était en fait d'apporter une réponse. Aux petites entreprises que les boulangers particulièrement mais aussi aux collectivités, dont certaines en fait se trouvent exclus des tarifs réglementés, alors même qu'elles remplissent les critères de chiffre d'affaires ou de budget et de nombre de salariés mais elles ont un besoin de souscrire une une puissance installée, forte parce que par exemple pour une collectivité. C'est une grosse pompe à chaleur pour les boulangers c'est un four et donc là cette solution de supprimer la mention de 36 qui avait ah, elle est très pertinente. Je veux juste vous faire remarquer ici qu'en fait dès le début, on aurait pu le faire parce que il me semble que ça relève du pouvoir réglementaire et qu'il aurait été beaucoup plus facile de corriger une erreur dans que de devoir corriger une erreur dans la loi et enfin pour finir, juste pour vous dire qu'à l'instar de ce que mon collègue Daniel Gremillet avait pu dire au moment de l'ouverture du texte sur le nucléaire, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il nous manque une vision. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois on parle de bric brics sur le nucléaire brut sur les énergies renouvelables aujourd'hui brique sur EDF et on apparemment le plan du mur

Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Mes chers collègues. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues. Le problème d'une entreprise nationale. C'est que sa stratégie dépend du calendrier électoral. C'est une évidence qu'il me semble utile de rappeler en préambule. Alors que des éloges de l'État actionnaire vont fuser à gauche. Comme à droite. Or les cycles d'investissement industriel s'inscrivent dans le temps long. Il s'accorde mal avec le calendrier électoral. Aujourd'hui un consensus politique. C'est pourtant formé autour de la nationalisation d'EDF. Ce point d'accord est un fait rare. Car en matière de politique énergétique. L'accord est l'exception et le désaccord la règle. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a eu que 2 grands accords historiques. Le 1er c'est le Conseil national de la Résistance. Les auteurs de la proposition de loi s'y réfère d'ailleurs abondamment et nos collègues socialistes saluent l'oeuvre du général De Gaulle avec une ferveur qui, je l'avoue ne laisse pas insensible. Le second accord historique, c'est le virage du tout nucléaire avec le plan Messmer de 1974 grande année. La France s'est alors engagée dans la construction. Du plus grand parc nucléaire au monde je ne pensais pas à ça. Ce développement industriel n'a pas été remises en cause par les gouvernements suivants. Cette remarquable constance a permis à EDF de bâtir un actif stratégique hors du commun qui a très largement contribué à la prospérité de la France grâce à une électricité abondante et peuchère. Pour justifier la nationalisation d'EDF, les auteurs du texte dresse le parallèle entre la France de 2023 et celle de 1946. Mais à vrai dire, mes chers collègues, la situation actuelle ressemble bien plus au 1er choc pétrolier qu'à la seconde guerre mondiale. La crise énergétique découle d'une guerre qui ne celui produit pas sur notre sol mais nous dont nous subissons indirectement les conséquences et qui nous obligent à agir. Et d'ailleurs comme il y a 50 ans la nation se rassemblent aujourd'hui autour d'un objectif, garantir la souveraineté énergétique en construisant de nouveaux réacteurs, c'est tout le projet me semble-t-il du gouvernement qui a annoncé reprendre la possession d'EDF. Afin de garder la maîtrise du parc nucléaire. Nos collègues socialistes reprochent encore au gouvernement de nationaliser EDF pour mieux la saucissonner. C'est assez fort de café alors que c'est la gauche qui a orchestré la mise à mal de la filière nucléaire française sous François Hollande. Puisqu'on sait depuis 2015. Qu'il suffit d'une loi pour fragiliser l'avenir de notre industrie nucléaire je ne suis pas certain qu'une proposition de loi pourrait garantir quoi que ce soit. Pour moi les choses sont assez claires, le gouvernement veut nationaliser EDF et le Parlement soutient cette initiative. Le reste n'est que spéculation sur l'avenir. À l'initiative de notre collègue Gérard longuet rapporteur. La commission des finances a largement réécrit le texte je salue ces travaux. Notre groupe préfèrent très nettement cette nouvelle mouture et qui a le mérite de limiter la portée législative du texte. Cette version a également le mérite de mettre en conformité, ce texte avec le droit européen. Alors que l'Europe. A plus que jamais besoin d'union face à la Russie. Face à la Chine. Face, même parfois à nos alliés américains. Il ne s'agit pas là d'un détail. C'est la raison pour laquelle. Le groupe se partagera entre un vote positif et une abstention. Je vous remercie. Merci ma parole est maintenant monsieur Daniel Breuiller pour le groupe écologiste solidarité territoire. Madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la. Commission chers collègues je salue la proposition de loi présentée et porté par Philippe Brun à l'Assemblée nationale qui s'inscrit pleinement dans la dynamique du projet des écologistes pour une république écologique dans le cadre des présidentielles 2022 renationaliser Électricité de France et en faire un outil stratégique puissant cohérent au service de la transition énergétique. Alors bien sûr, la commission des finances à supprimer le premier article de cette proposition de loi qui formalisait un acte de nationalisation, préférant une étatisation à supprimer l'énumération des filiales constitutive du groupe public unifié visant à s'opposer au démantèlement du groupe. Bref, la commission des finances a décousu cette PPL. Bien que le projet Hercule je vous entends, Monsieur le Ministre, s'il n'existe plus puisse cacher un Hercule bis. Les choix énergétiques pour notre pays peuvent diverger les notre Champ ici largement minoritaire et vous les connaissez mais lorsque l'on défend le choix du nucléaire. On doit aussi défendre un outil 100% public chaque décision de l'État bouclier tarifaire relèvement des volumes de la reine grand carénage, construction de 6 EPR, pèse sur les comptes d'EDF, dont la situation est déjà particulièrement dégradée. À cela s'ajoute l'incompréhension totale des Françaises et des Français sur le coût de l'énergie, l'énergie, l'accès à l'énergie joue aussi un rôle social et sociétal. C'est un bien de première nécessité qui comme l'eau doit être traitée en ce sens un bien commun essentiel des 15% de reste à charge du bouclier tarifaire n'ont pas le même impact, selon qu'on habite une passoire thermique qu'on est en situation de précarité. Ce sont les revenus modestes qui sont malheureusement toujours les premières victimes de ces hausses du coût de la vie. Les bailleurs sociaux, craignent une hausse des impayés, les syndicats de copropriétaires font face également à des difficultés nouvelles comme les artisans commerçants TPE-PME. Et je souligne sur ce point, notre accord avec l'amendement du rapporteur pour supprimer le plafond des 36 KW a. Seul un tiers des entreprises concernées par le bouclier tarifaire ont concrétisé une demande d'aide des collectivités, quant à elles, ne savent toujours pas dans quelle mesure elles bénéficieront ou non des aides de l'État. La PPL initiale propose un accès pour tous aux tarifs réglementés. On pourrait attendre de la chambre des territoires un plein soutien à cette revendication de bon sens pour nos collègues maires, la situation est grave. Les écologistes alertent depuis de nombreuses années sur l'urgence à s'engager fortement dans les énergies décarbonnées sur la fin de l'abondance, la mise hors marché et hors surconsommation

pourtant espérer souvent proclamé sur ces bancs, EDF pourrait redevenir le bras armé de notre pays pour une nouvelle politique énergétique. La proposition de loi de Philippe Brun répond à cet axe majeur et stratégique du retour d'EDF, sous le contrôle de l'État. Il serait inadmissible de voir les aspects rentable du groupe, comme le développement des énergies renouvelables être privatisée, selon la bonne vieille méthode libéral. Attise privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes et les déficits j'achèverait ce propos en évoquant la place des citoyens et des salariés dans ce débat. À quel moment les Françaises et les Français ont-ils été associés à ces décisions et aux orientations prises par le gouvernement serait-il d'accord pour financer des réacteurs dont le modèle je voudrais le rappeler, on l'oublie souvent Flamanville 1 19. 1 milliard d'après la Cour des comptes quand il devait en coûter 3 3 un débat national sur les choix énergétiques de la France est indispensable. Il est même essentiel ces choix ne peuvent se faire sans une nation éclairée aux enjeux climatiques, à leurs conséquences pour l'avenir. Monsieur Julien Bargeton, vous avez la parole pour le groupe de rassemblement démocratique progressiste et indépendant. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission. Donc ce texte. Notre groupe, je le dis tout de suite votera contre, pourquoi le travail du rapporteur est impressionnant je l'remercie d'ailleurs sa démonstration était brillante. Pour autant, la question que nous posons c'est pourquoi voter ce texte. Qui ne propose plus grand chose. Le texte avait été créé. Pour. Nationaliser. EDF finalement évidemment le gouvernement a répondu, ça a été dit il y a une au PS en cours et donc ça ne se justifie plus. Le rapporteur lui-même dès l'Assemblée nationale a d'ailleurs changé le titre de sa loi en commission, et puis il avait proposé un rachat à 14 euros qui finalement est plus cher que celui proposé ça a coûté un milliard et demi de plus pour les finances publiques. C'était dommage donc ce point-là est abandonné et dans sa sagesse, le Sénat a supprimé l'article 1er. C'est plus la peine d'y, d'y revenir Il reste un 2ème point qui est le point évidemment sur le groupe unifié et, là aussi, finalement, on fait un procès d'intention au gouvernement. Procès d'intention, on a beau le répéter projet Hercule est abandonné mais on répète que il faut quand même protéger etc, évidemment l'abandon. Également de la formule qui avait été proposés. Alors l'article de certes lui n'est pas entièrement supprimée mais enfin il est largement à modifier et son contenu et finalement réduit à sa plus simple expression et il n'apporte rien par rapport à la situation existante. 3ème point, ça a été souligné par tous les orateurs. Le tarif, tarif réglementé de vente là aussi nous avons eu vont eu les explications du du rapporteur et donc sur le tarif réglementé de vente la première rédaction était une rédaction qui était contraire au droit européen. Heureusement notre rapporteur le, le Sénat a proposé finalement un dispositif extrêmement réduit extrêmement restreint qui évite les difficultés auxquelles se heurtent Quand on regarde ça. Finalement, nous avons un texte. Ah c'est ce que l'éthique tels qu'il reste et encore c'est quand les archéologues trouvent des squelettes incomplets hein c'est-à-dire bon on trouve un bout mais on ne trouve pas l'ensemble. Il n'y a plus de nationalisation. Il n'y a plus de statut spécifique. Il n'y a plus finalement aucune des des réponses à ce qui correspond à l'objet et otite de la loi initiale dans, dans ce cadre-là, avec un texte aussi privé de sa substance. Vous comprendrez que le groupe de la majorité s'y opposera, merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est maintenant à Victorin Lurel. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, à deux jours près. Nous aurions pu. Fêter l'anniversaire de la loi du 8 avril 1946. À À deux jours près. Et moi j'y vois non pas une simple coïncidence. J'ai pensé et j'ai même rêver d'avoir une sorte de connivence, de pensée et d'action, que ce qui s'est fait avec Philippe Brun et la gauche et la droite à l'Assemblée. Nationale pouvait se répéter ici. J'ai sincèrement pensé ça. Et que. Ici. Sur ces bancs la notamment. On pouvait se réclamer de ses aïeux là et que nous pourrions-nous nous considérer comme les héritiers de du Conseil national de la Résistance. Et cette affaire-là a été prolongé par toutes les générations de politique depuis 46. On l'a vu en 74, le plan Messmer, mettre en place. ce réacteur. Engagé pendant une vingtaine. D'années des baisses de prix et faire. Un prix moyen. 28% inférieur au prix moyen européen. 17 centimes à peu près du kWh 28 centimes du kW/h pour l'Allemagne ce qui donnait un Avantage compétitif considérable. À la France, ce qui est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui. Hé bien, hélas. Mon rêve est en train de sombrer dans les marécages de l'idéologie. Ce rêve de de consensus transpartisan que nous souhaiterions et que nous appelions de nos voeux. Ne dit que ce qui s'est fait la barre on peut le répéter ici en préservant l'essentiel. Est là s'envoie. À la faveur de ce texte affronter deux visions. 2 visions diamétralement opposées, un peu orthogonal de dire que. L'étatisation n'est pas une nationalisation. Et que le texte proposé par Philippe Brun et par le groupe socialiste mais pas toute la gauche en général et et un taxi a du souffle et qui porte si j'ose dire une âme. Nationaliser, c'est rendre à la nation et ça implique au moins 2 choses. C'est le transfert des moyens de production mais c'est aussi l'utilisation. De ces moyens de production. En faveur des usagers. En faveur des citoyens. Et en faveur de la nation. Or ce qui s'est fait depuis. 2000 et, à la faveur de toutes les directives qui ont été prises depuis 96. Ensuite, en 2003. En 2009, en 2010, en 2019

poser des hybridations pour des croisements de de de de capital parfois donc des privatisations rampantes. Ce que propose le groupe. Socialiste, ce qu'a proposé notre collègue député, c'est de dire, retrouvons et un sur le fond une âme nouvelle et leur confiant pas simplement EDF qui est le moteur. De la souveraineté énergétique du pays. Nous leur confions pas à une élite, quelle que soit sa qualité, quelles que soient les grands commis d'État qu'on a pu avoir ne confions pas EDF et la souveraineté énergétique du pays à une élite. Anne technostructure qui n'a fait qu'une seule chose, c'est de dire je me soumets. Le terme est fort. Je veux pas reprendre. Ce qui a pu être écrit de manière à trois en littérature, on se soumet. Et j'avoue et je m'adresse à Gérard Longuet, notre excellent collègue. J'ai été personnellement. Malheureux. De voir que le consensus qu'on aurait pu trouver, on n'a pas su le trouver une occasion manquée. De dire que la nationalisation l'Europe quelque part c'est pas son affaire. Il y a une sorte de neutralité technologique bien de neutralité juridique que le monopole soit public ou privé c'est pas le problème de de de l'Europe c'est pas son problème. Son problème c'est l'ouverture du marché et je vanter. Une chose absolument affreuses mais très belle en sémantique qui consiste à dire si il y a un monopole. Monopole de fait au monopole. Juridique. Eh bien il faut simplement que le marché soit ouvert et qui voit donc contestable. La comtesse stabilité donc à la limite c'est pas le problème de l'autre, c'est un problème national et ce que je propose, Philippe Brun et ben c'est précisément d'avoir une arme national nationaliser EDF c'est réarmer la France nationaliser EDF faire de ErDF une entreprise intégrée verticalement intégrée d'intérêt général et d'intérêt national. Ça équivaut un ministère de la Défense, c'est la défense de la France ce que. On n'a pas su faire on passe à côté, au motif d'idéologie qu'il faut faire la tarification au coût marginal qui faut corrélé le prix de l'électricité à la dernière unité mise en oeuvre, à savoir du lignite peut-être du charbon allemand mais c'est ça et. Malheureusement à le problème et quand on on veut descendre pour l'usage des Français pour le plus grand bien des des Français de dire il faut un TRV eux qui soit à la disposition de tous. Non, on change le mode de calcul et c'est le coût d'approvisionnement du fournisseur alternatif qui n'a de fournisseurs que le nom c'est ça aujourd'hui le modèle qui est soumis et auquel nous nous soumettons tous je le regrette vraiment. Il nous faut un champion national. Il faut donc la nationalisation d'EDF avec défense des intérêts. De la France il faut. Des l'illimité le pays mais pour éviter des sessions il faut hein TRV revue et corrigée et voilà ce que nous remettons pas amendement dans le texte qui vous est soumis, nous réservons le vote en attendant en étant optimiste. Que vous nous ferez au sort je l'espère. Favorable.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise énergétique n'est pas seulement le résultat de la guerre en Ukraine comme vous essayez de le faire croire. Il ne suffira pas non plus de délier les prix du gaz, d'électricité ou d'ajuster le marché européen comme vous venez d'ailleurs de le faire au profit de la compétitivité allemande. Parce que le, ce résultat c'est d'abord celui de l'Europe libérale de la fracturation de notre entreprise intégrée historique EDF en plusieurs entités et de traders qui spéculent et touchent des dividendes record. Que dire encore de la reine sera qu'est organisée sur le dos d'EDF et des usagers qui affaiblit sa capacité d'investissement qui a enrichi les acteurs alternatifs et qui Kick-Ass progressivement les tarifs réglementés de vente de l'électricité. Ce bilan, c'est le vôtre et celui de l'alliance de tous les libéraux pour faire de l'énergie une marchandise comme une autre, alors que c'est un monopole de fait et qu'elle doit donc être sorti du marché est considéré comme un bien commun. Alors la droite son n'entend rien Les à l'offensive au moins dans les mots, indépendance énergétique, souveraineté, réforme du marché européen, protection de nos collectivités. Mais quand il faut passer aux actes, il n'y a plus personne. Nous vous avons proposé en décembre le retour aux tarifs réglementés pour toutes les collectivités. Vous l'avez refusé. Sortir du marché européen en janvier et faire valoir notre exception d'une production nucléaire à bas coût. Vous l'avez refusé et aujourd'hui une loi sur la nationalisation d'EDF, refusée ou tout du moins bien amputé de l'ambition initiale du texte de nos collègues socialistes. Je veux d'ailleurs saluer leur proposition de loi qui voulait un groupe unifié avec des actions non cessibles pour éviter la vente d'actifs comme dans le cas où Enedis et qui vous empêcherait de réactiver votre projet recule, que la majorité des salariés des IEG ont rejeté aujourd'hui tout le monde l'aura compris, la situation ne viendra pas de vous et de vos mesurettes pour corriger un système qui est voué à s'effondrer. 70 ans après l'Havre du père d'EDF et GDF Marcel Paul, résistant déporté ministe communiste. Il nous faut une nouvelle loi de nationalisation de tout le secteur énergétique. Aujourd'hui nous avons un double défi décarboner notre économie et sortir 15 millions de personnes de la précarité énergétique. Il faut d'ores et déjà préparer l'avenir sans vous car vos échecs et vos renoncements nous conduisent dans le mur. Plus de 50 milliards de bouclier tarifaire Darren supplémentaire de filet de sécurité n'auront rien réglé ni stabilisé, mis à part les profits d'acteurs alternatifs rapaces. Je propose donc que nous travaillons dès maintenant à un grand projet à la hauteur de Marcel Paul et de ses camarades un groupe public sous la forme d'un Epic. Il regroupe aurait en son sein EDF mais aussi Engie et Total énergies à 100 pour nationalisée et qui pourrait porter le nom de GODF groupe Énergie de France et là vous allez me dire mais combien ça va coûter. Eh bien l'affaire coûtera probablement une centaine de milliards d'euros, mais après tout, ce n'est que le double de ce que vous avez gaspillé l'an dernier. Ce groupe détiendrait un monopole public. Il serait un groupe intégré qui assuré la production, le transport et la distribution qui mettrait fin à la reine. Un groupe qui rétablirait l'ensemble des tarifs réglementés. Ces tarifs, sur la condition pour protéger les usagers les TPE-PME les collectivités et les grandes entreprises qui ont besoin d'une vision à long terme. Ils sont la condition pour garantir la stabilité pour réindustrialiser le pays et pour lui redonner la compétitivité dont dont on a tant besoin face à l'Asie et aux États-Unis. Il faudra pour cela renforcer le statut des IEG protéger tous les travailleurs et travailleuses de la filière, les salariés et celles et ceux qui sont aujourd'hui des sous-traitants ce statut et la condition pour maintenir les talents dont nous avons besoin pour la filière pour le pays et pour notre sécurité. Pour finir, Marcel Paul avait demandé à ses enfants, de veiller à vos attaques et de protéger cette entreprise qu'il qualifiait très justement d'instrument fondamental de la vie du pays. Vous qui avaient tout détruit et qu'il voulait continuer vous ne trouverez sur votre route avec ses petits-enfants et arrière- petits-enfants prêt à tout reconstruire. Je vous remercie. Enfin dernière intervenant Michèle Canet fait pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, le groupe de l'Union centriste vaudrait tout d'abord remercier sincèrement le rapporteur du texte. Gérard Longuet. Pour. La pertinence de ces analyses et la manière dont il a exposé la situation car finalement. On est sur un texte qui. Par notre fête à bord de tout simplement la politique énergétique de notre pays puisque c'est de cela qu'il s'agit. On a eu d'autres textes. Qui. L'ont évoqué, je pense au texte sur le nucléaire ou l'accélération du nucléaire. Le texte sur l'accélération des énergies renouvelables. Mais je crois que le débat n'a pas été clos et mérite d'être largement poursuivies et c'est l'occasion. Lors de l'examen de ce texte de le faire. Monsieur le Ministre, alors le groupe de l'Union centriste, disons-le clairement être attaché à ce qui est un mix énergétique qui permette d'assurer véritablement la souveraineté de notre pays en la matière le mix énergétique d'ailleurs ne doit pas s'arrêter à l'électricité. Je crois qu'il faut aussi que l'on soit attentif. À l'énergie d'origine du gaz par exemple du gaz. Bien Bien sûr, renouvelable. Mais aussi d'autres formes de production énergétique. Qui sont importantes pour pouvoir permettre demain à d'autres pays d'être particulièrement souverain autonomes en matière d'énergie et chacun sait et particulièrement le ministre de l'Industrie que vous êtes combien l'énergie état d'éléments indispensables pour la compétitivité de nos entreprises. Alors. Sur cette nationalisation bien sûr je ne partage pas du tout les propos qui viennent d'être tenus par notre collègue Fabien Gay, non. D'avoir. D'avoir un, un système monolithique ne permettrait pas de répondre au défi que auxquels nous sommes affrontés. Dans cette perspective énergétique tout simplement parce qu'il faut qu'on trouve une multitude de solutions et sa multitude de solutions sera bien sûr l'apanage d'un grand nombre d'opérateurs et si ces opérateurs peuvent effectivement dans le cadre légal que nous incitions. Pouvoir s'exprimer, hé bien nous pourrons apporter des réponses. Aux besoins de nos concitoyens en la matière. Disons-le assez clairement aussi peut-être qu'il faut s'interroger sur. La perspective de nationalisation de d'EDF parce que finalement ça coûte beaucoup d'argent, plus de 8 milliards d'euros. Était-il nécessaire. De procéder à cette renationalisation ne va été le pas mieux consacrer cet argent important à à moderniser notre parc de production, c'est franchement une question dont il faut se poser. Mais ceci étant, la décision a été prise, donc il faut qu'on en prenne acte et nous le faisons au niveau du, du groupe de l'Union centriste. Alors ce texte bien sûr à bord de différentes choses sur cette. Sur cette acquisition d'actions. Nous dirions que dans l'esprit de ce que fut la loi pacte. Votée il y a 5 ans. Nous pensons que. Il faut quand même favoriser l'actionnariat. Populaire l'actionnariat salarié, en particulier la question du partage de la valeur et pour nous, membres du groupe de l'Union centriste, quelque chose d'important Nous nous interrogeons c'est vrai sur. L'amendement que le gouvernement a déposé limitant les choses et nous préférions que. Nous en tenir à la rédaction du du rapporteur car il nous semblait qu'il avait trouvé le juste compromis. En la matière donc. Nous pensons que il faut quand même tenir compte de l'importance de la motivation de l'ensemble des salariés d'EDF et puis. Le rapporteur a également évoqué bien sûr une des principales dispositions du texte qui concerne l'extension du tarif réglementé. Nous pensons au niveau du groupe de l'Union centriste. Bien sûr qu'il faut s'en tenir aux règles s'européenne que nous avons édicté d'autant plus que le marché est ouvert au niveau européen justifiant. Qu'il y ait un respect de ces règles et nous devons dire que la proposition qu'a formulé le rapporteur de comptes circonscrire. Aux TPE. Le bénéfice et de l'étendre en faisant sauter la barrière des 36. Nous semble être une solution tout à fait pertinente car finalement à apporte des réponses. Ah bon nombre de situations que. Chacun d'entre nous avons pu relayer auprès du gouvernement. Tenant compte de la réalité observée sur le terrain. Ces boulangers qui effectivement avait des compteurs d'une puissance supérieure à 36.

pertinente à cet égard. Voilà donc quelques éléments que nous souhaitons au pouvoir. Évoquée aujourd'hui et puis nous allons pouvoir nous exprimer également dans le débat qui s'ouvre à l'instant, merci de votre attention.

Merci madame la la présidente. Monsieur le Ministre, chers chers collègues. Les expressions un. Discussion générale. Que nous venons d'entendre l'montrer. Il y a en réalité dans cet hémicycle 2 approches très différentes. le libéral très libérale de la commission des finances et de son rapporteur, Gérard Longuet. Qui laisse ouvertes toutes les options de cession ultérieure de filiales. Et celle-là notre. Centré sur le confortement de notre souveraineté industrielle en matière d'énergie décarbonée. Nous voulons garder dans le giron national EDF et toutes ses filiales. Coeur de métier. La production dans toutes ses formes. Énergies renouvelables hydraulique nucléaire thermique, le transport et la distribution RTE et Enedis sans rien toucher aux prérogatives et au statut particulier, eu égard au droit européen qui sont les leurs. Ainsi que les services, services énergétiques que rend le groupe aujourd'hui. Comme les aime imports et les exports d'électricité. Monsieur le Ministre. Vous avez laissé entendre que c'était le marché européen qui avait institué de l'exportation et de l'importation. L'exportation et l'importation existait bien avant la mise en place du marché européen. Je tiens à le rappeler ici. Comme je tiens à dire que porter la part du capital d'EDF SA. À 100%. Pour l'État n'empêchera pas des cessions de capital ou de filiales ultérieurement. Et je regrette. La porte reste ouverte pour des opérations de restructuration. Comme Hercule. L'objet de ce texte était. De garantie d'apporter des garanties par rapport à ça, ça ne sera pas le cas. Donc ce que nous voulons, je le répète, c'est une société EDF. Nationalisée dans le cadre de groupements public unifié et ça sera le sens mais des amendements que nous allons défendre. La parole est maintenant Monsieur Victorin Lurel. Merci madame la. Présidente. Oui. Le groupe auquel. J'appartiens. Tiens. Ah la nationalisation à une loi de nationalisation de l'entreprise. EDF. EDF n'est pas une simple entreprise. C'est une arme. C'est un bouclier. Et penser un seul instant qu'une opération. Simplifié une offre publique d'achat. Donc une étatisation donc une montée en capital suffit pour garantir. L'unité, la cohérence, l'intégration et éviter les dérives que l'on a pu constater pendant une vingtaine d'années dans la gestion et le management de cette entreprise est une illusion. C'est la raison pour laquelle nous tenons au principe de la nationalisation inscrite dans le préambule. La constitution de 2 46 il est repris dans le bloc de constitutionnalité si finalité qui est le nôtre. À savoir, ça doit devenir un bien commun bien de la nation qui doit être. Transféré ses moyens de production transférée mais surtout utilisé au bénéfice des nationaux. Voilà ce que l'on dit. Pour autant, on ne dit pas de s'enfermer et de ne pas faire dans l'international. On ne dit pas de ne pas faire dans la rotation d'actifs on veut préserver le coeur de métier. De EDF. C'est la raison de notre. Amendement, à savoir une entreprise nationalisée. Hurel, est ce que c'est vous qui présentez l'amendement numéro 2. C'est fait mais je le répète, ça me donne juste. Un, un temps pour dire on veut. Consolider et unifié EDF, et tenir à ce que Philippe Brun. Un groupe public unifié. On le fait pour la SNCF. J'ai entendu moi des arguments assez spécieux pour dire c'est une simple occurrence et qu'on ne pourrait pas le répéter. Non, on le répète et on a vu nos collègues communistes Fabien Gay déposer un amendement sur le CNR pour dire mais ça s'appelle bien une société anonyme. Hein. Intégré. Intégré hé bien on a proposé en commission. Ça a été refusé le mot national a été retenu mais on tient donc à cette entité et à, à, au concept de nationale et de nationalisation. Merci. Alors avant de donner la parole à Fabien gay pour présenter l'amendement numéro 8 qui est identique, j'informe le Sénat et que je suis saisi d'un chapelet de. Demande de scrutin public sur ces articles est ce qui vous permettra de vous préparer. Allez-y. Quand on a, on peut Pessin chapelet. Julien. Merci madame la présidente, monsieur le midi. Mes chers collègues. Nous nous tenons comme nos collègues socialistes au retour de l'article 1er et au terme nationalisation parce que ce n'est pas exactement sur le ministre. Ce que vous êtes en train de faire, en rachetant les actions. Des actionnaires minoritaires qui étaient institutionnelles ou actionnariat salarié ce que vous faites en ce moment c'est une régate étatisation et vous sortez EDF de la bourse, c'est-à-dire qu'EDF ne sera plus coté en Bourse. Ça sera donc une entreprise. Qui aura un capital 100% public mais dans lequel et vous le savez très bien puisque ça sera toujours sa structure une SA société anonyme vous créerez une Holding comme vous avez fait la SNCF et d'autres entreprises publiques, ce qui ne vous empêchera pas de choses d'abord hein de filialiser la 2ème chose de céder des actifs d'Dalkia Enedis et il va falloir que votre gouvernement répondent. Est-ce que oui ou non vous voulez céder Dalkia Enedis et la 3ème chose c'est que la Holding de tête sera 100% nationale, mais ça vous empêchera pas en réalité de CD aussi et d'ouvrir à des filiales à des capitaux privés et donc ce n'est pas exactement la même chose que vous êtes en train de faire et le projet que nous voulons la nationalisation et je me permettrais mais dans un débat à gauche tranquillement. Je pense que nous devrions ajouté à nationalisation, la transformation de la société SA en Epic, établissement public que nous connaissons, extrêmement bien, donc ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des assimilés et le statut des IEG va avec mais la transformation en épique elle nous garantit d'autres choses, donc je vous le dis hein. Monsieur le Ministre, ils nous nous tenons à ce que l'article 1er soit rétablie. Comme l'avait adopté l'Assemblée nationale.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre et chers collègues. Je je redis ici la, la, la nécessité de nationaliser le groupe EDF. Pour éviter tout tout démantèlement ou démembrement. Et. D'ores et déjà à ce stade du débat. Je voudrais attirer votre attention et ça permettra peut-être au au Ministre de de nous répondre dans dans quelques instants. la la problématique hein parce que ça n'est une des 2%. De capital propriété des salariés. Cette disposition va fragiliser. L'hydraulique la production hydraulique. Et probablement réouvrir le débat. Relatif. À la mise en concurrence des concessions. Hydraulique. ça serait une première étape de de démantèlement de démembrement de l'entreprise obligatoire. Qu'évidemment on veut éviter et qu'on pourrait éviter effectivement. En votant cet article 1er appelant à la nationalisation du groupe EDF. C'est pas une petite affaire. S'est avéré en termes de risques juridiques. Et je voudrais que le gouvernement peut être le rapporteur nous éclaire là-dessus. Parce que les conséquences. Pourraient être coïncide érable considérable. Je vous remercie. Merci je vais donc. Monsieur Aubry. Ah vous avez la parole. Merci madame la présidente, je, je comprends bien sûr. Le choix de l'étatisation. Fait par le gouvernement et est soutenu par le rapporteur. La situation actuelle d'EDF. Le coût du grand carénage le coût très optimiste des 6 premiers EPR 3 fois moins cher que Flamanville. Tout ça suppose effectivement qu'il puisse y avoir un acteur public c'est-à-dire nous-mêmes les contribuables pour venir. Financer ces dépenses considérables. Mais ça n'est rien à voir avec le projet initial de nationalisation. C'est un autre choix qui a été proposé par nos collègues et qui est défendu sur ces bancs de la gauche, le choix d'avoir effectivement un outil des politiques énergétiques, donc évidemment je voterai ces deux amendements identiques de mes collègues Lurel gay au nom de mon groupe et je le redis, il est temps d'avoir un débat sur la politique énergétique de notre pays et pas de débattre par petites tranches tranches d'EPR tranche d'accélération ou débats de cet après-midi de ces sujets. Bien s'il n'y a plus de demandes d'explications de vote sur ces amendements monsieur. je trouve dommage quand même que en une minute. Le, le ministre nous répondent pas quand même on a posé des questions sur la question. La différence entre re-étatisation et nationalisation et on vous pose une question simple, est-ce que vous vous engagez ici devant le Parlement à ne céder aucun actif. Enedis et Dalkia par exemple pourrait nous dire ce que vous vous êtes très à propos pour dire, il y aura pas d'Hercule. Très bien. On en doute, mais est-ce qu'il y aura oui ou non des cessions d'actifs puisque il y a pas de projet caché. Dites-le ici devant le Parlement a engagé, vous au moins sur cette question, je vous remercie madame la présidente. vais donc. Il n'y a plus d'explication de vote. Je vais donc. Métro ouvrir le scrutin public dont nous avons été saisis pour les abonnements de et huit par le groupe Les Républicains, le scrutin est ouvert.

ouvert. Ça ne demande à voter le scrutin est clos. Votants 343 338 pour 99 contre 239, le Sénat n'a pas adopté

le présenter. Sur l'article, madame la présidente. Franck Montaugé présentera cet article. Cet amendement. L'amendement numéro 3.

Nous tenons à avoir. Rétabli. La version originelle et à délimiter. Le périmètre des activités. De l'entreprise EDF. SA. En. Production en transport et en transport en. À 11 Denis en distribution commercialisation. Est en prestation de services énergétiques. il y a une nuance, c'est vrai qu'on a corrigé la chose sur le transport, autant on veut voir EDF rester si j'ose dire, une présence capitalistique au sein de RTE. Et je dirais Enedis autant nous respectons l'indépendance opérationnelle et stratégique. de RT. Donc l'écriture telle qu'elle est soumise. Et conforme au droit européen et conforme au code de l'énergie. Monsieur Gay, vous nous présenter l'amendement 9.

en deux en deux minutes, je je suis d'accord avec le rapporteur tout à l'heure qu'a dit qu'on avait déjà un groupe désintégré parce que c'est vrai. Qu'avant. EDF. Produisez transporter distribuer aujourd'hui ce n'est plus le cas pour des questions de concurrence, juste pour donner. Un peu qu'on fasse un peu le bilan de la libéralisation donc aujourd'hui. Enedis transporte mais dans le transport. Vous savez d'électricité comme la. Accompagner de d'un point à un point B. Vous en perdez c'est comme ça vous avez-vous par terre sans et vous arrivez à 95. Donc Enedis doit racheter de l'électricité mais peut pas le faire à EDF qui la détient pourtant quasi à 100% et doit donc la racheter au marché à des concurrents Directs et notamment la reine et donc sans provision ma marraine mais chez le concurrent Direct d'EDF pour lui-même réinjecté dans le réseau pour servir ce concurrent Direct vous voyez. Lorsqu'on sait tout ça évidemment c'est extrêmement compliqué. Mais quand même. Bravo, vous avez réalisé un chef-d', oeuvre d'une usine agace qui conduit quand même à des aberrations totales. on voit en 20 ans. Libéralisation du secteur de l'énergie qui est un monopole de fait et qui donc doit être sorti du marché. Tout ce que ça aura coûté à notre pays à EDF sur le dos des usagers. Franchement on n'en est plus là et donc je repose la question, Monsieur le Ministre, est-ce que on va garder un groupe intégré et est-ce qu'il aura oui ou non des cessions d'actifs avait la étatisation que vous voulez et notamment Dalkia Enedis et voilà je vous rends même qu'un secondes madame la présidente. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements. La commission, madame la présidente et défavorable à ces trois amendements je je reconnais la volonté. De Victorin Lurel et son groupe de s'efforcer de d'obtenir une un vote conforme à celui de l'Assemblée et de faire. Des gestes d'ouverture sur les réalités d'un marché qui est désormais cher Fabien Gay parfaitement concurrentiels et personne ne songe à le remettre et quand vous dites que. ne naturellement mais vous êtes assez largement minoritaire en France et en Europe, ce qui pose un problème pour l'autorité et l'aboutissement de vos propres projets. Il se trouve que l'électricité est désormais produit de façon très différente. Nous avons en effet le système nucléaire qui est un système unitaire en France nous avons. Le thermique qui n'est plus un système unitaire turbines à gaz ou même charbon puisque si Cordemais et EDF. Saint-Avold et gazelles et Gardanne tout temps et nous avons en ce qui concerne les énergies renouvelables. Des milliers de producteurs. Alors certains d'entre eux sont très importants, je pense aux éoliennes d'Engie ou de Total. D'autres sont des tout tout petits producteurs, y compris des des particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques, vous ne les priverait, plus de la liberté de produire qui s'accompagne évidemment d'une décision d'investir. J'ajoute et je me tourne vers mon excellent collègue Breuiller qui a des convictions écolo que je respecte mais que je ne partage pas. Il a cependant la passion les économies locales et circulaires qui passe en particulier par des réseaux autonomes qui ne serait d'ailleurs pas interconnectés, ce qui entre nous est quand même assez dangereux. Mais ce sont des producteurs indépendants qui n'entendent plus perdre leur indépendance. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de tenir compte d'un système dans lequel la production électrique est dominé par EDF. Et je m'en réjouis et je m'en réjouis parce que c'est une production de qualité, mais ce n'est plus une production monopolistique et c'est la raison pour laquelle Enedis comme RTE doivent être indépendants pour qu'elles offrent des services sur une la base d'une loyauté et d'une équité dans les traitements des producteurs indépendants qui auront demain comme aujourd'hui le droit de produire. J'ajoute que tout cela n'est quand même d'une construction européenne dont la signature a été donné en 2002. À Barcelone. Par l'ensemble un par un Conseil européen. Donc l'ensemble des gouvernements, je crois que la France était représentée par Lionel Jospin qui n'est pas un dangereux libéral. Quel est l'avis du gouvernement. les parts manquant d'EDF et en faire une société détenue à 100%, c'est pas pour, dans la foulée envisager quelques sections quelques cessions pardon de parts du capital d'EDF. Quelle qu'elle soit. Cela dit la priorité numéro un d'EDF aujourd'hui, c'est de restaurer sa crédibilité financière et ça passe déjà. Par des cessions d'actifs qui sont évidemment des cessions d'actifs marginaux qui sont déjà engagés à hauteur de 3 millions d'euros et donc si votre amendement est adopté aujourd'hui vous fragiliser la consolidation d'EDF. Par ailleurs, je le rappelle, le nouveau président directeur général d'EDF doit remettre au gouvernement et vous aurez évidemment toute la la la la la liberté pour l'auditionner une nouvelle feuille de route. Dont les objectifs sont essentiellement de 3 types. Hein. Restaurer les capacités opérationnelles d'EDF donc il faut le reconnaître qu'elles ont un peu pêcher régulière la consolidation financière et trois, la manière dont les investissements futurs et notamment la priorisation de ces investissements ont être proposé à l'actionnaire nous tous par la direction et donc évidemment aujourd'hui s'engager de manière. Totalement ferme. Hein. Une entreprise. Voire même une entreprise gelés y compris RTE Enedis puisque certains des amendements que vous proposez aujourd'hui propose de geler le tout en totale non conformité avec le droit par européen mais permettant même en danger l'indépendance d'RTE qui elle est essentielle dans le schéma actuel, donc oui la vie est totalement défavorable à ces amendements et j'en profite pour rappeler aux sénateurs. Non, je ne doute pas qu'il en est au courant que les pertes d'Enedis sont rachetés au coût de la reine à EDF et en aucun cas sur le marché à des prix exorbitants. Ah non non non je vous enverrai les textes.

d'être compétitif grâce à une énergie payé en gros au prix coûtant sur des investissements qui ont été payés par la représentation par le, par l'État français par la nation depuis 70 ans. Il va falloir le remplacer ce ce dispositif mais j'espère qu'on trouvera un dispositif qui permettra encore de réindustrialiser la France plutôt que de la désindustrialisé avis défavorable sur ces trois ou quatre amendements merci.

Correspond à ce que nous proposons dans cet amendement. En matière de production. De développement. D'exploitation et de maintenance de prestation de services énergétiques de transport et cetera voilà. Et dans le respect, contrairement à ce qui vient d'être dit strict du droit européen notamment concernant RTE et Enedis. Voilà parce que cette c'est l'intention de de de de cet amendement. Et je pense que ça ça, Un vote favorable. Donc encore une fois dans le cadre d'un groupement public. Unifiées. Et et d'un capital préserver et je et je redis ici que la question des 2% de capital des salariés est un problème majeur. Monsieur le ministre si vous pouviez nous répondre là-dessus. Ça serait très très très très si madame la présidente. Monsieur le Ministre, je vous répondrai pas sur la reine, puisque je crois qu'il y a il y a un amendement qui viendra. Sur le droit européen juste parce qu'on on a déjà ce débat depuis 2 ans. Tout le monde en train de s'asseoir sur le droit européen, sauf nous. les Portugais, les espagnols nous ont montré la voie, sur le marché européen en obtenant une dérogation. Les Allemands eux ils ont pas besoin. Ils nous ont encore tordu le bras il y a 15 jours et donc nous avons signé une réformette du marché européen qui continue à avant d'avantager l'industrie allemande à notre détriment et il s'assoit sur le droit européen à chaque fois qu'ils en ont besoin en réalité protéger leur industrie, ça a l'air de déranger personne. Mais par contre nous. Il faut absolument rester dans les clous du droit européen. Nous sommes les derniers à le faire, moi c'est pas grave si ça vous fait plaisir mais si c'est ça la réalité et la réforme du marché européen ici personne me dira les yeux dans les yeux qu'sera favorable à l'industrie française. Personne ne peut m'expliquer ça et. Je finis par vous dire que madame Lavarde vous a posé une question. Qui était extrêmement intéressante, 60 milliards de dettes et vous le dites. Le nouveau PDG Luc Rémont va devoir vous rendre une feuille de route sur savoir comment se désendetter et évidemment, comme investir. Donc. Vous êtes responsables en partie puisque la reine plus ça a coûté 8 milliards 4 l'an dernier quand même et donc on pourra continuer à biberonné les acteurs alternatifs. Ça continue à dépecer en réalité EDF et j'y reviendrai à racketter les usagers comment ils vont se désendetter, de 60 milliards. Est-ce que une des propositions sera de accélérer la cession d'actifs et notamment ben on commencera par les actifs qui rapporteront le plus Dalkia Enedis. C'est ça la réalité. Je vous remercie madame la présidente. Merci madame la présidente, j'aimerais que Monsieur le Ministre, puissiez répondre à la question de mon collègue Montaugé. Sur la présence des salariés de la participation, l'actionnariat des salariés 2ème chose vous avez évoqué. Les avantages de la reine, bien sûr qu'il y ait qu'il y en a mais moi j'ai une autre lecture. On a une autre lecture sur ce que veut dire toi absorbé et payer. Premièrement, acheter des renouvelables, qui sont très largement subventionné et qui sont intermittents mais il faut le faire et revendent au prix du marché. Ensuite la de 25% de l'énergie nucléaire historique. Sur le. Marché. À 42 euros, tout ça, c'est EDF qui accepte ça et je suis pas sûr que ça profite quand c'était car de compétitivité que nous avons avec cette composante. Historique amorti hé bien profite aujourd'hui à la à l'industrie française et à la à la nation. S'il n'y a plus d'explications de vote, nous allons donc passer au 2ème scrutin public sur d'abord sur l'amendement numéro 3. Je rappelle que cet amendement reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert.

non. Votants 343 exprimés, 339% contre 239 il y a deux autres scrutin public sur les amendements ne fait dit c'est ce que tout le monde serait d'accord pour qu'on considère que c'est le même vote.

c'est un amendement de repli puisque nous avons perdu le débat sur la renationalisation. Nous, nous n'aurons pas les piques au moins que comme la Compagnie nationale du Rhône. Cela ne reste pas une SA mais une société anonyme au moins d'intérêt général, voilà ce que nous demandons. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. N'a pas adopté cet amendement. Donc c'est un avis défavorable, j'imagine Monsieur le Ministre. Il y a encore un scrutin public sur cet amendement, on fait comme on a fait il y a un instant, c'est le même vote. OK même votre monde est d'accord, donc il n'est pas adopté il y a un amendement 19 du gouvernement. Madame Madame la présidente. Cet amendement me permet d'évoquer le sujet de l'actionnariat salarié. Dans leur discussion générale ou dans la discussion d'amendements par un certain nombre des sénateurs et les sénatrices ici présentes. Nous proposons. Je dirais, de rendre possible de l'actionnariat salarié au sein de l'entreprise EDF, même si pour être très clair, nous ne jugeons absolument ni souhaitable, ni même envisageable à très court terme. Pourquoi, parce qu'on est justement en train de racheter 100% du capital. Pour restaurer la capacité financière de l'entreprise. La capitale capacités pardon. Et sa capacité à investir donc non seulement faire ce genre d'opération aujourd'hui. C'est sans doute pas à faire un cadeau aux salariés, alors que la rédaction actuelle nous y forcerait dès le 1er janvier 2024 les forces sans doute à faire une très mauvaise opération financière mais au dollar serait évidemment totalement anachronique alors qu'on était exactement en train de faire le contraire, c'est-à-dire de racheter les minoritaires, y compris certains d'ailleurs détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié, vous le savez aujourd'hui l'État détient déjà 90% du capital et pourrait. Légalement, racheter les 10% restants du fait d'un certain nombre de recours qui ont été déposés l'état, le gouvernement s'est engagé à tendre que ces recours soit jugé, vous l'avez dit, madame la sénatrice début mai avant. Au cas où ces recours serait rejetée de procéder à l'acquisition de la totalité du capital. Vous avez voté dans l'article 1, le fait que l'État doit un tiers 100% du capital. Et vous nous demandiez pourquoi cet amendement était indispensable aujourd'hui parce que du fait de cet article hein si jamais nous souhaitions si jamais l'entreprise souhaitait si jamais l'actionnaire acceptait de procéder à la mise en place d'un dispositif d'actionnariat salarié en 2024, 2025 ou 2026, ça serait tout simplement impossible

Sans nécessairement un passage au Parlement à la direction de proposer un programme d'actionnariat salarié évidemment sans obligation doit en inaugurer pour laisser à l'entreprise. Le temps de ce je dirais remettre en forme avant d'y procéder, merci. Madame la présidente, mes chers collègues, la commission a exprimé un avis de sagesse. Parce que cette affaire est en effet très difficile et très sensible. Nous avons un immense respect pour l'entreprise EDF ce qui nous a conduits à soutenir un amendement de notre collègue Victorin Lurel qui fait d'EDF et on. Dans le texte de la commission, une entreprise d'intérêt national, ça n'a pas de signification juridique autre que le reconnaître que la communauté des salariés dans l'histoire d'EDF a bien fait son travail. 82.000 salariés en 5 salariés sont Tech ont été actionnaire où sont actionnaires d'EDF. Aujourd'hui c'est l'expression d'un engagement dans leur entreprise qui confortent cette image de communauté, c'est la raison pour laquelle. La Commission. Souhaitait et avait proposé un texte qui. Donnait cette possibilité en l'encadrant dans une période courte. Et c'est le période le problème de la période courte qui apparaît avec force. Madame Lavarde la fait valoir dans le débat en commission. Nous avons trop d'inconnues, celle que j'ai évoqué à la tribune sur l'avenir du marché. L'avenir de l'organisation. Le marché de l'énergie électrique. très optimiste. Il est, il sera nécessairement en croissance parce que la décarbonation de notre société passe par l'électricité. Donc je n'ai simplement aucun doute sur le fait qu'il nous faudra produire de plus en plus d'électricité et que l'entreprise qui a le bénéfice de l'expérience de plus de 50 ans de 58 réacteurs nucléaires est quand même mieux placées que n'importe quelle autre entreprise pour conquérir des des positions nouvelles forte. Mais ce n'est pas encore dans un cadre clair et donc nous avons besoin de savoir si il y aura des contrats. D'achat de long terme autorisé s'il y aura des contrats par différence si il y aura la possibilité d'acheter des parts de centrales nucléaires pour avoir des droits de tirage comme Excellium on profite je sais de quoi je parle, je l'ai mis en place comme Ministre de l'industrie aux siècles précédents. Donc nous avons toute une série de questions qui méritent. D'obtenir des réponses avant que d'engager l'économie des salariés dans ce qui reste toujours une aventure vous savait très bien que lorsque l'on fait de la publicité pour une offre. on dit. N'est. Les performances passées n'engage pas l'avenir et donc pour protéger. Les salariés, nous souhaitons. Sagesse, sagesse positive à l'égard de l'amendement du gouvernement.

Monsieur Moto G, vous avez. Et merci madame la présidente. Nous n'avons pas eu d'explication claire du ministre sur les conséquences juridiques de cet amendement. Sur les concessions hydrauliques dans le cadre européen. L'analyse que nous en faisons. C'est qu'avec cette mesure vous lancer une torpille contre le groupe EDF, je pèse mes mots. Vous allez devoir mais je pense que c'est peut être votre intention première. Détacher l'hydraulique du groupe EDF donc démantelés et ce sera le le le le commencement. Peut-être de la fin. À l'instar de ce qui s'est passé pour l'entreprise nationale qui était Gaz de France à une époque alors. Voilà. Cela nous lasse pas de de de de nous inquiéter. Ce débat est crucial. S'il reste une part de capital. Autre que d'État. Au sein du groupe. On va être, vous allez être confrontés à cette question là, je pense que les territoires vont peu apprécié de voir mis en concurrence peut être par obligation. Les concessions hydrauliques sur le territoire national. Est-ce qu'encore une fois, vous pouvez nous préciser votre analyse par rapport à ce point. Extrêmement important. Merci. Qui dit quand même que donc le l'amendement vise à ce que les anciens salariés pourront donc être actionnaire d'EDF, de sorte à ce que les salariés du groupe ne soient pas forcés de vendre leurs titres lors du départ de l'entreprise. enfin, ce que je ne crois pas c'est que vous venez de nous réexpliquer que vous allez monter à 100% du capital. Donc à un moment ils ont déjà vendu leurs titres, ils peuvent toujours être dans l'entreprise et donc l'exposé des motifs semblent dire qu'ils ont encore ces titres et qu'il ne serait pas forcés de les vendre au moment où ils partent alors je. S'il y a quelque chose qui est pas très clair et de. C'est toute la procédure de mise en oeuvre en fait c'est soit l'état détient 100% du capital et on dit et ça peut permettre et pour tout un tas de raisons, j'ai exposé tout à l'heure à voir sa pertinence, notamment pour venir permettre le financement de ces investissements conséquents qui ne vont pas permettre le financement Dividendes, soit on dit qu'effectivement on veut apporter quelque chose à ses salariés qui ont fait l'histoire du groupe qui ont fait l'histoire de notre politique. Énergétique et notre notamment notre politique nucléaire mais à ce moment-là il faut que ce soit clair pour eux et là j'avoue que ça ne l'est pas.

ne change rien aux questions que vous vous posez, monsieur le sénateur, donc on va s'assurer que j'ai bien compris votre question et si vous m'y autorisez, on répondra par écrit, mais le fait que la l'actionnariat salarié soit optionnel ou ou ou obligatoire, à mon avis, ne change en rien les débats qu'on a par ailleurs sur les concessions hydrauliques sur lesquels il faut évidemment qu'on soit extrêmement ferme. Donc je vais essayer de clarifier effectivement. Nous achetons 100% du capital. Et donc si le jugement du tribunal des muets conforme à ce à quoi on s'attend on aura dans la foulée, la capacité d'acheter les 5% du capital restant l'État détiendra 100% du capital. Si Si dans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans la situation de l'entreprise et dans une meilleure situation on l'autorise par cet amendement éventuellement à envisager et à mettre en oeuvre un accord d'actionnariat salarié sans avoir à repasser par le Parlement. Et cet accord d'actionnariat salarié. Comme c'était le cas dans la dans l'accord précédent permet à la fois de. Aux salariés d'acheter des actions du groupe et de les détenir et de les conserver ultérieurement au cas où il quittera le groupe par exemple pour prendre leur retraite donc c'est juste pour reproduire. En avant des dispositions qui existaient, d'ores et déjà dans l'accord d'actionnariat salarié aujourd'hui et c'est en aucun cas évidemment l'idée de prolonger les actions détenues aujourd'hui par des salariés, au-delà de l'achat qui, je le confirme, passera bien à 100% du capital jusqu'à. Jusqu'à ce qu'on en décide autrement dans le cadre de la gestion d'entreprise et dans le cas d'un accord d'actionnariat salarié. Merci monsieur. Merci madame la présidente. Comme quoi l'actionnariat salarié. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous vend. Tous les jours puisqu'à priori pour vous. Ça devrait même remplacer le salaire, intéressement, participation, actionnariat salarié, c'est bon pour vous et les salaires. Pas du tout. Cette affaire d'actionnariat salarié sur EDF. On va les défendre parce que c'est une compensation. Il faut se rappeler l'histoire. C'est pas historique l'actionnariat le salarié chez EDF. Ça a commencé en 2005 lorsque vous avez décidé d'ouvrir au capital et donc c'était en réalité une compensation pour les salariés, 130.000 à l'époque sont devenus actionnaires salariés et ils auront perdu de l'argent parce que ceux qui ont racheté le titre en 30 euros et qui seront obligés le revendra 11 ou 12 euros auront bien perdu. De l'argent et donc là vous expliquer et c'est pour ça qu'ils vous ont attaqué notamment sur une question et les dernières décisions que vous avez prises, notamment les 20 TWh supplémentaires qu'on fait perdre 8 milliards IV et qui ont fait baisser. En réalité le prix de l'action au moment où il est sorti en bourse et c'est pour ça que vous allez pouvoir le racheter entre 11 et 12 euros. Donc là vous nous expliquez que vous êtes en capacité. En quelque sorte de spolier les actionnaires salariés aujourd'hui. Vous allez reprendre 100% et peut-être demain vous allez leur reproposé. De redevenir actionnaire salarié. Il y aura un problème quand même le ministre ou vous voyez bien quand même. Personne ne comprend rien à ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie. Merci donc sur cet amendement du gouvernement qui a un monsieur qui venu. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Bon effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale. Le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à ce que il y est. Le développement de l'actionnariat salarié qu'il aussi des notions de partage de la valeur et c'est vrai que le, les propositions du rapporteur nous semblait empreinte de bon sens, compte tenu de la discussion qui vient d'évoquer le groupe va s'abstenir. Merci donc sur cet amendement du gouvernement qui a reçu un avis de sagesse de la commission et pour lequel il y a une demande de scrutin public. Nous allons procéder au scrutin public. Qui, à cet instant est ouvert. Voilà.

Tout le monde a voté. Le scrutin est donc clos. Alors votants 343 exprimés, 209 pour 183 contre 26. Le Sénat a donc adopté. Nous avons maintenant hein n'amendement. Ah pardon j'ai failli zapper le vote sur l'article. Article de. Demande de scrutin public également. On va le faire.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin est donc clos. Votants 343 exprimés, 315 pour 216 francs 99 le. Sénat. Adopter. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 18. Monsieur Montaugé. Si madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, quels que soient les les bords où nous siégeons dans cet hémicycle. Nous en appelons au renforcement de notre souveraineté nationale. Au sens 1er du terme. Il s'agit de doter o souveraine donc à à notre peuple la possibilité par le vote de ses représentants, de décider des questions et sujets qui engagent la vie de la nation. Depuis près de 80 ans, EDF a été au coeur de la performance économique de la France. Nous devons à cette entreprise et aux générations de salariés qui se sont succédé une part importante de la compétitivité de notre industrie et plus largement de notre économie. C'est encore vrai aujourd'hui. Malgré les difficultés provoquées qui ont été évoqués par la mise en place du marché européen, donc beaucoup de consommateurs, quel que soit leur taille peinait à voir les effets positifs, induits EDF pour les activités de coeur de métier. Cet amendement doit être un levier fort d'amélioration de la compétitivité nationale dans le contexte de transition énergétique et climatique que nous devons collectivement réussir. C'est pour cela que le Parlement aussi doit être saisie de tout sujet de réorganisation concernant EDF. Cet amendement. Quel est l'avis de la commission. Voilà. La commission est défavorable. Madame la présidente, pourquoi parce que il n'appartient pas au législateur de diriger au quotidien une société nationale une société nationalisée un épique. Chacun fait son métier et le parlementaire contre le gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement. Même avis, Monsieur le Ministre. Voilà et par scrutin public sur cet amendement double avis défavorable. On va le voter pour avoir procédé au scrutin public. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin votants 343 exprimés, 339% contre 239, le Sénat n'a pas adopté l'amendement numéro 4 de Monsieur Lurel. C'est vous qui le présenter. Il s'agit de rétablir dans son texte original originel. La. La l'évaluation donc le rachat de l'entreprise EDF. Un peu à l'instar de ce qui avait été fait en 46 par une. Instance. Commission administrative nationale. D'évaluation. Présidée par. Des fonctionnaires indépendants. Nous pensons-nous, que l'offre publique d'achat simplifiée. N'aboutira pas, contrairement à ce que moi j'ai pu entendre ici il y a quelques certitudes, comme si nous maîtrisions. Les délais judiciaires. De la cour d'appel de de Paris et du Conseil d'État mais moi j'en suis pas sûr. D'autant plus qu'il y a des possibilités de recours ultime d'appel de cassation. Ce n'est pas évident. Donc on a une loi de nationalisation. Qui est peut être une aubaine pour le gouvernement à à parer au plus mauvais au plus pressé. Au cas où. Et donc, nous vous demandons. De voter cet amendement. Pour rétablir le principe d'une nationalisation d'EDF. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Ici on n'est pas favorable puisque l'article 1er été supprimé. L'avis du gouvernement, mais ma vie. Monsieur le Ministre. Monsieur. Vous voulez une explication de vote je crois. Oui merci madame la présidente. Je suis peu intervenue sur les précédents mais je voulais quand même rappeler, je l'ai dit lors de la discussion générale que si EDF est dans la situation qui est la sienne, ça n'est pas parce que ça n'était pas une entreprise nationale c'est c'était par. C'est ça, on ne peut pas reprocher à l'entreprise privée EDF d'être dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui EDF et dans sa situation uniquement parce que la filière nucléaire a été malmené par des gouvernements socialistes sous l'influence de groupes écologistes et c'est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le nucléaire et dans la situation actuelle. Donc je pense qu'il faut quand même le rappeler. Il y a une prise de conscience qui est tout à fait salvatrice d'une très grande majorité des Français et même des groupes politiques qui qui forment la gauche aujourd'hui et qu'prennent conscience que si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Il faut une énergie décarbonée, et donc il faut relancer le nucléaire mais ça n'est pas. Parce que ça n'était pas une entreprise nationale que EDF se trouve dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Est ce qu'on pourrait imaginer que sur cet amendement de rétablissement de l'article 3. De la version initiale, on est le même vote que sur l'article sur les amendements de rétablissement de l'article hein. Ce qui nous épargnerait scrutin public qui a été demandé et donc on considérait que le Sénat n'a pas à votre adopté l'amendement.

On a voté l'amendement de rétablissement. Il n'a pas été adopté. Donc il a pu l'article. Sur le mode de calcul et le deuxième pour le retour aux tarifs réglementés pour toutes les collectivités et les TPE-PME. Et le dernier, un amendement de repli pour les collectivités juste sur l'été. Hervé et la reine parce qu'il y a évidemment un lien de cause à effet. D'ailleurs je pense que il faudra regarder sur les 60 milliards d'endettement, ce qu'a réellement coûté la reine qui a été votée en en 2010 dans le cadre de la loi Nome. Et je ne crois pas que c'était un gouvernement socialiste. À l'époque. Non il y a une vraie question autour de la reine et pour répondre à tout à l'heure à l'interpellation de monsieur le rapporteur. C'est vrai qu'il y a des acteurs alternatifs qui produit. Mais sur les 90 aujourd'hui. Il y en a de véritables c'est Angie et Total énergies tout le reste sont des factures Rather et sont en réalité des suceurs de sang d'EDF. Permettez-moi le. Le dire comme ça, et donc si il n'y avait pas d'reine et si on suspendait la reine. Ces 88 acteurs alternatifs tomberez c'est comme ça et d'ailleurs pour vous dire, il n'y a pas que le groupe communiste Fabien Gay, qu'il ne demande j'ai vu que le rapporteur Monsieur Armand. Qui député Renaissance demande la suspension très rapide de la reine, vous voyez donc quand il y a des gens qui commencent à travailler sur la question. Ils se rendent compte de l'ineptie de ce système et ils ne demandent pas le rénover. Il demande à le suspendre et sur le retour au tarif réglementé, juste une question parce que les gens doivent savoir ça c'est que, aujourd'hui, plus il y a Darren moins il y a des traitements et donc c'est vrai que les acteurs alternatifs. Aujourd'hui, ils doivent aller se fournir pour 70% sur la reine à 40 euros et après en réalité sur le marché. Donc comme le prix à à à des, à dévisser cette année ils ont été des fois 200, 300 400, 500 euros le mégawattheure, avec un pic. Tout le monde connaît au mois d'août à 1200 mais en réalité aujourd'hui nous avons un problème, c'est que depuis 5 ans ce n'est pas l'empilement des coûts et le coût réel c'est que on prend en compte pour l'augmentation du tarif les qu'augmenter la partie du taux d'écrêtement. Pour les acteurs alternatifs qui doivent aller se fournir sur le marché et donc en réalité on ne paie plus avec le tarif le commenter le coût réel de l'énergie on paye en réalité aujourd'hui les dividendes des actionnaires des acteurs alternatifs. C'est ça la réalité et donc le tarif réglementé, il augmente non pas sur les cours réels mais sur cette part d'écrêtement et donc sur le Trading du marché, c'est ça la réalité depuis 5 ans et c'est pour ça que ça dévisse et c'est pour ça que le tarif réglementé, il a augmenté en réalité beaucoup ces 2 dernières années, mais bien avant. Depuis 2017, il ne cesse d'augmenter tous les six mois, donc il faut en revenir sur un tarif réglementé qui s'applique sur les coûts et il faut en finir avec la reine qui rackettent. D'un côté. EDF et qui rackettent aussi les usagers, c'est ça la réalité. Voilà je vous remercie et donc j'ai présenté les 3 ans en même temps. Merci bien. Monsieur le rapporteur, va donner son avis sur les trois en même temps. Madame la présidente. La commission n'est pas favorable. Ces trois amendements parce qu'ils sont en, en opposition avec ce que nous avons établi. D'accord. Accords gouvernementaux transposée en droit français et en particulier dans le code de l'énergie sur la capacité d'ouvrir les terres VE. À l'ensemble des consommateurs sont justiciables de des TRV eux les résidentiel c'est-à-dire les particuliers et les professionnels dès lors des professionnels dès lors qu'ils ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Alors on a envie d'aider tout le monde sauf que c'est assez coûteux. J'ai cru comprendre. Et d'autre part, alors ça c'est un 1er problème nous serions en contradiction avec les règles européennes. Ensuite on, on, en effet, on irait subventionné on on irait casser des contrats qui sont établis actuellement entre des des entreprises et des fournisseurs alternatifs privés. Qui serait fondé à dire puisque la loi nous oblige à prendre en charge des TRV or EDF évidemment des TRV. D'alternatifs, à ce moment-là ils sont retournerait faire le gouvernement en disant puisque vous nous cassez des contrats où on gagne notre vie pour nous obliger à vendre moins cher, on suit, on va voir ce que veut dire, moins cher. Rembourser nous alors là ça coûterait bonbon et puis 3ème remarque le. Le TRV est calculé par la creux par un empilement et par un jeu assez complexe en effet de lissage dans le temps. Et nous ne pourrions avoir ces prix que dans une. Dans une perspective assez longue que madame Lavarde qui connaît mieux le sujet que moi pourrait expliquer il faut. Un recul. D'environ 12 mois je crois, pour pouvoir établir des TRV nouveau donc on est dans un système qui est à peu près non praticables et c'est la raison pour laquelle je vous propose de se borner à limiter. Au 36 E qu'avait à faire à supprimer les 36 qui avait, dans le cadre de l'Europe. Monsieur le Ministre, votre avis sur ces trois amendements. à tous les consommateurs. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'en avez arrêté mais il reste pour nous un aviez à cavalier totale à cette proposition de loi et sans rapport si je puis m'exprimer ainsi, avec le schmilblick. Cela dit, il est là aujourd'hui il vous êtes arrivé comme telles. Il faut donc on en discute et c'est vrai que vous avait limité son coût. En en limitant l'effet aux TPE en disant voilà c'est les TPE. Toutes les TPE, qu'elle soit. En fait consommatrices. Individuel comme vous et moi ou qu'elle soit consommatrices intensif comme certaines boulanger dont on a beaucoup parlé j'en comprends j'en c'est moins coûteux. Évidemment que ce qu'avait voté l'Assemblée. Alors c'est vrai qu'il y a de l'incertitude sur le coup. Tout simplement parce que ce type de dispositif il est exposé au marché et que son coût varie toutes les semaines en fonction du prix de marché. C'est d'ailleurs un de ces dangers. C'est que vous exposez alors soit les finances d'EDF au choix. Six EDF qui paye, soit les finances de l'État. A un coût de marché qui, lui, on l'a vu, depuis un an, un an et demi est extrêmement volatile. Et donc en décidant. De supprimer le plafond du TRV alors soit pour toutes les entreprises de l'ordre de 20 milliards, j'avais 10 18 et pourquoi j'avais des 18 à l'époque parce que l'écart entre le prix de marché. Quand j'étais à l'Assemblée nationale et l'écart du TRV étaient de l'ordre de 200 euros le mégawatt pour une consommation de l'ensemble des entreprises concernées par l'amendement brins de l'ordre de 100 térawatts, donc on arrivait à 20 milliards 18 pour être précis. Aujourd'hui votre amendement et coûte moins cher pour 2 raisons, d'abord parce que vous en limiter l'impact. on est sur une consommation de l'de 20 térawatts et puis l'écart a lui aussi baissé, parce que le prix de marché a baissé donc aujourd'hui votre amendement il coûte à peu près un milliard d'euros, 50 euros d'écart entre le TRV. Le prix de marché pour à peu près 20 TWh mais si demain ou après-demain. Le prix de marché explose et ben il coûtera 2 3 4 5 6 7 milliards d'euros et il faudra qu'on en assume les conséquences, soit directement sur les comptes d'EDF, dont on souhaite aujourd'hui tous, qu'ils soient préservés, soit sur les comptes de l'État dont on reconnaîtra tous je pense qu'ils sont quand même pas dans un état fantastique. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été le gouvernement était défavorable à l'ensemble de cette généralisation du TRV

entre 50 et 80 milliards d'euros sur le bouclier tarifaire. On a aujourd'hui beaucoup aider les ménages beaucoup aider les entreprises, y compris les énergies intensive. On va continuer à le faire, je préfère qu'on le fasse dans le cadre actuel que dans le cas de cet article, merci. Merci Monsieur Lurel pour une explication de vote.

C'était bien il me semble. De ta couleur politique. Donc que ce soit partagé, on le sait bien. Et que EDF aujourd'hui des problèmes et depuis toujours, il faut revoir le système lui-même et en particulier les marchés électriques en Europe, il faut avoir le courage de dire, ici et ailleurs que dans la stratégie qui a été adopté, contrairement à ce qui a été fait depuis 46 ans 74 par Messmer, aujourd'hui on est tributaire, est soumis à l'Allemagne. Il a d'autres concurrents, il faut le dire, l'Avantage que nous avions en nucléaire profite à d'autres et on, on n'ose pas le dire. On vient de perdre un combat taxonomie on vient ne dit que les réacteurs classiques ne seront pas intégrés et ne recevront pas un subventionnement public alors que c'était un combat homérique. Eh bien aujourd'hui, c'est un combat d'arrière-garde que nous conduisons et c'est la raison pour laquelle faire de dire une entreprise nationale intégrée vertical. Public et unifié était une urgence mobilisatrice pour les Français que nous sommes. Si la parole est maintenant à monsieur sont. Monsieur le Ministre, je, je profite de, de votre intervention. Ce que j'ai bien entendu et je veux je veux bien me faire confirmer ce que vous avez évoqués sur TRV tarifs de marché et la grande fluctuation, vous avez évoqué les boulangers mais il y a malheureusement pas que. je pense qu'il est important d'envoyer un message. Au public concerné puisque un certain nombre de fournisseurs à l'Automne dernier. Honte écrit alors abonné en disant écoutez, on ne peut plus tenir les tarifs. qui nous lier de manière contractuelle. Envolée des prix. Ça a été multiplié parfois par 5 6 7 8. Et puis aujourd'hui donc à ce moment-là, il aurait été proposé de signer de nouveaux contrats parfois. Contrat triennal. Dont aujourd'hui l'opérateur dit lui-même ah mais maintenant je ne peux plus y toucher. Je le dis parce que comme il se trouve que ce fournisseur à 3 lettres dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il va y avoir besoin d'une chose on clarifie la situation d'abord, l'État aura la main. Et à défaut vous l'avez dit, soit l'opérateur, le le le fournisseur. Revoit ses conditions. On nous dit que c'est pas possible j'entends soit l'État viendra en compensation mais il faut le dire. Aujourd'hui. Parce que derrière il y a des entreprises, vous le savez et je pense que l'État un message envoyé pour garantir un traitement je dirais équitable des situations

Merci madame la présidente. Je voudrais juste. Informé que de deux amendements ont été. Déclarées irrecevables au titre de l'article. 45 relatifs à la reine, nous c'est nous étions et nous pensons qu'il est souhaitable de limiter le volume de la reine à San TWh d'une part et d'autre part, de permettre le passage de 42 euros à 49,5 euros. EDF a besoin de ressources financières pour faire face à ses besoins d'investissement en particulier. Et depuis la loi d'août 2022. Et là l'avis du Conseil d'État sur la nécessité ou pas de notifier cette évolution de prix à à l'Union européenne. il est possible de, de procéder à cette à cette révision. C'est absolument nécessaire et il aurait été intéressant de savoir quand le le gouvernement. Va va procéder à à ceux-là. En théorie c'était possible depuis le 1er janvier 2023. Je vous remercie on a besoin d'une filière nucléaire brillante qui permettent même de CD de l'électricité à nos voisins et là-dessus. Nous sommes en accord. Je voulais revenir sur ces trois amendements et plus globalement sur l'article 3 bis évidemment. On ne peut qu'être favorable dans le principe. À l'extension. du tarif réglementé. C'est difficile d'être contre, cependant. D'un autre côté. Faut quand même aussi être responsable. Particulièrement pour les membres de la commission des finances. C'est quand même de l'argent public, évidemment on peut étendre à tout le monde. Le tarif réglementé. Nous y sommes tous favorables mais derrière, ce sont les finances publiques qui sont mises en cause et donc je voudrais formuler 3 remarque à ce stade certaines que j'ai déjà formulées lors de la commission des finances. La première, et le le ministre vient de le dire. Cet. Cet article 3 bis ne figurait pas dans le texte initial. Alors les auteurs font ce qu'ils veulent. Il n'en reste pas moins que ça ressemble fortement à un cavalier législatif, qui n'avait rien à voir avec le texte initial relatif à la nationalisation d'EDF 2ème remarque. là-dessus. Nous avons déjà eu des échanges en commission de finances avec le président de la commission des finances. Il est incontestable que quel que soit le payeur et le ministre-vient de le dire. Au final, c'est le contribuable qui paiera. Et donc, incontestablement, même si pour des raisons de procédure, on peut plaider le contraire. Incontestablement, cet article aurait dû. Être frappés de l'article 40. Et et il aurait dû être jugé irrecevable irrecevable de façon incontestable puisqu'il grève nécessairement les finances publiques et ma troisième remarque découle des 2 premières cet article 3 bis n'a rien à faire ici, ils devraient plutôt s'intégrer dans un PLF afin que nous puissions avoir une étude d'impact sérieux sur le coût de cette mesure. Monsieur. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on est d'accord que les tarifs réglementés. Ça a existé pendant 50 ans. Pour tout le monde. Résidentiels, entreprises, collectivités. Tout le monde y avait accès. Ça marchait plutôt bien hein. J'ai jamais vu personne s'en plaint dans à l'époque. Premièrement 2ème chose monsieur le rapporteur, j'ai déjà répondu nous dit c'est les règles européennes. Oui mais et tout le monde dirait déroge. Tout le monde demande des dérogations, pourquoi nous, nous ne demandons pas une dérogation pour protéger nos collectivités et nos petites entreprises en leur permettant le tarif réglementé par leur imposant aussi à des collectivités, des entreprises qui souhaitent rester dans des contrats a marché libre tant mieux pour elle mais celles qui voient leur facture exploser. On est tous élus de départements. Vous citez les commerçants les boulangers des collectivités et on est qu'au début de la crise hein ça va encore durer 2 ans et demi hein. Les factures vont continuer à pleuvoir. 3ème problème, c'est le ministre et où il va falloir qu'il est quand même à un moment donné quelqu'un parle au 30 juin. 5 millions de personnes n'auront plus accès aux tarifs réglementés du gaz. Les particuliers en pleine crise du gaz, est ce que nous allons laisser faire cette chose ou pas. Est-ce que nous nous allons quand même prendre une initiative ou parlementaire ou gouvernementale pour les prolonger en pleine crise ou est-ce qu'on va toutes et tous les laisser s'enfoncer. Sur le prix du marché. Il faudra répondre. Et puis dernière chose, monsieur le ministre. Vous dites ça coûte cher, certes. Quand on a proposé le retour aux tarifs réglementés pour toutes les collectivités ont on départ, on nous a dit 60 milliards, et puis quand il y a une étude 3 milliards et demi. 3 milliards et demi et vous l'avez dit combien. Bouclier. Tarifaire sécurité filet de sécurité à Rennes supplémentaires rien que l'an dernier avec des trous dans la raquette, 50 à 80 milliards, donc 3 milliards et demi pour le retour au tarif réglementé et 50 à 80 milliards que vous avez jeté à la poubelle et donner aux acteurs alternatifs. Voilà la réalité.

Auraient leur place dans un PLF très très volontiers, mais je voulais en profiter aussi pour répondre à mon collègue kaput. Qui nous prête beaucoup de pouvoir et je le remercie, c'est vrai que 50 milliards de grand carénage, 56 milliards pour six EPR dans l'estimation gouvernementale, parce que quand même le père, un coup de 19 milliards mais on va en faire six pour 56 milliards et 64 milliards de dette, c'est aussi un tout petit peu d'argent, donc 3 milliards pour les tarifs réglementés de vente, ça me paraît tout à fait acceptable. Monsieur le Ministre. dans les discussions au sein de la commission des finances, ni celle de l'Assemblée nationale ni celle évidemment du Sénat. Pourrait éventuellement se réserver se réserver le droit de de de de porter cette controverse devant le Conseil constitutionnel. On verra. vous mais vous m'excuser si je vous réponds pas sur le gaz on passe déjà pas mal de temps sur l'électricité aujourd'hui, vous aurez quand même l'occasion de discuter dans le cas de la programmation pluriannuelle de l'énergie de toutes ces discussions importantes sur la manière dont on doit envisager envisager la fourniture d'électricité, de gaz et plus généralement d'énergie en France pour les années qui viennent et vous l'aurez en temps voulu. Juste quelques chiffres qui vont permettre j'espère à la fois de préciser la question du du rapporteur général Husson et et les questions que vous avez mentionné en passant sur le coup d'de différents dispositifs quand même Bouclier tarifaire pour les particuliers plus TPE plus petites collectivités inférieures à 36. Kilovoltampères ce que vous proposez aujourd'hui d'élargir. Aux TPE, quelle qu'elle soit. Ça a limité à 15% la hausse des prix au lieu de 120% sur 2 ans, le coût pour les finances publiques, c'est 30 milliards en 2022 et 45 en 2023, y compris les collectivités territoriales dont vous parliez. Le cap à 280 euros le mégawatt. Ça c'est important. Monsieur le rapporteur général. Vous nous disiez qu'est-ce qui se passe si on n'est pas aujourd'hui couverts par le TRV. On a adopté d'ailleurs sur la suggestion d'un certain nombre d'entre vous, un cap à 280 euros le mégawatt. Pour le prix de l'électricité pour toutes les TPE qui, vous l'avez dit, ont eu la malchance d'avoir un contrat qui s'interrompaient à l'Automne dernier et qui se sont retrouvés du coup à négocier un peu le couteau sous la tente, des contrats qui était bien au-dessus de ce qu'ils avaient auparavant et donc c'est 280 euros le mégawatt sont intégrés en moyenne sur ta l'année dans les factures qui sont actuellement envoyés par les fournisseurs d'énergie, y compris pour un certain nombre de boulanger ou d'autres TPE concernées. On a aussi adopté un amortisseur électricité pour les PME. Et pour les collectivités territoriales. Alors ça c'est un peu plus compliqué mais c'est cohérent avec la réglementation européenne qui fait qu'on prend en charge 50% du surcoût au-delà de 180 euros le mégawatt. Et ça ça coûte entre 2 et 3 milliards d'euros à la collectivité nationale et enfin pour les ce qu'on appelle les énarques intensif donc et pour les plus grandes entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Un guichet qui permet aujourd'hui à un certain nombre d'entreprises de faire valoir la hausse de leurs coûts de la facture d'électricité ou de gaz et de demander des aides qui à ce stade correspondent à 250 millions d'euros attribués depuis quelques semaines et sans doute une accélération assez forte puisqu'on voit l'accélération importante depuis 10 jours avec les factures de 2023 qui arrive, on a ajouté à votre d'ailleurs suggestion un filet de sécurité de 430 millions d'euros adopté elle été 22 pour les collectivités. Dans le cas de la loi de financement rectificatif. Bref, tout ça, ça nous coûte beaucoup d'argent, on peut en être fier parce qu'au fond, l'inflation en France est inférieur. Ailleurs en Europe, et les entreprises ont plutôt bien passé la crise, contrairement à nos craintes. Mais soyons conscients quand même que tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Merci. Est ce que on pourrait dire que sur ces trois amendements. Le vote est le même que sur l'amendement 14 de monsieur Voilà et que donc ils ne sont pas adoptés. Sur l'article 3 bis. Il n'y a pas de demande de scrutin public donc il est pour. Vous votez l'article avant que je vous passe la parole pour le 15.

Monsieur l'amendement 15 pardon. Merci. Oui c'est c'est une demande de rapport je sais que le Sénat n'en n'en est pas fan sur le coût du bouclier tarifaire. Bon vous venez nous répondre nous donner. Des des premiers chiffres. beaucoup beaucoup d'argent, on a du mal à d'ailleurs à avoir. À avoir les chiffres exacts. Est ce que vous pouvez nous confirmer que ça a coûté 20 milliards en 2022 et 37 milliards prévus en 2023 et juste pour que les gens comprennent. Ça veut dire quoi. Le bouclier tarifaire. enfin l'État indemnise les acteurs alternatifs en leur donnant de l'argent public pour appliquer le bouclier tarifaire par exemple ce que vous venez dire sur les. Sur les boulangers. Il avait un contrat à 40 ou 50 euros le mégawattheure.

ensemble que les présidents de groupe et le président de la commission des finances peuvent cesser de bouillonner tous les deux, voilà pourquoi monsieur Guelfi Ministre d'intervention. Je finis juste ça

Donc le ministre de l'Économie a réuni les énergéticiens et leur a dit maintenant le contrat ne doit pas dépasser 280 euros le mégawattheure. Sauf que ces énergéticiens déjà y'pour plus de 70% de l'énergie qu'ils vous revendent il achète au prix de 40 euros. Donc il y a que les 30 derniers %, même si même si l'acheter. Imaginons à 900 euros le mégawattheure. Les 30 derniers pour 100. Même à 280 euros il ferait déjà des bénéfices, et ça suffit pas. Qu'est ce que fait le gouvernement, il donne de l'argent public aux. Acteurs alternatifs pour appuyer qu'est ce bouclier tarifaire pour en quelque sorte l'indemniser. C'est-à-dire que le boulanger comme n'importe quel commerçant comme n'importe quel chef d'entreprise comme n'importe quel usager il Irak était 2 fois d'abord par l'augmentation de sa facture électrique et en même temps en tant que contribuable, parce qu'il participe à donner de l'argent aux énergéticiens. C'est un pur scandale et l'affaire donc a coûté près de 50 milliards d'euros en 2 ans et il faut le dénoncer, je vous remercie. Eh bien, la commission, madame la présidente, mes chers collègues, n'est n'est pas favorable à cet amendement et pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il s'agit bien d'une étude d'un d'un rapport que vous demandez au gouvernement. Eh bien nous, nous souhaitons faire notre rapport par nous nous-mêmes parce que c'est l'indépendance du Parlement qui s'exprime à travers le travail de ses rapporteurs. Il se trouve que la commission des finances et je salue son président a demandé au rapporteur spécial madame Christine Lavarde de présence de préparer un contrôle budgétaire sur cette affaire parce que il y a ceux qui perdent et il y a ceux qui gagnent. Et on aimerait savoir comment et combien ceux qui gagnent apporte en contribution à l'État vous la vie est évoqué dans les débats budgétaires parce qu'il se trouve que si le prix augmente, il y a des entreprises qui touche et qui touchent plus que d'habitude, sans nécessairement vous avez raison Monsieur Gay avoir dépensé pour autant. Nous avons des producteurs qui produisent de l'énergie renouvelable, tant mieux pour eux, c'est bien, c'est parfait ça tous les avantages, mais qui ne sont absolument pas tributaire du prix des de l'énergie fossile et qui empoche tranquillement car vous savez que alors je je reviens pas sur les démembrements puis je vais dépasser encore longtemps mais enfin l'appel. Sur un appel est prioritaire aux énergies renouvelables. Donc ils vendent leur mégawatts à un prix qui est simplement délirant et je je pense qu'ils doivent en restituer et c'est la raison pour laquelle la commission des finances a confié à madame Lavarde soin de d'évoquer ce sujet de la profonde. Je vous rappelle qu'on a un 2ème texte hein derrière. la toute la toute la liberté pour examiner tout ça et de la poser toutes les questions que vous souhaitez au gouvernement rappeler aussi aux sénateurs GEC. Sur la reine évidemment celui qui en bénéficie, c'est le consommateur. Ultime c'est pas le distributeur qui prend une marge très encadré et qui vend l'électricité au rabais au coût de production d'EDF et c'est pour que l'ensemble des consommateurs, y compris industrielles, j'y tiens puissent bénéficier des investissements de la nation depuis 77 ans pour bénéficier en France d'une électricité décarbonnée en volume et pas cher.

sur le fondement de l'article 44 bis ça rappellera des souvenirs à certains. Concernant le droit d'amendement des. Des parlementaires et des sénateurs, en l'occurrence et dans le cadre de la sincérité des débats. Je voulais vous soumettre une modification de notre vote sur l'article 3 bis. Donc il y a une incompréhension et le groupe socialiste souhaite voter l'article 3 bis dans le cadre du vote précédent. Je ne sais pas si cela est possible techniquement. À ce stade, acte de votre mise au point et. Comme c'était un vote à main levée. Donc c'est pour. La liste de ceux qui sont là. Dimanche quoi. On peut pas revoté on finit les amendements ont et puis après on verra.

C'est une demande de rapport qui a eu la sagesse de la commission un peu mieux rédigé que ce qui avait été soumis et qu'on vous demande d'agréer. Quel est l'avis de la commission. La Commission avait en effet émis un avis de sagesse. La rédaction Nouvelles. Bon un peu particulière parce que elle pose le principe. L'intérêt de nationaliser. Ça c'est le 1er volet du rapport et un simultanément un calendrier des étapes de mise en oeuvre. Ça veut dire qu'en fait, le jugement est donnée avant même que le l'étude soit engagée. C'est un peu contradictoire. Moi je suis gênée par le la référence au calendrier aux étapes parce que ça ça suppose le problème résolu et donc. Si tu sais manche. Moi je suis je suis pas favorable à cette rédaction. Je ne peux pas parler au nom de la commission, sauf à la réunir.

C'est un avis défavorable. Non, non pas parce que nous sommes contre les rapports nous adorons les les produire comme vous le savez, cette disposition n'a pas de rapport avec la nationalisation d'EDF et de Électricité de Mayotte, vous le savez est un opérateur distinct, qui n'a qu'une participation, EDF n'a qu'une participation minoritaire, moins de 25%, l'actionnaire majoritaire étant le département de Mayotte. Très bien. Il y a une demande de scrutin peu de Oui merci madame la présidente. Alors le, le rapporteur a tout à fait raison. Cette nouvelle rédaction est un peu problématique mais surtout je voudrais demander aux auteurs de l'amendement, pourquoi ils se sont intéressés à l'ex-Christine Mayotte comme vient de le rappeler justement le ministre on est quand même dans un actionnariat qui est déjà largement public puisque 50%. De si le département de Mayotte. Mais pourquoi ce qu'Électricité de Mayotte. Pourquoi vous êtes pas intéressé à ce moment-là aux entreprises locales de distribution enfin accessoirement elles font sur une partie du territoire national. Ce que fait aussi EDF et alors pour vous dire Électricité de Strasbourg est détenu à 88,64% par EDF, développement et environnement et à 11,36% par d'autres actionnaires qu'allez-vous faire de. UEM à Metz qui est détenu à 85% par la ville de Metz à 15% par la Caisse des dépôts, je vais vous épargner la liste de toutes les électrices enfin des entreprises locales de distribution mais j'avoue que ce voit pourquoi Mayotte arrive là comme ça en plus avec une nouvelle rédaction qui est. Un peu abscons. Donc on nous avons un avis défavorable.

On va donc considérer que sur l'amendement numéro 5 même votre que sur. Alors on va le scrutin public. Ah non oui scrutin public sur celui-là monsieur Duret vous voulez prendre la parole pour. Je pas bien entendu madame la présidente. Pourquoi on s'est intéressé à Mayotte, parce qu'on est dans une zone monétaire. Deuxièmement cette. J'allais presque d'une continuité historique en 1975. Le président Valéry Giscard d'Estaing. Avec la même structuration du capital à nationalisé la speed. En Guadeloupe, l'aspect des Martinique à la Réunion et en Guyane, aujourd'hui à la même structure à Mayotte avec des difficultés, on a un monopole EDF pour le transport dans les et demi, donc vous voyez c'est c'est c'est différent. Ensuite, il y avait une ambiguïté sur l'application des TRV Dans les outre-mer aujourd'hui, c'est réglé le compte de l'énergie et clair, je veux bien admettre que la nouvelle rédaction précise les modalités et que. Que on on on ne discute pas. C'est vrai du principe de la nationalisation. On admet qu'il faut nationaliser et qui fut le feu un calendrier. Voilà. Elle était l'amendement et qui avait reçu un avis de sagesse. Il y a donc je j'ouvre le scrutin public un scrutin public sur cet amendement, messieurs les huissiers. Donc il a reçu un double avis défavorable, le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter Le scrutin est clos. Votants 342 exprimés, 336% contre 236 E Sénat n'a pas adopté, je me vois l'article 3 ter, qui est pour.

Donc je recommence. Qui est pour l'article 3 terme ah bah voilà.

Qui est pour, je recommence pour alors. Un, deux, trois. C'est l'article 3 ter là qu'on est en train de voter. Monsieur Lurel et vous faites quoi avec vos mains. cinq, six. Huit, neuf, 10. 11 12 13 14 15 16. Il est adopté. Et l'article 4 est supprimé et je vais suspendre quelques instants la séance pour régler quelques petites questions évoquées tout à l'heure par le rappel au règlement du président. La séance

La séance est reprise. Je donne la parole au président rénale. Madame la présidente, je vous demande une minute de suspension pour que la commission se réunissent pour étudier un amendement de rétablissement et ensuite. Pouvoir faire une 2ème, délibération de l'article 3 bis l'application de l'article 43 alinéa 4 du règlement, et tout d'abord une minute de suspension pour que la commission se réunisse. Et me mandatent officiellement. La séance est suspendue pour une minute.

D'abord. La séance est reprise et en application de l'article 43 Je vous la donne d'abord président OK j'allais. Dire pourquoi vous le donnez. Malaisie. Merci madame la présidente. C'est juste pour vous donner le résultat de la commission. à la commission des finances demande donc une 2ème délibération sur l'article 3 bis en application d'Arte 43 dîner alinéa 4 du règlement, madame la présidente. Merci. Donc quel est l'avis du gouvernement, sur cette demande de délibération. la vie plutôt défavorable la première délibération lui semblait en fait. Plutôt pas mal. D'accord.

C'est juste que si vous êtes contre. Si vous êtes pas contre vous n'avez pas la parole il y a pas d'explication de vote. Est-ce que vous êtes contre. Je suis contre. Vous êtes contre la 2ème délibération. Et dans ce cas, vous faites le contre. Exactement, je fais l'opposition contre. Il me semblait comme l'a rappelé le ministre, que. Les auteurs de la proposition s'était rendu compte que c'était à la fois un cavalier que cet article 3 bis était un cavalier et qu'il était y'recevable. C'est la raison pour laquelle le président de la commission des finances s'était rendu compte et avait voté contre n'avaient pas voté cet article 3 bis. Ça me paraissait tout à fait logique donc cette seconde délibération ne me paraît totalement inopportune. C'est, je dirais même que c'est presque un passage en force. Madame la présidente, pour reprendre des arguments que nous avons eu par le passé. Si j'osais mais je n'irai pas jusque-là. Donc il me semble en revanche. Que sur le fond de cette seconde délibération elle elle ne s'impose d'autant pas d'autant moins que j'ai bien compris que la réécriture de l'article 3 bis par le rapporteur. Gérard Longuet et meilleure effectivement que l'écriture. Première. De de l'amendement de l'article de telle sorte qu'il est peut-être ça qui a un petit peu a induit en erreur. Nos collègues des rangs de la gauche, il n'en reste pas moins que sur l'argument développé par le rapporteur sur le fait que.

PME et l'effet de seuil existera toujours. On le décales uniquement. À aux plus grosses entreprises, mais il y aura toujours un effet de seuil sur cet article 3 bis. On est bien dans le sujet, c'est la raison pour laquelle. Madame le président. Il me semble effectivement que cette seconde délibération n'est pas opportune. nous bien entendu, que vous étiez contre mais. C'est en application de l'article 43 alinéa 4 que cette seconde délibération va être soumise au vote du Sénat c'est donc conforme au règlement. Donc qui est pour cette seconde délibération. qui s'abstient. La seconde délibération et donc et donc décidé, conformément à l'article 43 alinéa 5 mois. Lorsqu'il a dû à une seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération se renvoient la commission qui doit présenter un nouveau rapport, la commission a déposé un amendement de rétablissement de l'article 3 bis que vous avez, que nous avons là Je vous lis rédiger ainsi cet article. Oh il arrive. Monsieur le rapporteur, va vous le présenter. Monsieur le rapporteur. Vous pouvez présenter en, en un mot, Favorable à revenir au texte de la commission car ce qu'elle est l'avis du gouvernement. Les mêmes raisons, tout à l'heure que j'ai longuement exprimé défavorable. D'accord. Je vais donc mettre aux voix cet amendement.

pour laquelle je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin est donc clos. Votants 343 exprimés, 329 pour 206 heures contre 123, le Sénat a adopté. Et nous allons maintenant. Pour suivre l'ordre du jour avec la discussion de la proposition de loi constitutionnelle. Chez ce. 30 secondes. Pour la rotation des équipages.

Pardonnez-moi mais il faut laisser s'installer. La commission des lois. Nous poursuivons l'ordre du jour avec la proposition de loi constitutionnelle visant à créer une loi de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements et à garantir la compensation financière des transferts de compétence proposition doit présenté par monsieur Éric Kerrouche et plusieurs de ses collègues dans la discussion générale. La parole est d'abord à l'auteur de la proposition de loi Monsieur je lisais pardon et je ne vous regardez pas Monsieur le Président. Mais vous avez la parole pour un rappel au règlement. Un rappel au règlement, madame la présidente. Juste sur l'organisation de nos travaux enfin du groupe socialiste se termine à 20h est ce qu'on imagine. Réussir à faire tout parce que d'abord calcul ça fait 1h45. Il reste 1h10. il y a une 10 minutes de suspension. Et donc la prolongation prévu jusqu'à 20h 10. Monsieur le Président, vous allez me dire que ça change pas grand chose d'autre question. J'ai bien compris. Écoutez on va avancer. Monsieur

Que les objectifs fixés au sein d'une loi d'orientation pluriannuels soit décliné au sein d'une loi de financement ou de finances il permettrait en tout état de cause d'inscrire les débats sur la fiscalité locale dans une nécessaire. Pluriannualité. Si notre proposition de loi constitutionnelle a opté pour une loi de financement des collectivités nous souscrivons entièrement aux propos du rapporteur spécial de la mission budgétaire RCT du PLF 2020 Loïc Hervé, que je viens de reprendre. En fait. Notre proposition est une proposition qui est une preuve de ses propositions partagées par. Des acteurs d'origine. Et de viser différentes. L'Association des maires de France pour commencer qui l'a fait savoir par la voix de son précédent président François Baroin pour la révision constitutionnelle de 2018, réaffirmé dans la contribution à l'élection présidentielle de 2022 et plus récemment par son communiqué de presse du 14 mars 2023. Par aussi une grande partie des maires que nous avons interrogé en 2019 et qui nous ont dit à 80% qu'ils étaient d'accord avec cette possibilité par également la Cour des comptes dans ces rapports, 2013 2016 2018 par les rapporteurs, Charles de Courson et Christophe j'et. Qui ont abouti aux mêmes conclusions, en mai 2018 dans le cadre de leur mission flash sur l'autonomie financière des collectivités locales par notre collègue Roger Karoutchi qui a déposé un texte et une proposition de loi constitutionnelle dont le texte est quelque peu comparables aux nôtres. Le constat est donc partagé. Parce que. La révision constitutionnelle de 2003 n'a pas permis de garantir, vous le savez l'autonomie fiscale des collectivités locales pour se réduire à une autonomie financière interprétés de manière stricte par la jurisprudence du Conseil constitutionnel lors de la suppression de la taxe d'habitation notamment. Cette consécration de de de l'autonomie financière n'ayant été au final pour reprendre le professeur Michel Bouvier qu'un rendez-vous manqué est une illusion. Il en est de même de la jurisprudence dans l'appréciation des mécanismes de compensation financière des transferts de compétences. C'est particulièrement édifiant, vous le savez, en ce qui concerne les dépenses sociales de nos départements. Malgré de nombreuses QPC qui ont été soulevées par les collectivités, aucune n'a prospéré face à l'interprète tension strict de notre conseil constitutionnel. L'autonomie financière des collectivités a donc été vidé de son sens alors que il s'agit quand même de garantir la libre administration. Donc le respect de l'organisation décentralisée de notre République. La part de fiscalité s'est progressivement réduite au profitation au profit de dotation. Donnée par l'État. Les dernières dispositions budgétaires issu de la loi de finances de 2023 ont encore fait la démonstration de cette évolution avec la diminution de la CVAE. Nous nous retrouvons donc dans un système qui est de plus en plus opaques et illisible en octobre 2022, la Cour des comptes, souligné que je cite la sédimentation historique des recettes. Et a fait le constat que notre système était de plus en plus complexes et à bout de souffle. Ce système opaque illisible entravent l'action des collectivités locales qui n'ont pas de visibilité sur les réformes fiscales les décisions d'attribution des dotations d'investissement ou alors l'imposition des normes de toute nature. L'éparpillement des mesures budgétaires et fiscales concernant les collectivités locales dans la loi de finances ne fait qu'ajouter à la confusion qui s'est installée dans les relations financières entre l'État et nos collectivités ou l'État cherche souvent à faire payer. Aux collectivités justement ce qu'il ne souhaite plus assumer. notre proposition qui réside dans deux points, d'une part la création d'une loi de financement des collectivités territoriales d'autre part une compensation dynamique dans le temps des transferts opérés. S'agissant de la loi de financement des collectivités locales. Je rappelle que c'est quelque chose qui est historiquement. Ancrée. Avec le rapport d'Olivier Guichard de 1976 repris régulièrement notamment dans le rapport Lambert Malvy. Les objectifs de cette loi de financement sont simples. Un cadre de référence unique pour le Parlement, un outil de transparence pour une meilleure information des élus locaux. Une lisibilité et une visibilité pour les collectivités territoriales à même de conférer ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire de la prévisibilité. également désengagement financier de l'État et enfin une clarification des responsabilités de chacun. Ainsi la loi de finances articulé comme peut être le PLFSS. Le texte Le texte principal. Qui. Fait l'équilibre financier de l'État elle viendrait s'inscrire comme un complément et on ne nous aurions un trépied avec une loi de finances, une loi de De la sécurité sociale et une loi de financement des collectivités. Mais le texte a d'autres ambitions, d'abord la clarté et la sincérité des débats parlementaires en ce qui concerne. Les collectivités. La reconnaissance au sein de notre édifice constitutionnel des collectivités locales qui représentent 20%. Des dépenses du budget de la nation et 57% de l'investissement local. Cette évolution permettrait également de mettre fin à l'infantilisation constante des collectivités territoriales par l'État et elle constituerait cette loi un espace de dialogue justement entre ces mêmes collectivités et l'État central. Certains arguments nous ont été objecté par la rapporteure des écueils pratique au regard du calendrier parlementaire. Il y aurait déjà matière à discuter du calendrier d'examen de la loi de finances qui mériterait tout simplement d'être revu. Problèmes d'articulation avec la loi de finances mais. La loi de finances initiale retrace les versements de l'État à la sécurité sociale, ce qui n'empêche pas le vote par le Parlement d'une loi de finances de la Sécurité sociale. On nous a parlé aussi d'un pouvoir de contrainte supplémentaire pour le gouvernement et en fait. C'est déjà le cas, les atteintes à la libre administration sont légion gel diminution des dotations contrat de Cahors. Nous pensons plutôt que c'est le manque de transparence qui menace l'autonomie il ne s'agit pas ici de faire un parallèle entre cette loi de financement des collectivités territoriales et la loi de financement de la Sécurité sociale puisque au nom de la libre administration des collectivités. Il ne s'agit pas de fixer un plafond et et et de lui donner un caractère prescriptif. Autre argument, l'utilisation possible du 49.3, je ne vois vraiment pas la différence avec la situation qui existe déjà le 49.3 pouvant être utilisées et il a été largement sur la loi de finances. L'absence de loi organique enfin qui empêcherait de se prononcer. Nous sommes prêts à y travailler avec vous madame la rapporteure notamment. En déclinaison de la PPL de notre collègue Karoutchi que vous avez cosigné. S'agissant de la garantie dynamique. L'article de notre texte prévoit une garantie effectivement dynamique dans le temps du transfert de compétences. Là aussi je ne vais pas épiloguer. C'est une demande réitérée demande réitérée des collectivités territoriales, cette disposition avait été intégrée lors de l'examen du projet de loi 3DS à notre initiative, et malheureusement retiré en CMP. c'est vrai que. Le président Philippe Bas avait également intégrer cette disposition au sein de sa PLC qui a été votée mais cela ne suffit pas à retirer l'intérêt de ce que nous proposons. Ce texte vise surtout à réaffirmer le le rôle que jouent les collectivités locales dans l'organisation décentralisée de la République. Cette reconnaissance est pour nous impérative et elle ne peut pas, elle ne devrait pas être sacrifié sur l'autel de la politique partisane. D'où la proposition que nous faisons aujourd'hui de travailler ensemble, comme nous avons pu le faire pour Lausanne. Il est temps pour conclure de sortir de la verticalité du pouvoir qui place l'État et les collectivités locales dans un rapport de défiance permanent cette loi permettrait une nouvelle avancée des libertés et de la démocratie locale. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur de la commission des finances pour avis, il y a 40 ans, les lois de faire instaurer la décentralisation. 20 ans plus tard, ce nouveau principe d'organisation de la République était gravé dans le marbre de la Constitution. Les fondements constitutionnels de la décentralisation sont nombreux et consacrent notamment de principe. D'une part la libre administration des collectivités territoriales et d'autre part leur autonomie financière. Les 2 sont liés, car sans autonomie financière. Pas de réelle marge de manoeuvre aujourd'hui nous partageons un constat avec les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle dont nous débattons l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales est insuffisante alors que nous traversons une crise inflationniste énergétique s'interroger sur le niveau et la présider prévisibilité pardon des ressources des collectivités territoriales. N'est ni un gadget ni une lubie de parlementaires. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces sujets ne serait-ce que pour éviter que l'investissement local ne fléchissent alors qu'ils représentent une part déterminante de l'investissement public. Aussi les auditions menées dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi constitutionnelle, ont souligné. D'une part l'amoindrissement des marges de manoeuvre fiscale et financière des collectivités territoriales. Du côté des recettes du fait de la suppression de la taxe d'habitation et de la CVAE. Du côté des dépenses avec l'introduction des contrats de Cahors ensuite le défaut de prévisibilité suffisante des élus locaux sur leurs ressources en raison d'une absence de programmation budgétaire pluriannuelle puis l'insuffisante lisibilité des élus sur les décisions financières et l'attribution des dotations l'enchevêtre ment des réformes successives ont opacifiés. Les modalités d'attribution des dotations pour les collectivités territoriales le défaut également d'information des collectivités territoriales en amont des projets de loi de finances et lors des décisions d'attribution des dotations ont été largement souligné. l'émiettement des mesures budgétaires et fiscales ayant un impact sur les ressources comme les dépenses des collectivités territoriales dans le projet de loi de finances nuisant à une appréhension globale des relations financières entre l'État et les collectivités. C'est pourquoi, mes chers collègues, je crois que nous sommes aujourd'hui, tous d'accord sur à la fois la nécessité de remédier à la situation actuelle des collectivités territoriales qui ont vu leur marge de manoeuvre se réduire et l'urgence de corriger les nombreux défauts du cadre législatif et constitutionnel actuel des finances locales pour les collectivités territoriales. Face à l'absence de garanties réelles de l'autonomie officiait finance. Sierre et fiscales des collectivités territoriales. La proposition de loi déposée par notre collègue Éric Kerrouche propose de solutions d'inégale portée d'une part la création d'une loi de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. D'une part la rénovation des modalités de compensation financière des transferts de compétences pour mieux appliquer le principe qui décide. P. Je ne peux que partager pleinement l'objectif recherché par cette proposition de loi qui s'attend qui s'attache à répondre aux attentes légitimes des élus locaux. Toutefois, il semble que les mesures proposées présente un certain nombre de difficultés opérationnelles et juridiques n'apportant aucune réponse imparfaite au souhait de lisibilité et de prévisibilité des élus locaux sur leurs ressources financières. En première lieu 1er plusieurs des personnes auditionnées et en particulier l'ensemble de la, des associations, des élus locaux se sont. Interrogé sur l'utilité de la création d'une loi de financement spécifique aux collectivités territoriales et à le regroupement pour atteindre cet objectif. Ainsi les associations des locaux ont rappelé que l'institution d'une telle loi ne figurait pas parmi leurs demandes et que d'autres mesures leur semblait répondre davantage à leur attente. En 2ème lieu une telle loi de financement n'empêcherait pas une révision annuelle du montant des concours financiers de l'État aux collectivités, conformément au principe d'annualité budgétaire. Dès lors, il ne serait pas certain que l'inscription dans la constitution d'un véhicule financier spécifique aux collectivités territoriales et à leurs groupements aurait une incidence majeure sur l'autonomie financière de celle-ci ou sur la prévisibilité de leurs ressources en troisième le et de l'avis quasi unanime des personnes entendues élus locaux comme professeur de droit ou de finances locales un tel véhicule. Révèle le risque de confier au gouvernement un nouvel outil procédural lui permettant d'imposer unilatéralement aux collectivités territoriales et à leurs groupements de nouvelles réductions de leurs marges de manoeuvre financières comme tout véhicule financier le gouvernement serait libre de faire usage des facultés prévu à l'alinéa 3 de l'article 49 ou d'autres d'opter par voie d'ordonnance. Les mesures proposées. Si le Parlement ne respectait pas les délais d'examen un parti. En 4ème lieu, ces dispositions se heurte à de nombreux écueils juridiques est parti est pratique. En particulier la difficulté d'isoler dans les finances publiques, les ressources des collectivités territoriales de celle de l'État, de la même manière, il serait nécessaire de tirer les conséquences de toute loi de financement sur les recettes et les charges de l'État dans la loi de finances. Ceux qui s'en de facto en relativiser l'intérêt. Enfin l'insertion d'un nouveau texte financier dans le calendrier parlementaire déjà très chargé est un point de vigilance qui peut sembler anecdotique mais doit être soulevée en cinquième le ce sujet me semble être le plus irritant entre nous. La proposition de loi constitutionnelle disent les collectivités territoriales et le regroupement, or aujourd'hui les groupements émanation des communes ne bénéficie pas en matière financière des mêmes garanties que les collectivités territoriales, car ils n'en sont tout simplement pas. Dès lors, ces dispositions modifierait les équilibres constitutionnels et institutionnels existants au sein du bloc local et reviendrait à accorder au groupement des garanties applicables aujourd'hui seulement aux collectivités territoriales. Enfin s'agissant des dispositions relatives au réexamen régulier des compensations financières de transfert et de compétences et une amélioration des modalités de compensation à l'article de. Je ne peux qu'être favorable à ce principe, elles sont là. La tradition constitutionnelle. D'un principe cher à la présidente de la délégation aux collectivités territoriales qui décide. P. Néanmoins je tiens à rappeler que les principales dispositions de cet article ont déjà été adopté par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale qui est libre de les inscrire à son ordre du jour. En outre, la proposition de loi ambitionne détendre ces garanties financières regroupement et dès lors, par cohérence avec la position constante de notre commission sur ce point je ne pour y être que défavorable. Ah si cher collègue. Si cette proposition de loi pose un débat essentiel, celui de l'équilibre à trouver en matière d'autonomie financière comme fiscale des collectivités territoriales au sein d'un état unitaire et décentralisé les solutions qu'elle y apporte m'apparaissent imparfaite et insuffisante pour répondre à l'enjeu soulevé d'autant plus que le sujet a déjà été largement exploré par la proposition de loi de notre collègue Philippe Bas. C'est pourquoi je vous propose de ne pas adopter cette proposition. Pour terminer, j'ajouterais qu'il m'apparaît préférable de traiter ces sujets dans le cas d'une réflexion plus large sur la place des collectivités territoriales dans l'architecture institutionnelle actuelle. Cette réflexion est pour l'heure, porté par le groupe de travail transpartisan sur la décentralisation. Initiée par le président du Sénat et dont notre président de la commission des Lois François-Noël Buffet et le rapporteur général. Dans ce cas nous avons discuté déjà la semaine dernière à l'initiative du rapporteur général du budget de la commission des finances Jean-François Husson de propositions couvrant l'ensemble du Champ des finances locales. Dans ces conditions, je forme le voeu que nous continuerons à cheminer ensemble pour redéfinir les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, convaincu que l'autonomie financière des collectivités territoriales est une condition indispensable à l'effectivité de la décentralisation en l'espèce, je vous invite donc à ne pas adopter cette proposition de loi constitutionnelle.

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les présidents des commissions des lois et des finances. Madame le rapporteur, chers collègues. Bien qu'une majorité de ses membres se soit prononcée contre l'adoption de la proposition de loi constitutionnelle déposée par Éric Kerrouche et plusieurs de nos collègues. La commission des finances partage le diagnostic qui a conduit à son dépôt. Le manque de prévisibilité budgétaire qui frappe les collectivités territoriales, d'une part et la sous-évaluation de plus en plus manifeste des compensations de compétences. D'autre part constitue malheureusement de réalité à première vue l'instauration d'un éventuel projet de loi de financement des collectivités territoriales paraît séduisante. Cependant, le sujet n'est pas aussi simple et l'institution d'une loi de financement des collectivités territoriales aurait tout d'une fausse bonne idée. Non seulement celle-ci risquerait de se retourner contre les collectivités locales territoriales en gros en conférant au gouvernement un nouvel outil de contraintes financières mais elle poserait des difficultés d'articulation majeures avec la loi de 2, finances. Indépendamment du Canada Andrié un tel dispositif impliquerait de sortir du PNF, les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales soit. Un peu plus de 107 milliards d'euros, excusez du peu. La commission des finances pourrait difficilement admettre une telle atteinte au domaine des lois de finances. À l'inverse si on adoptait une solution intermédiaire, et que les transferts financiers de l'État, c'est-à-dire un peu moins de la moitié des ressources des collectivités territoriales continuait à relever des droits de finance l'intérêt supposé. de financement des collectivités territoriales à la portée essentiellement programmatique s'avérerait très limitée. Plutôt qu'une révision constitutionnelle et aux conséquences et à la mise en oeuvre incertaine. C'est à l'édification d'une nouvelle gouvernance et finances locales que nous devrions nous attacher. Une telle évolution est indispensable pour que les collectivités puissent réellement être associé à la préparation des textes financiers qui les concernent. À plus forte raison dans le contexte d'un recours croissant à la fiscalité partagée. Nous avons besoin de repenser les espaces de discussions entre le gouvernement, les assemblées parlementaires et les associations d'élus, comme l'a rappelé la Cour des comptes. Cette nouvelle gouvernance pourrait passer entre autres par une réelle réflexion sur la composition. Et le Champ de compétence du comité des finances locales. Je souhaiterais d'ailleurs connaître l'avis du ministre de et du gouvernement sur ce point particulier mais peut-être à une autre occasion puisque nous avons. Un temps contre s'agissant du second objectif de la proposition de loi constitutionnelle, à savoir le renforcement des exigences de compensation financière des transferts de compétences. Je partage le constat dressé et la proposition qui est faite, la commission des finances avait déjà

déjà adopté une nouvelle adoption de ce dispositif serait donc superfétatoire. à sa mise en oeuvre. Celles-ci supposent un travail d'objectivation des charges supportées par les collectivités territoriales au titre des différentes compétences et qui ne peut être menée que dans le cadre d'une concertation approfondie. Pour toutes ces raisons, la commission des finances a émis un avis défavorable à l'adoption de cette proposition de loi constitutionnelle.

monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le président de la commission des finances. Monsieur le rapporteur pour avis madame la rapporteure pardon monsieur sénateur qui rouge mesdames et messieurs les sénateurs. Je vais être bref pour que tous les inscrits puissent s'exprimer et je vais en conséquence. Accélérer un peu le débit. Qui est le mien. mien. 40 ans. Presque 41 ans, vous l'avez dit tout à l'heure madame la rapporteure. Avec la promulgation de la loi du 2 mars 82 que le mouvement décentralisateur a été engagée. Dans notre pays. Non ce pays dont on sait combien l'histoire politique est ancré dans une tradition. Jacobine. Cette année et très précisément, mardi dernier, c'est la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République qui souffler ses 20 bougies. Voilà donc 20 ans que notre Constitution proclame que l'organisation de la République et décentralisé. je sais que ce que cette proclamation signifie pour votre assemblée dont chacun sait combien elle est attachée à la démocratie locale et à la représentation des territoires ainsi souligné initiative du président Larché, le Sénat a formé un nouveau groupe de travail sur la décentralisation. Représentatif de tous les groupes politiques de cet hémicycle et je veux rendre hommage à cette initiative. Déjà les sujets de préoccupation apparaissent. Le président Larché les a d'ailleurs publiquement évoqué. Il s'agit en particulier des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales et de l'approfondissement de la différenciation territoriale. Le gouvernement et particulièrement à l'écoute des réflexions sur ces sujets. À l'initiative du président de la République. Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les associations d'élus locaux afin d'échanger sur les enjeux d'une réforme institutionnelle notamment en matière d'un renforcement de la décentralisation et de l'autonomie financière des collectivités. Il s'agit de questions délicates. Mais dont les attentes sont claires, plus de clarté dans les compétences exercées plus de proximité dans l'élaboration des solutions et plus de responsabilités aux collectivités à la condition bien sûr de disposer des moyens juridiques et financiers associés associés aux compétences transférées. Les auteurs de cette proposition de loi constitutionnelle tout comme le rapport. De Madame la sénatrice Canayer expose. Me semble-t-il parfaitement les enjeux auxquels les collectivités sont aujourd'hui confrontés. Si le ratio d'autonomie financière des collectivités territoriales. Est aujourd'hui historiquement élevé aux alentours de 70% pour les communes, départements et régions, certaines voix d'élus locaux s'élèvent pour demander davantage de visibilité sur leurs ressources d'autres vont plus loin et appellent à une réforme des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Par ailleurs, alors que l'article 72. De de notre constitution prévoit que tout transfert de compétences doit s'accompagner d'une compensation financière à la nouvelle charge créées à la date du transfert certaines collectivités. Être confrontée à une forte augmentation de la charge que représente. Un transfert Un transfert de compétences en réponse à cette problématique. La proposition de loi constitutionnelle. Monsieur le sénateur Kerrouche a pour objet de créer une loi de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ainsi que de garantir la compensation financière des transferts de compétences en instaurant un vrai examen régulier des ressources transférées. La création d'une loi de financement des collectivités territoriale a été proposée dans le rapport Lambert Malvy d'avril 2014 et dans trois rapports de la Cour des comptes je cite la Cour des comptes, constituerait un instrument efficace au service de la gouvernance des finances locales. Cette loi de financement des collectivités territoriales, aurait pour objectif de déterminer les ressources des collectivités territoriales et de retracer l'ensemble des relations financières des collectivités territoriales, avec l'État. Il est vrai, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'un tel instrument législatif offrirait l'Avantage de garantir un espace de discussion parlementaire consacrée aux finances locales. Mais toutefois, il faut relever qu'existe déjà la possibilité de faire suivre un débat du Parlement. De faire suivre pardonnez-moi d'un débat au Parlement. La remise du rapport prévue à l'article 7. De la LOLF, qui porte sur la situation des finances publiques locales sur l'évolution de leurs charges et de leurs dépenses et sur les conséquences du projet de loi de finances sur celle-ci. Ce débat a eu lieu pour la première fois lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023. En outre, il faut prendre en garde. Les conséquences concrètes d'une telle réforme pour le débat parlementaire. En effet le champs. De ces lois de financement. Des collectivités territoriales seraient exclusif de celui des lois de finances. Or de nombreux sujets Antunes. Implication budgétaire au niveau national et et au niveau local font par exemple la hausse de la dotation globale de fonctionnement ou la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises opéré en 2023, plus une comme l'autre ont des conséquences fini financière pour l'État, comme pour les collectivités et nécessiterait d'être abordée lors de l'examen de la loi de finances, comme lors de l'examen d'une loi de financement des collectivités serait-il alors judicieux dans ces circonstances de scinder dans 2 véhicules distincts. Les aspects nationaux et les aspects locaux serait-ce même possible À l'information du Parlement dans un calendrier budgétaire encore plus restreint par l'examen de 3 textes financiers Il n'est tout simplement pas certain comme l'ont très justement souligné les travaux de la commission que ce nouvel instrument soit adapté à l'objectif. Que nous partageons tous, à savoir donner aux collectivités une visibilité à une protection financière suffisante pour la réalisation de leurs actions. La seconde mesure de cette proposition de loi consiste à réviser les règles de compensation financière des transferts de compétences afin d'y introduire un mécanisme de re-examen périodique. Tout d'abord, j'observe que le principe de libre administration des collectivités territoriales prémuni déjà les collectivités contre une dégradation excessive de leur situation financière, du fait de l'évolution de leurs charges. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de l'affirmer dans 2 décisions du 30 juin 2011. Les mécanismes de compensation doivent être suffisant. Pour que ne soit pas entraver la libre administration des collectivités concernées par ailleurs dans un objectif de bonne gestion des finances publiques. La capacité des collectivités locales à financer les compétences transférées, doit pouvoir s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs ressources et de leur dynamisme et pas uniquement à l'aune des recettes directement affecté lors du transfert historique de compétence. Enfin, la comparaison entre le niveau des ressources et de dépenses transférées poserait de grandes difficultés méthodologiques, l'évolution ultérieure. Du niveau de dépenses des collectivités dépend des circonstances nationales mais également des choix de gestion de la collectivité locale. Une telle mécanique induirait entre l'État et les collectivités. Un examen de l'exercice. De chaque compétence au niveau global. Mais ensuite inévitablement aussi au niveau individuel, or les choix une collectivité de porter l'effort sur une telle compétence ou telle autre sont consubstantiels à la libre administration vous l'avez compris, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement n'est pas favorable. En l'état. À cette proposition de loi constitutionnelle et je veux être très clair. Les pistes qui sont avancés ne sont pas à balayer d'un revers de main, loin de là. Mais elle semble pour l'heure soulevé plus d'interrogations. Que de solutions surtout cette proposition de loi intervient dans un contexte où. Un bilan plus large pourrait être dressé en matière de. Décentralisation les problématiques dont cette proposition de loi se saisit sont réelles mais ce ne sont pas les seuls président Larché évoquée, celle de la différenciation des collectivités territoriales. C'est un sujet que le gouvernement avait souhaité porter avec le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique mais la réflexion doit se poursuivre en témoigne d'ailleurs les travaux en cours au sein du Sénat. Par le groupe de travail transpartisan évoqué au début de mon intervention ainsi que les travaux initiés par le président de la République avec les associations d'élus locaux sur ce sujet comme sur les autres. Le gouvernement sera bien sûr particulièrement attentifs à la restitution des conclusions de ces groupes de travail. 20 ans après la décentralisation. Nous avons connu l'apparition dans notre. Dont L'apparition dans notre Constitution. Il faut poursuivre notre réflexion commune. Pour nos collectivités territoriales afin qu'elle puisse exercer pleinement leur mission au service de nos compatriotes. Merci la parole Madame Pentel pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues. La proposition de loi constitutionnelle de nos collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain n'est pas la première du genre, on peut citer en particulier la proposition de loi constitutionnelle adoptée par le Sénat en 2020. Nous saluons toutefois cette nouvelle initiative et qui est aussi l'occasion de débattre des finances locales et des options qui permettraient d'améliorer leur cadre légal. Ceux-là viennent notamment un complément des travaux de la mission d'information sur l'impact des décisions réglementaires et budgétaires de l'État sur l'équilibre financier des collectivités locales d'un j'ai l'honneur d'être rapporteure depuis le 1er mars. Contrairement aux administrations de l'État et de la sécurité sociale les administrations publiques locales ne font en effet pas l'objet d'une loi de financement. Didier et qui examiné chaque année au Parlement. Les mesures de financement des collectivités sont actuellement disséminés dans le PNF hein. Première partie avec la fixation du montant des dotations et les impositions transférer et 1 seconde partie avec les crédits de la mission Relations aux collectivités territoriales et la répartition de ces dotations. Il est vrai que le principal obstacle à une telle loi de finances maintient peut être à la Constitution elle-même qui consacre un son article 72, la libre administration des collectivités territoriales. C'est pourquoi le volet dépenses de la loi de financement ne pourrait avoir qu'un caractère indicatif. Toutefois, elle aura le mérite de mieux distinguer ce qui relève des finances de l'État et des finances locales. Nous saluons aussi le 2ème axe de la proposition de loi qui vise à renforcer le principe déjà présentes dans la constitution de compensation financière des transferts de compétences dans le temps. c'était permettrait sans doute un meilleur suivi et un meilleur contrôle de ces compensations. De surcroît, je m'aperçois qu'il s'agit de d'une véritable revendication de la part des associations d'élus. Que nous auditionnant dans le cadre de la mission d'information. Un fait le transfert de de dispositions du PLF vers le PLF c'était ne devrait-il pas s'accompagner d'une réduction équivalente des délais d'examen du PLF afin de conserver un ordre du jour réalisable à l'Automne. Il faudrait d'ores et déjà anticipé les dispositions qui pourraient contenir cette future loi organique, il faudrait un particulier veiller à ce que les lois de financement des collectivités améliorent la prévisibilité de leurs recettes sans pour autant devenir une forme de tutelle gouvernementale. Ces observations faites-le. Les membres du groupe RDSE voteront en faveur de cette proposition de loi constitutionnelle dans le rejet la semaine dernière un commission et probablement aujourd'hui un séance nous apparaît davantage liée à des considérations politiques que techniques. Merci. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances. Mais madame et monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. L'idée d'une loi annuelle de prévision des dépenses des collectivités territoriales ne date pas d'hier, les premières propositions remonte, on l'a dit au mois d'avril 2014 lorsque Martin Malvy, Alain Lambert avait formulé ses propositions dans un rapport intitulé pour un redressement des finances publiques fondée sur la confiance et l'engagement de chacun. Force est de constater que quasiment 10 années plus tard. Ce constat de défiance entre l'État et les territoires est resté le même. Il est à rappeler pourtant que le Conseil constitutionnel s'efforce de consacrer à jurisprudence constante, l'exigence de protection de l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Dans une décision de du 24 juillet 91 les rappelait déjà à titre d'exemple, que les ressources des collectivités ne doivent pas être être réduite au point d'entraver leur libre administration pourtant plus de 30 années plus tard la voilure de ces ressources n'a cessé de se recroqueviller sur elles-mêmes. Les collectivités décentralisées n'ont pu qu'observer avec impuissance leurs ressources fiscales et budgétaires fondent comme neige au soleil sans que les compensations ne viennent véritablement corriger les pertes subies. Après la baisse de la DGF, la suppression de la TH et de la CVAE ou la révision prochaine des valeurs locatives cadastrales. Les communes ont souvent d'autre choix que de répercuter la compensation manquante sur la fiscalité des particuliers ou bien d'accélérer les coupes budgétaires grande ainsi la tentation pour le législateur de canaliser les velléités de recentralisation de l'État, c'est le cadre juridique nouveau que propose la proposition de loi de notre collègue Éric Kerrouche suggérant la création d'une loi de financement des collectivités territoriales et de leurs regroupements. Certes, donner une existence constitutionnelle a une nouvelle loi de finances spécial serait l'opportunité de mettre fin à l'émiettement des versements de l'État aux collectivités et à la faible lisibilité qui en résulte un émiettement entre budget général prélèvement sur recettes et compte spéciaux qui conduit à des débats parlementaires distinctes et donc à des votes séparés et pesant in fine et sur l'exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Une loi de financement des collectivités consacrerait ainsi la place des administrations publiques locales de le triptyque institutionnel et financier de notre pays aux côtés de l'État et du système de santé. Il apparaîtrait toutefois que l'intention originelle de notre collègue si louable qu'elle fut pour nos territoires doivent se heurter au cadre constitutionnel existant et que celui-ci Vienne compromettre l'objet même poursuivis par la proposition de loi car c'est pas ce que c'est à leur adoption qui est conditionné le fonctionnement même de notre service public et de nos institutions que les lois de finances offre au gouvernement impuissant Arsenal en complément de celui offert par les lois ordinaires. Enchâssées le financement des collectivités dans le cadre de la LOLF. C'est offrir au gouvernement une opportunité de faire usage du 49.3 à autant de reprises qui le jugera nécessaire. C'est aussi lui accorder le droit d'atrophier les temps du débat le fondement de l'article 47 s'est laissé au gouvernement. Dans le cas d'une procédure parlementaire qui excéderait les délais prévus par la Constitution la possibilité de légiférer par ordonnances et ainsi de conserver toute sa mainmise sur les versements aux territoires de leur montant et leur ventilation c'est ouvrir la perspective de loi de financement rectificative de lois, de règlements des collectivités et de démultiplier ainsi les véhicules législatif au cours desquels ces outils constitutionnels pour être, être, être activé. Bien davantage qu'un nouveau souffle à apporter au principe d'autonomie des collectivités. C'est plutôt un nouveau carcan qui pourrait leur être imposé. Si l'objet de la démarche est de garantir que le Parlement puisse tenir un délai un débat annuel sur les dépenses des collectivités. Qu'à cela ne tienne, nous pourrions tenir ce débat dans le cas d'une loi d'orientation et de programmation. Cette option aurait d'ailleurs l'Avantage d'être plus vertueuse et moins contraignante et s'articulerait avec sagesse avec le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012. Par ailleurs, fédérer dans le PLF toutes les contributions de l'État au sein d'une mission budgétaire unique serait une immense valeur ajoutée pour la lisibilité de notre, de nos comptes et le suivi des transferts de compétences, nombre de nos collègues l'emporter à de maintes reprises à cette tribune. Nous avons besoin d'un séisme institutionnel pour nos territoires et je ferais à ce propos bien les propos du président Gérard Larché qui avait défendu pour les finances locales. L'objectif de ressources stables et planifié une évaluation régulière des compensations et d'une contractualisation bâtie sur le consensus un État trop jacobin aura raison de la démocratie locale, sauf à ce que le Parlement lui donne les conditions de s'épanouir chers collègues sénateurs continueront à donner à cette démocratie locale les moyens de son épanouissement. Notre groupe s'en réfère à bien sûr à la ville. La commission, il ne votera pas cette proposition de loi, même si elle en salue vivement à l'intention je vous remercie. Merci la parole est maintenant Emmanuel Capus pour le groupe les indépendants, autrefois.

Madame la présidente. Monsieur le ministre. Mes chers collègues. Je vais essayer d'aller vite effectivement, j'ai compris qu'on était contraint. En raison de léger cafouillage dans les votes du du texte d'avant nous n'y sommes pour rien. Dans un contexte incertain, les élus locaux sont inquiets. Ils craignent de ne plus pouvoir agir sur le terrain. Or, c'est pour cela que les élus locaux s'engagent. Pour agir sur le terrain. Avec l'inflation qui renchérit le coût des projets. Les récentes évolutions de la fiscalité locale et la crise démocratique qui dévalorise leur statut. Les élus locaux se sentent. PC. Ils ont donc besoin de sécurité. C'est notre rôle au Sénat de leur apporter ces éléments de sécurité. Sans aucun doute cela passe en partie par les finances locales. C'est pourquoi cette proposition de loi constitutionnelle a le mérite de poser un sujet essentiel. L'autonomie financière des collectivités locales. À cette question. Nos collègues socialistes apporte une réponse. Créer une nouvelle catégorie de loi de financement. L'objectif. Intéressant et de formaliser de façon lisible et transparente les relations financières entre l'État et les collectivités. L'idée n'est pas nouvelle, elle a souvent été évoqué dans cet hémicycle à droite comme à gauche. La Cour des comptes aussi a soutenu dans plusieurs de ces rapports. Nul doute que le serpent de mer continuera de faire parler de lui, tant que nous n'aurons pas purgé le débat. C'est pourquoi une clarification est nécessaire et bienvenu. Notre groupe considère toutefois qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. Cette nouvelle loi de financement aurait immanquablement est fait pour effet de renforcer la dépendance des collectivités vis à vis de l'État. Nous pensons donc. Quel pourrait être contreproductives. On a déjà rappelé les récentes évolutions de la fiscalité locale. Notamment la suppression de la taxe d'habitation et la CVAE. Ces réformes continuent d'interroger les collectivités. Je ne veux pas refaire les débats ici que nous avons déjà eu en loi de finances et j'ai indiqué que j'allais accélérer mais je veux tout de même rappelé l'objectif de ces réformes supprimer des impôts injustes. que son mon pardon parce que son montant ne dépendait pas des revenus. La CVAE parce qu'elle pénalise les entreprises industrielles et donc le tissu économique des territoires. La compensation de ses impôts. Par affectation d'une fraction de TVA doit permettre aux collectivités de bénéficier. De ressources pérennes et dynamiques. Ces réformes doivent précisément sécurisé les ressources. Des collectivités. Certes. Avec une loi de financement spécifique. Les compensations apparaîtrait peut-être de façon plus lisible. Mais de problèmes majeurs se poserait encore. D'une part, mes chers collègues. Examiner les flux financiers entre l'État et les collectivités. Sans discuter, en même temps des impôts qui affecte l'économie 7. Analyser la dépense sans la recette et donc réduire les collectivités à des postes de coup. D'autre part raisonner en grand agrégats. Ne donne aucune garantie sur des cas particuliers et ne saurait rassurer les élus. Ainsi. Une telle loi de financement examiné à la hussarde entre le PLF et le Plfss risquerait d'appauvrir les débats sur les finances des collectivités, elle renforcerait une gestion nationale et centralisée des problématiques locales, ce n'est pas notre vision d'une république décentralisée qui fait confiance à ses élus locaux pour changer les choses sur le terrain, je vous remercie.

la présente, proposition de loi pour objectif de sécuriser les relations financières entre État et collectivités et de donner de la lisibilité dans les flux de compensation des transferts de compétences dans le temps. Les auteurs de la PPL, c'est que nous étudions souhaité répondre aux demandes des élus locaux et aux réflexions poussées de la Cour des côtes à l'heure de l'urgence climatique, le manque de lisibilité et de visibilité et de transparence que les que les collectivités pour les collectivités de leurs ressources, en particulier celles émanant de l'État freine la réaction pourtant essentiel pour le quotidien de leurs administrés. Comme pour l'avenir de notre pays dans sa globalité, c'est essentiel pour permettre aussi une articulation local des stratégies nationales. La création d'une loi de financement des collectivités territoriales, était une des mesures portées par le candidat Yannick Jadot lors de l'élection présidentielle afin de porter un approfondissement de la décentralisation dans un triple direction plus de démocratie, plus de justice territoriale plus d'écologie et si elle constituerait un outil de meilleure information des citoyens et des élus et en définitive de responsabilisation de l'ensemble des acteurs de l'équilibre des finances publiques locales. Il s'agit là dans le jeu important au moment où les collectivités territoriales doivent réaliser des investissements massifs dans la transition écologique. Nous apporterons donc notre soutien à cette proposition, tout en restant vigilant aux modalités de sa mise en oeuvre et d'une mise en oeuvre d'une avancée nécessaire qui pourra d'ailleurs être complétée par les travaux des groupes, présidés par le président Larquier. Merci monsieur Bargeton pour le groupe Rassemblement démocratique. Progressiste et indépendant. Vous avez la parole. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre mais. Mesdames et messieurs, chers collègues. Alors cette idée. D'une loi de financement des collectivités territoriales. Reprend un amendement que notre collègue Kerrouche avait déposé à à la proposition de loi de Philippe Bas sur les libertés locales. À l'époque d'ailleurs le rapporteur Mathieu Darnaud s'y étaient opposés. De même, que s'est opposé. Le groupe de travail mis en place par Gérard Larché, qui n'a pas repris cette cette proposition d'ailleurs une partie des propositions consistait à mettre en place plutôt un débat, une sorte de débat d'orientation des finances locales et cette proposition a été reprise dans la modification de la loi organique relative aux lois de finances qui est intervenu sous l'égide de Éric Woerth et de Laurent Saint-Martin lors du précédent quinquennat et donc a été repris l'idée était reprise l'idée d'un débat mais mais pas plus. Bon il y a déjà beaucoup d'arguments qui ont été avancés contre cette proposition. D'abord je trouve paradoxal et étrange de la part de. Souvent de parlementaires qui s'oppose à l'idée de contractualisation de d'aller plus loin avec une loi de financement. Si on refuse le le première, la première étape. Pourquoi vouloir aller plus loin, à la rigueur je dirais qui peut le plus peut le moins. vous vous êtes souvent opposé la contractualisation ensuite cette loi donnerait un dernier mot à l'Assemblée nationale. Je suis pas sûr que le swing, le Sénat souhaite que il y est finalement comme pour les textes budgétaires, une prépondérance de l'Assemblée là-dessus et puis la comparaison avec les lois de financement de la Sécurité sociale. et périlleuse et dangereuse, en tout cas le mérite d'être. Parce que lorsque ça a été mis en place en 96, c'était pour rétablir l'équilibre financier de la Sécurité sociale. Et d'ailleurs notre collègue Lefèvre a bien parlé d'un risque de carcan. Je suis pas sûr non plus que ce soit ça l'esprit de la loi mais qu'en ferait un législateur une fois que vous avez créé cet outil un législateur lauréat disposition et pourrait en faire ce qu'il faut, il faut donc être à mon avis, extrêmement prudent en la matière. D'autres éléments peuvent aussi expliquer que nous ne sommes pas favorables à cette disposition, même si il y a des idées dans dans ce qui a été exposés qui sont intéressantes. Le 2ème point. On le sait c'est l'idée de garantir les. Transferts de compétences aux collectivités locales d'un point de vue financier, alors. Je ne peux pas partager vous comprendrez certain nombre d'éléments qui ont été posées, la Cour des comptes rappelle en 2021 que. Les recettes locales sont beaucoup plus dynamique que les dépenses et c'est ce qui explique d'ailleurs 4 7 milliards d'excédent. Et d'ailleurs la Cour des comptes rappelle dans ce rapport que seul l'État et la secrétaire et sociale ont participé à la gravement de du déficit public et que pour les collectivités locales c'est zéro 15 points alors c'est zéro 15 points mais c'est rien du tout par rapport au déficit public en général de 2022 1021 notamment liées au Covid et pourquoi parce que ça n'a pas été rappelée. Mais désormais les transferts aux collectivités locales sont adossés à la TVA qui est un impôt qui a montré son dynamisme et qui dans un contexte de croissance maintenue montre encore son dynamisme. Bien sûr ça peut varier. Ça peut changer mais pour l'instant le choix de l'adossement à la TVA a finalement été un choix dynamique pour les recettes des collectivités locales. Je ne reviendrai pas non plus je ne serai pas taquin pour rappeler quand même que dans un précédent quinquennat il y a eu 11 milliards de baisse sous François Hollande pour les collectivités locales après un milliard et demi en 2015 et que l'enveloppe normée a été créée pour la DGF en 2016 la DGF, nous l'avons sanctuarisé, et nous l'avons même ajouter 320 millions l'an dernier. Il faut donc quand même rappeler ce 4 budgétaire d'ensemble. Je ne reviendrai pas, faute de temps sur le filet de sécurité. Le bouclier tarifaire, la charte pour les fournisseurs tous les dispositifs qui ont mis étaient mises en place pour faire face à l'inflation que subissent aussi les collectivités locales, enfin les remarques et les réserves exprimées par notre collègue. Me semble de bon sens sur le fait que il y a quand même la liberté des collectivités locales qui s'oppose à ce que on puisse finalement venir pour voir comment est dépensé l'argent pour La parole est à Cécile Cukierman. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues. Tout d'abord dire peut-être le sentiment de frustration, puisque pour un débat effectivement aussi important mais c'est la règle des niches parlementaires nous allons avoir un débat tronqué. Un débat qui nécessiterait très certainement le temps le temps des explications. Le Temps des échanges pour répondre et effectivement et et j'en remercie les collègues du groupe socialiste d'avoir déposé ce texte qui répond à une exigence de l'ensemble des élus locaux qui est celui du financement des collectivités territoriales qui souffre aujourd'hui cruellement de moyens. Depuis plusieurs années sur l'été rappelé et auxquels s'ajoutent et là aussi sur l'a été rappelé les multiples crises que nous traversons depuis maintenant quelques années. Alors si la création d'une loi de financement peut paraître séduisante, il nous semble que ce qu'attendent avant tout et surtout les élus locaux, c'est aujourd'hui plus de prévisibilité plus de visibilité pour pouvoir mieux anticiper et ainsi bâtir leur budget et répondre par les différences dépenses d'investissement et de fonctionnement aux besoins des populations. Nous craignons que la la l'article tel qu'il a été rédigé renforce finalement le caractère autoritaire de l'État sur la gestion des collectivités territoriales. Elles ont actuellement besoin de 100 milliards d'euros pour assurer pleinement leur mission de service public, c'est à ce défi-là qu'il nous faut répondre et encadrer les dépenses ne permettra pas de combler les décennies de désengagement de l'État. La libre administration des communes peut être remise en cause, elle ne dispose plus des ressources propres et dépendent. Donc davantage du bon vouloir de l'État. taxes et impôts qui ont été supprimés. Ces dernières années mais aujourd'hui à l'échelle communale. La taxe foncière demeure l'unique recette La multiplicité cela vient encore d'être dit des taxes dans notre pays. Est importante et je redis ici ce que j'ai dit ailleurs, le problème de notre pays, c'est très certainement celui que nous payons trop de taxes mais pas assez d'impôts. Une loi de programmation pour les collectivités territoriales nous aurait semblé et il nous semble beaucoup plus approprié plus pertinente pour répondre aux enjeux de financement mais aussi de visibilité de transparence qu'attendent les élus locaux. Pour que c'est le débat budgétaire soit également plus efficace, il serait judicieux de prévoir un temps de débat dans la loi de finances sur les finances locales qui ne Perrin ne permettrait pardon. Une forme de recollement. Des différentes recettes et dépenses affectées aux collectivités territoriales, nous pourrions également proposé la création d'un jaune budgétaire qui permettrait de regrouper toutes les données relatives aux dépenses de l'État et instaurer plus de transparence. Le 2ème. Objet de cette proposition de loi et celui du transfert des compétences. Transfert de compétences nombre, parfois qui se sont opérés sans compensation. En tout cas sans compensation à l'euro près ni même d'ailleurs la volonté des élus Et en l'état. Vous l'aurez compris, nous aurions aimé avoir un débat sur chacun des articles. Nous allons donc retirer les interventions sur l'article prévu pour permettre à ce texte d'aller au bout. Nous aurions aimé. Exprimer les raisons d'un votre compte sur l'article hein mais je crois que je je viens d'expliquer. sur l'article 2 et en l'état et au vu de. Ces votes un fixe primer sur les articles parce que y compris, nous pensons que créer une loi de financement viendrait appliquer y compris le fameux 49 3 sur les collectivités territoriales, nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi, je vous remercie. Merci madame Françoise Gatel pour le groupe Union centriste. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le Président Madame et messieurs les rapporteurs dont je salue le travail. Je salue aussi l'initiative de notre collègue Éric Kerrouche qui met le projecteur sur un sujet essentiel et parfois existentiel du financement des collectivités locales et leurs groupements mon cher collègue. Votre constat est pertinent et largement partagée. Alors que la conduite de l'action publique nécessite lisibilité sécurité et visibilité. Elle est soumise à des convulsions budgétaire à l'émiettement des financements et un dérapage du coût des compétences transférées du à des rajouts de normes à l'insu du plein gré si je puis dire des collectivités. Tout ceci donne donc une lisibilité très flou. Or, on le dit, quand c'est flou, il y a un loup. Mes chers collègues. Kerrouche. Je pense que votre proposition de loi elles-mêmes contient Alou. Si l'autonomie financière que vous souhaitez servir. Est une composante du principe constitutionnel préexistants de libre administration, force est de constater, vous avez raison les limites du principe, encore une fois votre diagnostic est bon mais le remède que vous prescrivez ne l'est pas, me semble-t-il. Il relève d'une bonne intention mais qui comme souvent risque de paver l'enfer des collectivités. En effet, une loi de financement des collectivités ressemble fort à la loi de financement de la Sécurité sociale. Doit-on ici rappeler l'objectif et l'effet d'une telle loi, qui est de plafonner des dépenses par un indice. Je ne doute pas mon cher collègue Éric Kerrouche du succès de votre PPL auprès de Bercy et de la Cour des comptes. Pardonnez-moi mais vous réinventer les contrats de Cahors 6 léonins et créer ainsi un piège qui se refermera sur les collectivités, ça n'était pas votre intention mais c'est l'effet. L'article 2 de la PPL propose la rénovation des modalités de compensation financière des transferts de compétences selon le principe cher au Sénat de qui décide paye. Nous ne pouvons qu'adhérer à la révision du coup des transferts toujours victime de nouvelles obligations qui s'agrègent au fil du temps. Cette disposition est si pertinente, vous le savez bien, qu'elle a déjà été adopté par le Sénat en septembre 2020 et attend patiemment dans l'antichambre de l'Assemblée d'évoluer. Par ailleurs, des travaux en cours au Sénat. Je parle de la mission d'information du RDSE sur l'impact des décisions réglementaires de l'État sur l'équilibre financier dont je salue la rapporteure notre collègue Guilaine Pentel. Le groupe de travail transpartisan conduit par le président Larché, dont le président de la commission des Lois L rapporteur général contribueront sans aucun doute approfondir et structurer la réflexion du Sénat autour des exigences que vous évoquez sécurité visibilité cher Éric Kerrouche vous l'avez compris, le groupe centriste aime beaucoup votre diagnostic mais n'aime pas du tout votre prescription et donc rejettera ce texte, je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux. Moi aussi je vais être très bref. J'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle qui n'est pas identique. C'est le moins qu'on puisse dire à celle de notre collègue Kerrouche

ce qui me gêne un petit peu, je le dis franchement c'est que. Nous souhaitons tous insisté sur l'autonomie fiscale et financière, et je suis toujours inquiet par rapport à des gouvernements impécunieux qu'ils soient de gauche ou de droite, sur le fait que si on met un peu trop la marque sur il faut faire en sorte que les compensations soient à l'euro près, il s'empresse de dire pas de problème on va transférer et et on va compenser ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs par la suite. Moi je préfère évidemment qu'on se batte davantage sur l'autonomie fils fiscale et financière, c'est-à-dire sur le fait que les collectivités continue de disposer d'impôts locaux réel avec de véritables rentrées financières et ne soit pas sur la ligne de se dire que finalement on va de plus en plus dépendre de l'état de ses dotations parce que ces dotations, on l'a bien vu quelles que soient les gouvernements, de. Ans la en la matière qu'qui soit de gauche ou de droite quand tu. Le budget va bien ça va encore quand le budget n'est pas terrible. Et ben les collectivités locales sont la variable d'ajustement parce que c'est tellement plus facile. La vérité. Tout de même. J'entends bien tout ce qui est dit sur il ne faut pas l'inscrire dans la Constitution la vérité quand même c'est que. Beaucoup d'associations, je pense à l'association des maires d'Île-de-France mais à d'autres sont favorables. Pourquoi. Sont favorables à l'idée, peut-être pas un tel ou tel texte. Mais à l'idée pourquoi parce que quand on nous dit oh la la mais attendez si vous mettez ça dans la Constitution, vous rendez pas compte de la contrainte. La seule chose dont je me rends compte c'est que les gouvernements de gauche ou de droite qui ont supprimé la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la CVAE Laurent fait sans avoir le moindre état d'âme par rapport aux collectivités locales sans débat. Sans rien du tout, ça a été comme ça. Bonjour. Et par exemple pour la, la, la dernière en date. Bon c'est c'est souvent des engagements dans des campagnes électorales ou de désengagement politique mais qui ne sont pas réellement débattu sur le fond au Parlement. Donc moi je propose monsieur le garde des Sceaux alors vous n'êtes pas un ministre du Budget, vous ne pouvez pas avoir tous les postes mais. Je, je propose qu'on on travaille. Alors il y a déjà des groupes mais moi je dis à mon collègue qui est, je ne vais pas voter sa proposition parce que bon je suis un peu gênée par l'article 2 et le sous-entendu que cela pourrait vouloir dire par rapport à l'état. Pourrait faire une proposition commune. Peut être à travers les présidents de groupe peut être à travers. Le groupe K que préside Gérard Larché, mais il faut qu'il y ait une proposition commune. Est-ce que ça doit être dans la Constitution. À mon avis oui puisque ce serait. Clairement établie dans le budget, mais si ça ne l'est pas, qui a en tout cas une solution pour que les collectivités locales ne se retrouve pas seule systématiquement face au pouvoir exécutif. Il faut trouver une solution pour que il y ait. Une structure liée un texte qui est quelque chose qui fasse en sorte que les uns ou les autres ne se sentent pas dépossédés de leurs pouvoirs mais que l'on renforce les collectivités je vais arrêter là puisque montant va être contraint mais en tout état de cause moi je me battrai pour l'autonomie fiscale. Ça veut dire pour qu'on laisse

Merci Monsieur le Président, Karoutchi donc que la discussion générale est Close. La commission n'ayant pas élaboré de texte nous passons l'addition des articles de la PLC initial. Alors nous commençons par l'article 1 que je vais donc de ce pas métro voix qui est pour.

Oui merci madame la présidente. Alors actuellement, mes chers collègues, l'interprétation de l'article 40 de la Constitution. Nous empêche empêche le Parlement de formuler des propositions et des amendements dont la finalité est d'opérer des transferts de compétence. Entre les collectivités territoriales. Aussi la répartition des compétences entre les collectivités est-elle l'apanage aujourd'hui du gouvernement. Le Parlement et singulièrement le Sénat. Représentant les collectivités est ainsi totalement empêché et ne peut être force de propositions en matière de transferts de compétences. En effet, comme le précise le rapport d'information commis par le président Marigny en 2014 qui fait encore référence en matière d'application de l'article 40, les transferts de charges doivent être analysé comme la création d'une charge pour une personne publique compensée par la diminution d'une charge pour une autre personne publique. Cela concerne aussi le transfert de compétences entre collectivités. Les amendements et propositions doivent donc être à cet égard considérée comme irrecevable, aujourd'hui. Et ce rapport précise également que cette interprétation correspond à une jurisprudence constante de l'Assemblée nationale comme du Sénat, renvoyant à une décision du Conseil constitutionnel de 1976. mes chers collègues, cette jurisprudence méconnaît gravement le fait que tout transfert de compétences entre les collectivités s'effectue, eu égard à l'article 72 de la Constitution dans le respect du principe de neutralité budgétaire. Quand on transfert d'une collectivité à une autre on transfère la compétence on transfère les charges ça ne transfère aucune charge. Cet amendement vise donc ça ne crée aucune charge cet amendement vise donc à préciser que l'article 40 de la Constitution ne s'applique pas aux propositions et amendements parlementaires prévoyant des transferts de compétence et donc de charges entre collectivités afin de renforcer la place de l'initiative parlementaire et singulièrement la place de l'initiative sénatoriale dans l'organisation décentralisée des compétences locales. locales. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Oui. Monsieur le sénateur Capu vous souhaitez prévoir Sans ambiguïté. Un cas de dérogation. À l'article 40. Plus précisément, vous souhaitez que. Que les, les propositions de lois ou amendements tendant à prévoir des transferts de compétences entre collectivités territoriales ne puisse pas faire l'objet d'une déclaration dirait de. En l'état du droit, l'article 40 s'oppose sans ambiguïté à un transfert de compétences entre personnes publiques dans la mesure où ce transfert de se traduira forcément par une création de de charges pour la personne destinataire. Pour autant, les présidents successifs des de la commission des finances ont adopté à cet égard une jurisprudence particulièrement favorable à l'initiative parlementaire sont ainsi considérées comme recevables les amendements se bornant à redistribuer le poids d'une même charge au sein d'une même catégorie de collectivités notamment entre. Les communes et les EPCI. Il en va de même pour les délégations de compétence y compris entre collectivités relevant de strates différente dans la mesure où la compétence demeure juridiquement à la collectivité d'élégantes. donc nous ne sommes pas favorables, surtout qu'. Cela paraît fort peu opportun d'introduire dans un texte constitutionnel au détour de cette. Proposition de loi constitutionnelle un dérogations unique à l'article 40 pour les seuls transferts de compétences entre collectivités territoriales. Selon vous ouvrirez en effet la porte à un débat sans fin sur la mise en place d'exception sectorielles. À la règle commune. Donc nous sommes défavorables. Que des avis du gouvernement. Vie que la commission, madame la présidente. Si monsieur le garde des Sceaux. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu Monsieur capuche. Pardonnez-moi.

Ont été jugés irrecevables Arctique 40. Au motif qu'ils étaient sensé créer une charge il manquerait aucune vous transférer par exemple la compétence écoles de la commune au département ou de la compétence collège. Au à la région à la région et réciproquement. Vous ne crée aucune charge pour l'État. Je veux dire vous avez une compétence qui est transféré d'une collectivité à une autre. C'est totalement neutre et c'est d'ailleurs ce que prévoit la Constitution. C'est totalement neutre constitutionnellement. Donc il me semble que ça ne crée aucun risque financier pour l'État. C'est totalement neutre et je veux dire c'est quand même se tirer une balle dans le pied nous sénateur. De considérer que le fait de de de nous priver de pouvoir transférer une compétence d'une collectivité à une autre, c'est quand même notre rôle, on est les représentants des collectivités territoriales. Il me semble qu'il n'y a à la fois aucun risque financier. Et qu'il y a une parfaite logique à inscrire dans la Constitution le fait que le Sénat. L'Assemblée et l'Assemblée nationale. En tous les cas le Parlement dans son ensemble peut parfaitement transférer une compétence à partir du moment où c'est neutre. Je suis de revenir sur une interprétation beaucoup trop rigoriste. À mon avis. De. L'article 40. Voilà. Merci je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mais maintenant on voit l'article 2 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je vais. Mettre ensuite la proposition de loi. Consensuel au vote par scrutin public puisque c'est de droit y a-t-il des demandes d'explications de vote et je voudrais, avant de donner la parole éventuellement d'appeler au scrutin remercier l'ensemble de des collègues présents ici, qui ont été extrêmement bénévoles en pour tenir les délais. Et le garde des Sceaux. Si bien sûr je remercie aussi le garde des Sceaux. Voilà. Qui s'est restreint. Y a-t-il des explications de vote. Non, je n'en vois pas donc le scrutin. Est ouvert.

c'est bon. Plus personne ne demande à voter Le scrutin est donc clos. Votants 343 exprimés, 324 pour 86 contre 238, le Sénat n'a pas adopté j'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte. Sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la couvert ce professionnel de santé est parvenu à la 200 un texte commun. Je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu mardi 11 avril à 14h 30 pour le débat sur le thème l'avenir de la ressource en eau, comment améliorer la gestion. Et la séance est levée.